La séance est reprise, l'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle. Toujours du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 et dans la discussion générale, la parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Madame Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure générale de la commission des affaires sociales, mesdames et messieurs les rapporteurs. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Le retour du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2023 en seconde lecture devant votre assemblée, me donne l'occasion au nom du ministère des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées et du ministère de la Santé et de la prévention dans saluer l'importance et l'ambition. L'importance pour nos concitoyens de tous les âges et de toutes les situations de vie l'importance pour les professionnels qui les accompagnent des premiers, au dernier jour de la vie, à fortiori dans le contexte d'incertitude et de tension que nous connaissons l'inflation, les pénuries de professionnels et les doutes quant aux grandes transformations en cours se ressentent dans de nombreux secteurs. Et le texte dont vous reprenez l'examen constituent une part de la réponse ambitieuse du gouvernement en la matière. Le 1er rôle du PLFSS c'est d'abord de financer. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'Ondam est ainsi proposé à un niveau historique de 3,7 % hors dépenses de la crise sanitaire. Cette augmentation conséquente s'inscrit dans la droite ligne de l'effort d'investissement que nous avons réalisé ces dernières années, notamment avec le Ségur de la santé. Pour soutenir l'hôpital face aux épisodes hivernaux nous ajoutons un milliard d'euros pour l'année 2022 comme voter au sein de cette chambre cela s'ajoutent aux 543 millions supplémentaires pour faire face au surcoût de Covid adopté à l'Assemblée. Grâce aux sénateurs, et notamment à la rapporteure Imbert ce texte sécurisent la garantie de financement pour le second semestre 2022. Pour 2023, à l'Assemblée nationale a créé un dispositif transitoire de financement des hôpitaux afin de permettre un retour progressif à la normale. Nous n'oublions pas la médecine de ville alors que la négociation conventionnelle s'ouvre, elle fait aussi l'objet de toutes nos attentions mais nous ne perdons pas de vue nos responsabilités après la crise, ce PLFSS entend garantir la soutenabilité de la sécurité sociale, c'est pourquoi des mesures d'économies juste et proportionnée sont demandés à la radiologie ou à la biologie. En ce qui concerne le secteur médico-social, l'Ondam accompagnera de 5 1 % contre 4,3 en 2022, pour atteindre 30 milliards d'euros, ce sont près de un milliard et demi d'euros de financements supplémentaires. Avec notamment 600 millions d'euros dédiée aux revalorisations salariales, c'est-à-dire aux suites du Ségur et de la conférence des métiers, ainsi qu'à l'augmentation du point d'indice dans la fonction publique et son extension au secteur privé. 500 millions d'euros pour le soutien de l'accueil à domicile avec la réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile et la création de places pour réduire les refus de prise en charge auquel certaines personnes sont confrontés. 200 millions d'euros pour recruter des soignants ah Nepad ce qui nous a inscrit dans la trajectoire annoncée de recrutement de 50000 professionnels sur les prochaines années et enfin plus de 200 millions d'euros de compensation de l'inflation. Réponse ambitieuse, donc avec des moyens financiers conséquents inédit pour des politiques de santé du grande tâche du handicap et de la famille. Mais le rôle du PLFSS c'est aussi d'améliorer la vie de nos concitoyens et de préparer l'avenir. Je pense en 1er lieu à la transition démographique et qui est en cours dans notre pays en 2030 un tiers de la population aura plus de 60 ans. Or le virage à domicile hier que la majorité des Français appellent de leurs voeux, hé bien en cours et c'est pour cela que nous faisons le choix tout d'abord de renforcer les services de soins infirmiers à domicile avec le financement de 4000 nouvelles places en cohérence avec notre trajectoire d'augmentation de 20 pour 100 d'ici à 2030. C'est pour cela aussi que nous ajoutons 2 heures de présence supplémentaire chaque semaine pour les 780000 personnes bénéficiaires de la pas à domicile. C'est comme cela que nous apportons de la sérénité à des gestes de soin et que nous aidons les professionnels à retrouver le sens de leur métier. C'est pour cela, encore que nous renforçons la lisibilité de l'offre qui est crucial pour que les bénéficiaires exerce un libre choix et un choix éclairé. D'abord avec la poursuite de la logique de guichet unique, engagé en 2022 que nous consolidons avec le forfait coordination. Ensuite, avec l'introduction de davantage de souplesse pour les bénéficiaires de la pas. Je salue à ce titre, le travail accompli entre le gouvernement et le Parlement qui a permis d'aboutir à une solution appropriée en s'inspirant de ce qui existe pour la prestation de compensation du handicap, la même possibilité de report des heures non utilisés sur six mois sera ainsi demain, appliquée au plan à part. Un autre résultat de dialogue de qualité entre le gouvernement et les assemblées, c'est l'amélioration de l'accompagnement financier des départements par la Caisse nationale de solidarité, de l'autonomie. Les mesures de revalorisation des rémunérations des salariés des aides des services d'aide à domicile, ont eu un impact marqué sur les finances des départements, le gouvernement en a ainsi pris acte. Je pense aussi évidemment aux mesures relatives au handicap. L'augmentation de 5,2 pour 100 de l'objectif national de dépenses pour le veau, les personnes en situation de handicap est inédite. Elle nous permet d'accélérer la mise en oeuvre de grands objectifs et de politique prioritaire, il s'agit entre autres de développer davantage les relations entre l'école et les établissements médico-sociaux, par exemple en renforçant la création de services d'accompagnement à la scolarisation en milieu ordinaire ou de poursuivre le déploiement des unités de scolarisation dédié aux élèves poly-handicapé. De diversifier les modalités d'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes pour favoriser l'accompagnement dans leur lieu de vie habituel. Je pense aussi à la poursuite des mesures concernant l'autisme et les troubles du neuro-développement avec 80 millions d'euros prévus ces financements permettront ainsi d'étendre aux 7 12 ans la politique de détection précoce. Qui est l'une des réussites majeures de la stratégie nationale et qui a permis à près de 30000 enfants depuis 3 ans, d'être détecté à temps et donc correctement accompagnés. Là encore le texte porté une ambition forte dès l'origine, amplifié au cours de la navette parlementaire et je pense tout particulièrement à la à la création de briques informatique nationale afin d'harmoniser les systèmes d'information, des maisons départementales des personnes handicapées et de faciliter leur interopérabilité ceux-ci simplement pour garantir une meilleure équité de traitement sur le territoire. de l'universalité des droits. J'exprime ici le voeu que nous conservions à l'avenir un tel esprit de coconstruction, dans la perspective de la prochaine conférence nationale du handicap. Dans ce PLFSS des mesures relatives aux familles, elle concerne en particulier la réforme du complément de mode de garde qui doit permettre à chacun et chacune de pouvoir occuper un emploi mais aussi lutter contre les inégalités à la racine, dès la petite enfance. Nous modifions ainsi le barème du complément de mode de garde pour permettre aux familles qui ne recourent pas à la crèche, de pouvoir faire garder leur enfant au même coûte par une assistante maternelle. De même, nous étendons le CMG au-delà de 6 ans et jusqu'à l'entrée au collège pour les familles monoparentales. L'engagement du gouvernement aux côtés des familles monoparentales, dont 30 % vivent dans la pauvreté et 90 % sont des femmes et Total il passe aussi depuis le 1er novembre par l'augmentation de 50 % de la pension alimentaire minimale. Cette mesure doit faire baisser le taux de pauvreté des familles monoparentales de de le de points. à cela s'ajoutent les créations de nouvelles places d'accueil pour combler les 200000 places manquantes d'ici 2030, nous savons que 160000 par ne reprennent pas leur travail, faute de solution, c'est donc un enjeu d'égalité des chances de développement pour les enfants d'accès à l'emploi et de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, pour leurs parents. Ces mesures forment la première Pierre du service public de la petite enfance, engagement de campagne du président de la République qui s'inscrit dans la droite ligne de ce qui a été fait avec les mille premiers jours nous y travaillerons avec responsabilité et ambition tout au long de ce quinquennat avec les collectivités locales. Permettez-moi maintenant d'en venir au volet santé. En la matière, la première vocation de ce texte, c'est d'améliorer l'accès à la santé pour tous. Nous capitalisons donc sur les mesures d'urgence prises cet été, le président de la République l'avait annoncé et c'est une mesure forte face aux territoires sous-dotés, nous exonérant de cotisations retraite les médecins retraités qui souhaiteraient continuer à s'engager dans notre système de santé. Nous actionnant également plusieurs leviers pour reconquérir du temps soignant dans tous les territoires, je pense tout d'abord à la création d'une 4ème année de consolidation au diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Un véritable projet pédagogique permettra durant 7 années supplémentaires d'internat d'accompagner les futurs médecins à leur installation rapide. Une mission lancée conjointement par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de la Santé, de la prévention permettra par ailleurs de concerter avec l'ensemble des parties prenantes sur les conditions de succès de cette réforme. Nous souhaitons également à l'heure où s'ouvrent les négociations conventionnelles et créer un cadre plus adapté. Cela permettra d'accompagner pleinement les engagements réciproques qui feront l'objet des discussions dans le cadre du CNR, santé. L'objectif est d'améliorer la réponse aux besoins de santé dans les territoires et de créer les conditions d'un renforcement du temps soignant dans les zones sous-denses. Enfin nous simplifions et nous renforçons la politique d'aide à l'installation. Le gouvernement entend harmoniser les dispositifs d'aide en renvoyant l'ensemble de ceux qui sont portés par l'État aux champs conventionnels, sauf pour les étudiants et les remplaçants. En parallèle, les territoires seront invités à généraliser des guichets uniques pour apporter plus facilement des réponses concrètes à toutes les questions que se posent les jeunes médecins avant de s'installer en libéral. Enfin, il faut souligner que ce PLFSS permet de se projeter au-delà de l'année à venir. Il a ainsi pour ambition de remettre durablement l'éthique au coeur du système de santé. Il en va ainsi du recours à l'intérim. Malgré une volonté de la part des pouvoirs publics de mieux le réguler. Il a pris trop d'importance, avec un coût financier inacceptable à l'heure où nous devons rééquilibrer les comptes de la Sécurité sociale. Surtout, il engendre une déstabilisation des services et des équipes, notamment dans les territoires démographiquement fragiles en professionnel de santé. Ce PLFSS renforce donc la régulation de l'intérim. Et je veux rappeler l'amendement du groupe RDPI, qui permet d'appliquer les mesures du PLFSS aux entreprises intérimaires situé à l'étranger. Cette évolution ira de Pair avec les travaux à engager sur l'accompagnement des débuts de carrière au service des jeunes professionnels. Enfin, ce Plfss transforme le système de santé en accélérant le virage préventif. Et cela passe par plusieurs mesures importantes. Les rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie constitue une innovation majeure. Vaccination dépistage des cancers, santé sexuelle habitudes de vie dépistage auditif et visuel santé mentale les termes abordées au cours de ces rendez-vous seront très large adapté en fonction des âges selon une approche globale de la santé de la personne. Ces rendez-vous de prévention seront intégralement pris en charge par l'assurance maladie, sans avance de frais, de façon à réduire les inégalités. Par ailleurs, le Covid 19 là, montrer la prévention, c'est en grande partie la vaccination. Ce Plfss prévoit donc sur la base des recommandations de la Haute autorité de santé d'étendre aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes la prescription et la réalisation des vaccins. Cette mesure permettra très concrètement de simplifier le parcours des passions en augmentant le nombre de professionnels habilités à vacciner. Ce PLFSS renforce également la prévention. En améliorant la santé sexuelle, le gouvernement souhaite faciliter les dépistages des infections sexuellement transmissibles, au-delà du seul VIH qui pourra désormais se faire sans ordonnance et sera intégralement remboursé pour viser tout particulièrement les jeunes de moins de 26 ans. Enfin, donner le choix aux femmes de disposer de leur corps. C'est bien sûr assurer le recours à l'IVG, mais c'est aussi s'assurer que la contraception d'urgence soit accessible à toutes. Nous proposons donc d'élargir à toutes les femmes majeures, la délivrance gratuite de la contraception d'urgence hormonale en pharmacie, le tout sans conditions de prescription médicale. En un mot ce PLFSS concrétise notre ambition de faire de la prévention un pilier à part entière de notre système de santé. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, voilà les premières briques que pose ce PLFSS c'est un texte de responsabilité, c'est un texte qui répond aux urgences aujourd'hui tout en préparant les défis de demain, c'est un texte qui conserve certains de vos apports qui signe que ce débat a été fécond en première lecture dans votre chambre, je vous remercie. Merci madame la ministre, je vais donner la parole à Madame Élisabeth. Tu dois rapporteur général de la commission des affaires sociales pour dix minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, chers collègues, oui, Madame la Ministre, vous avez raison, c'est un texte important, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, c'est important pour 2 raisons : la première c'est que ces 600 milliards d'euros et que c'est 5 fois le budget de la défense je n'arrêterai pas de le répéter pour dire combien c'est important la 2ème raison, c'est que ça concerne l'ensemble de la protection sociale des Françaises et des Français et que cette en fait un rendez-vous, un rendez-vous important, le Carrefour de la protection sociale pour notre pays, après l'échec de la commission mixte paritaire, sur ce projet de loi, l'Assemblée nationale a examiné ce texte en nouvelle lecture, les députés ont pu débattre en séance, de l'article liminaire, qu'ils ont amendé pour coordination de la première partie relative aux comptes de 2021, qu'ils ont curieusement adopté conforme, pourquoi curieusement car cela signifie qu'ils ont adopté l'article 1er dans sa version Sénat en suivant, donc les préconisations de la Cour des comptes, pour autant, même après ce vote, l'article 2 qui approuve le tableau patrimonial n'a pas été amendée de ce fait, l'un des articles affiche donc un déficit de 29,5 milliards d'euros pour l'année dernière et l'autre un déficit de seulement 24 3 milliards d'euros, une telle discordance est pour le moins curieuse et pourrait amener le Conseil constitutionnel à s'interroger sur la sincérité de ces dispositions s'il en était saisi, enfin, les députés ont examiné la deuxième partie sur les comptes de l'année en cours essentiellement pour adopter une nouvelle rallonge de l'Ondam 2022, à hauteur de 500 millions d'euros afin de compléter les financements octroyés au système hospitalier afin de compenser les surcoûts liés à l'épidémie de Covid 19 pour les établissements de santé en 2022

madame la Ministre, comme nous l'avons constaté en commission, cette nouvelle révision est de nature à conforter la grande prudence du Sénat quant aux estimations du gouvernement, pour ce qui concerne l'enveloppe de 2023 qui n'est que de 1 milliard d'euros. Une fois passé l'examen de ces 5 articles, la suite a été beaucoup plus expéditive, puisque le gouvernement a engagé sa responsabilité à 2 reprises, l'une au tout début de la 3ème partie, l'autre au tout début de la 4ème partie il n'y a donc eu aucun débat en séance sur ces 2 partis en nouvelle lecture. Et ni la partie recettes ni la branche maladie n'auront fait l'objet d'un quelconque débat en séance publique à l'Assemblée nationale lors de ce Plfss en première lecture, comme en nouvelle lecture. De ce fait, Madame la Ministre, c'est bien ce que le gouvernement a souhaité retenir retenir qui nous arrive aujourd'hui. Or, reconnaissons que les apports du Sénat qui figurent dans ce texte sont particulièrement modeste, on retiendra pour l'essentiel dans la partie recettes un amendement à l'article 11 bis qui aligne le régime social des rachats de RTT et des heures supplémentaires pour les entreprises de 20 à 249 salariés sur le volet, autonomie, on s'illuminera la reprise d'un amendement de Bernard Bonne qui traduisait l'une des recommandations du rapport sur le contrôle des Epad, à savoir le plafonnement du montant des excédents pouvant être mis en réserve. Enfin sur le volet maladie je signalerai le maintien de la prolongation de la garantie de financement des établissements de santé, on peut évoquer aussi un amendement encadrant le développement de la biologie médicale délocaliser qui intervient lorsque le prélèvement ou la phase analytique d'un examen de biologie et réalisé en dehors d'un laboratoire de biologie médicale je précise enfin que, comme notre rapporteur de branche Corinne Imbert et notre présidente Catherine Deroche l'avait fortement souhaité le report de l'entrée en vigueur de la réforme du financement de la réforme de financement des activités de soins de suite et de réadaptation sera donc au 1er juillet 2023. oui c'est à peu près tout, il me semble que c'est bien modeste pour ce qui concerne les mesures véritablement normative, je précise que les auteurs d'amendements trouveront dans le rapport écrit un tableau qui retrace le sort de chacun d'entre eux. évidemment. Aucun des amendements les plus significatifs, adopté par le Sénat n'a été retenue, c'est le cas de l'article additionnel. Défendu par René-Paul Savary qui introduisait pour améliorer l'emploi des seniors et engager le redressement de notre système de retraite, c'est le cas des différentes mesures que nous avons proposé afin de restaurer un contrôle parlementaire en cas de dépassement de l'Ondam et de son enveloppe Covid 19 que nous considérons sous-estimé, c'est le cas de l'amendement qui se contentait d'accorder au ministre un pouvoir supplémentaire, celui de refuser une convention médicale dont les conséquences financières seraient incompatibles avec l'Ondam, voté par le Parlement, c'est le cas de la contribution des organismes complémentaires d'assurance maladie que nous souhaitions matérialisée au sein de ce Plfss, je le rappelle, à hauteur de 300 millions d'euros, et c'est le cas de notre refus du transfert de 2 milliards d'euros de charge de la branche vieillesse à la branche maladie. Quant à l'Ondam 2023 malgré les hausses incessantes de celui de 2022, le gouvernement n'a toujours pas estimé nécessaire de le revaloriser à l'occasion de la nouvelle lecture cette donc de nouveau le montant que le Sénat a rejeté en première lecture, qui revient de l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ces marqueurs même des apports plus modestes et potentiellement plus consensuel, n'ont pas été par exemple sur l'un des l'intérim médical ou sur l'encadrement des téléconsultations au bout du compte, même si nous avions des points d'accord dans le texte d'origine, on peut considérer que c'est particulièrement maigre et pas toujours respectueux des débats riches et sérieux que nous avons pendant toute une semaine. Dès lors, comme cela est hélas devenu la tradition même si les circonstances sont bien différentes, il est temps de constater que Poursuivre la navette ne servirait plus à grand chose, d'autant que le gouvernement va très probablement utilisé de nouveau la procédure de l'article 49 alinéa 3 en lecture définitive et qu'il a déjà clairement indiqué ce qu'il souhaitait retenir de nos propositions. De ce fait, la commission des affaires sociales proposera au Sénat d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable sur ce Plfss pour 2023 afin de marquer nos désaccords sur le fond et sur la méthode, je vous remercie de votre attention. Merci madame la rapporteure générale. Alors, dans la suite de la discussion générale, la parole. Monsieur Bernard Jomier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour six minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission madame la rapporteure, mes chers collègues. ce budget de la Sécurité sociale est intéressant évidemment parce que c'est le 1er du quinquennat et qui il prend place donc dans cette nouvelle situation politique voulue par les Français au mois de juin qui est que, du fait de l'absence d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, les mouvements politiques et nous les parlementaires sommes invités à faire preuve de compromis politique. Depuis le début de cette législature, nous avons vu ainsi le gouvernement sur des projets de loi passer des compromis avec les républicains, puisque c'est le mouvement qui, à l'Assemblée nationale peut garantir l'adoption définitive d'un texte et que par ailleurs le tropisme vers la droite de la mouvance présidentielle et, de plus en plus nette au fil du temps pour ceux à qui cela aurait échappé. Et nous arrivons au 1er texte budgétaire soumis au 49 3 et donc la question qui se poser. Et la vérité que nous allions voir apparaître, c'est est-ce que le gouvernement s'est converti à ceux de cette demande de compromis des politiques des Français, par conviction ou au moins par réalisme ou est-ce qu'au fond subsiste la tentation de la brutalité à à Lyon nous avoir un 49 3 brutale et autoritaire, ou un 49 3 de compromis politique. Hé bien, je crois que nous avons la réponse. La réponse, c'est que le travail des oppositions, a été balayée aucun amendement de notre groupe. Et exactement utile porté sur des thèmes d'intérêt pour les Français utile était adopté par l'ensemble du Sénat Assemblée qui, elle, malgré des oppositions de fond entre les groupes politiques à une pratique du compromis politique et parce qu'il y a cette partie pratique du compromis politique, nous avons su nous présenter des amendements adoptés par nos collègues de la majorité sénatoriale, hé bien le gouvernement a balayé tout cela. Et il revient la bouche en coeur pour nous proposer une deuxième lecture, mais de qui vous moquez-vous. Je vais vous dire de la volonté des Français exprimée dans les urnes au mois de juin car vous tournez le dos à cette volonté de compromis politique vous nous assigner vous nous assigner à notre identité propre en refusant tout travail en commun et j'y viendrai sur des articles de fond et qui va profiter de cette posture du gouvernement ce qui jeudi soir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale se sont livrés à cette séance au sens terrible debout applaudissant les propos les plus outranciers, pendant que le bloc central des oppositions de gauche et modérée était silencieuse, c'est aux extrêmes que vous donnez raison par cette posture politique ce 49 3 dans ces conditions là, sur le budget de la Sécurité sociale, vous rendez un mauvais service à notre démocratie politique et quant au fond. Et quant au fond, l'année dernière à cette même tribune je formé le souhait que les élections présidentielles soient l'objet d'un débat sur la santé et de nouvelles orientations en la matière est-ce que ce budget de la Sécurité sociale tire la leçon de la pandémie que nous vivons encore aujourd'hui aucunement. Aucunement aucune disposition. Et ce qui le porte, ce que nous soutenons totalement le virage de la prévention, annoncé par le ministre de la Santé aucunement sur le tabac quand le Sénat rétablit le texte initial du gouvernement, le congrès des buralistes demandent au ministre des comptes publics de changer le texte et le gouvernement revient sur sa proposition, quand il s'agit de protéger notre jeunesse par la taxation des bières sucré et aromatisé ou par les peuvent, comme ça a été proposé par notre collègue Catherine Procap Catia est-ce que le gouvernement ouvrent la porte, rien du tout, il balaye tous ces amendements le virage de la prévention n'existe pas aujourd'hui à l'heure où nous débattons des professionnels de santé protestent aujourd'hui, ce sont les psychiatres, demain ce seront les infirmières après-demain, ce seront les médecins généralistes hier et demain, c'est l'hôpital public, le monde de la santé est en rébellion Le monde de la santé cri qui n'a pas les moyens de remplir sa mission et on réduit l'Ondam de l'hôpital public en dessous de l'inflation et on réduit l'Ondam, des professionnels de ville à la moitié de l'inflation. Mais écoutez, nous ne sommes pas là pour faire du cinéma ou pour perdre notre temps la rapporteure a raison à quoi sert une 2ème délibération dans ces conditions, vous avez balayé tout notre travail, vous ne souhaitez pas de compromis vous usez légalement du 49 3 un objet constitutionnel qui vous est confiée, mais l'usage que vous, en fait il est mauvais, il est brutal et nous le rejetons. rejetons. La parole est à madame Laurence Cohen pour le groupe communiste République. Qui un citoyen et écologiste pour quatre minutes chers collègues. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, en ouverture des débats en seconde lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023, le ministre de la Santé a annoncé une rallonge de 543 millions d'euros pour l'hôpital au titre de l'année 2022 cette enveloppe doit permettre d'absorber, selon ses propos, les surcoûts liés à l'épidémie de Covid 19 et de soutenir l'hôpital et tous les personnels qui le font fonctionner ces 543 millions viennent s'ajouter aux 570 millions débloqués pour faire face à l'épidémie précoce de bronchiolite qui imposent actuellement une très forte tension sur les urgences pédiatriques ces crédits supplémentaires sont une bonne nouvelle pour les services hospitaliers mais pourquoi attendent d'être acculé pour le faire, pourquoi ne pas entendre et reprendre nos propositions, celles de notre groupe en les inscrivant dans la loi de financement de sécurité sociale initial à chacune de nos propositions allant en ce sens, vous avez répondu par de l'autosatisfaction mais preuve que votre budget n'était pas si extraordinaire que ça puisque vous votez des rallonges et même si nous saluons ces moyens supplémentaires, ils ne pourront couvrir uniquement que le doublement de la rémunération des heures de nuit pour l'ensemble des personnels et le paiement des heures supplémentaires, jusqu'au 31 mars seulement, ce qui signifie que ce PLFSS 2023 est marqué par une insincérité financière que le gouvernement souhaite sans doute rectifié en fin d'année lors de l'examen du Plfss pour 2000 vingt-quatre celui qui va continuer à plonger l'hôpital dans une situation explosive, d'autant plus avec un Ondam Ciba en dessous de l'inflation en réalité si ce Plfss 2023 et remarquables, c'est par toutes les mesures urgentes qui ne contient pas, je n'ai pas la possibilité de toutes les évoquer ici, mais j'en citerai quelques-unes rien pour combattre véritablement les déserts médicaux, les inégalités sociales et territoriales de santé aucune disposition pour combattre la marchandisation des médicaments, pas de prise en compte de l'ampleur de la crise de la de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie et là je pourrais multiplier les exemples qui démontre votre incapacité à anticiper et surtout votre absence de volonté à renforcer à redresser notre service public de santé, en ce 29 novembre journée nationale de mobilisation et de grève dans le secteur de la santé mentale, je voudrais apporter mon soutien et le soutien de l'ensemble de mon groupe au personnel, victime d'une crise sans précédent, et ce dans un souci silence assourdissant des tutelles, 4 organisations syndicales réclament un Ségur spécifique face à l'abandon de la psychiatrie, qui subit des suppressions de lits, des fermetures de centres médico-psychologiques une pénurie très forte de personnels, le personnel soignant se dit dans l'impossibilité d'exercer correctement leur son métier il y a donc urgence à revaloriser à investir le secteur de la psychiatrie publique enfin je voudrais interpeller une nouvelle fois le gouvernement sur la nécessité de réindustrialisation de réindustrialisation de notre pays et la mise en place d'un dispositif permettant de reprendre la main sur la production et la distribution de médicaments, ce dispositif que nous appelons de nos voeux, a pour nom le pôle public du médicament, il se décline au plan national et européen, il est urgent de mettre en place, vous savez, mes chers collègues, qu'il y a une pénurie dramatique des antibiotiques, et singulièrement de l'Amoxicilline qui est un traitement courant pour les enfants, quand allez-vous agir contre la toute puissance de grands labos pharmaceutiques qui décide de tout, des prix des molécules de la durée de vie de tels ou tel, traitement malheureusement pas pas dans ce budget de la Sécurité sociale, alors si on ajoute à tous ces manques à tous ces refus de sortir notre système de santé de la tempête, dans lequel il se trouve, le mépris des parlementaires que nous sommes, avec l'utilisation à quatre reprises de l'article 49 alinéa 3 de la pour passer outre les débats là de l'Assemblée nationale, et de ne même pas garder en CMP, les propositions qui avait recueilli l'unanimité au Sénat, il est impossible de voter en faveur de ce Plfss pour 2023 je vous remercie. si la parole est à monsieur Olivier Henno pour le groupe Union centriste pour six minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame, le rapporteur général, mes chers collègues je vais entamer mon propos par une citation d'un humoriste que j'adorais que j'adore toujours Raymond Devos une mauvaise rengaine c'est un air qui commence par vous rentrez par une oreille et qui finit par vous sortir par les yeux. Eh bien, il en est ainsi du 49 3 et plus encore de ce 49 3 qui retient très peu de nos débats, j'allais dire, rien ou presque rien parce que il y a 49 3 et 49 3, celui-ci est un 49 3 dans une version rude dans une version hard, comme diraient les jeunes le PLFSS du conseil des ministres, et pour le reste, circulez, il n'y a rien à voir les 49 3 répétition sur les débats budgétaires, c'est un peu comme le poil à gratter au début cela chatouille puis cela irrite et avec le temps cela devient insupportable, l'abus du 49 3 n'est pas illégal, bien sûr, mais là à défaut congénital, par nature, il assèche l'envie, j'allais dire le désir de trouver des accords il assèche l'envie et le désir de négocier l'envie et le désir du débat de la discussion parlementaire et de la co-construction. Moi qui ne craint pas de revendiquer une filiation avec feu le MRP se retrouve cela tout à fait regrettable, alors j'entends ceux qui disent cela toujours été comme ça, c'est la 5ème République peut être, mais d'abord, j'en suis pas totalement sûr et puis pardonnez-moi je trouve cet argument assez faible, voyez-vous, cher collègue, j'ai eu l'honneur d'être collègues de Maurice Schumann au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, de 92 à 98 c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais il manie à la perfection la dialectique entre légalité et légitimité, je ne développerai pas à l'excès, cette question, mais l'abus du 49 3 pose la question de la légalité de la légitimité, je sais que cette dialectique doit être manié avec précaution, avec nuance mais c'est un sujet d'ordre constitutionnel, il pose aussi la question des marges de manoeuvre des ministres lors de la discussion parlementaire vis-à-vis de Bercy, c'est encore un autre sujet, voilà pour la forme mais comme disait Victor Hugo, qui siégea ici même la forme, c'est le fond qui remonte à la surface et sur le fond, notre rapporteur général, Élisabeth Doineau, a dit l'essentiel, je veux simplement au nom du groupe UC insister sur quelques sujets qui nous tiennent à coeur, reconnaissant que tout n'est pas à jeter dans ce PLFSS la majorité sénatoriale a d'ailleurs défendu des axes structurants, elle peut en être fier, je pense notamment aux amendements portés par notre groupe est soutenu par la majorité, l'élargissement et l'exonération de cotisations patronales spécifique à l'emploi ça saisonnier dit TODE l'exonération d'impôt sur le revenu et de CSG sur les chèque carburant versées par les employeurs, ou encore l'annulation du transfert aux Urssaf des cotisations Agirc-Arrco le paritarisme, c'est notre ADN, et nous en serons toujours les avocats, Madame la Ministre, permettez-moi aussi de regretter l'abandon d'amendements concret sur la démographie médicale, l'intérim, les biologistes ou encore les téléconsultations vous donner la priorité aux vieillir à domicile, très bien, nous la partageons et donc fort de ce constat, le Sénat sur l'initiative du groupe UC avait adopté un amendement tendant à accélérer le déploiement de 2 heures de temps social prévu dans le texte, tant pour les personnels des que pour les bénéficiaires de la

il s'agit d'un enjeu majeur de soutenabilité de la dépense et de la juste compensation due aux collectivités territoriales, avec Valérie Létard : nous avions appelé de nos voeux, une réforme des concours de la CNSA pour les départements là au corps votre message politique est limpide : pas de soutien envers nos territoires et départements ou collectivités locales et territoriales qui en ont pourtant fort besoin par ailleurs, vous avez aussi écarté la consultation de l'ADF, dans le cadre de l'alignement de la forfaitisation de la pas sur les modalités de forfaitisation de la PCH au profit de la saisine du Conseil national d'évaluation des normes, le refus de territorialisées et regrettable sur cette question, comme tant d'autres, le groupe UC vous le dis n'est pas qu'acceptable que l'État décide et que les collectivités locales, doit se contenter de payer, j'en viens à la politique familiale de ce Plfss le modèle de la famille française évolue, il a besoin du soutien de de l'État et à une véritable politique ambitieuse qui accompagne et donne un cap

je le répète, pour nous, la politique familiale n'est pas une politique sociale, c'est une politique familiale et de ce point de vue, vous ne nous empêcherez pas de penser que le transfert des Ziggy de 2 milliards d'euros de la branche famille vers la branche santé est un bien triste symbole avant de conclure, dans ce tableau un peu sombre, je veux évoquer de lueur l'amendement d'Annick Jacquemet sur le contrôle des établissements et celui de Nathalie Goulet sur l'obligation de verser sur un compte domicilié en France ou dans la zone, c'est pas les prestations soumises à condition de résidence, vous l'avez compris le groupe UC votera cette question préalable, même si, même si nous n'aimons pas ce procédé, par nature, d'abord parce que nous sommes perplexes, vous l'avez compris sur nos débats passé et leur utilité et puis parce que nous n'avons aucune illusion sur le l'utilité d'un nouveau débat sur ce PLFSS et parce qu'en matière parlementaire comme dans la vie réelle, nous n'avons aucun goût particulier pour le vélo d'appartement, je vous remercie. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, cette nouvelle lecture vient clore les débats du PLFSS qui aura été marquée cette année par des conditions d'examen particulièrement difficile de 49 3 à l'Assemblée en première lecture une semaine de discussions au Sénat, suivie de de nouveau 49 3 l'assemblée en nouvelle lecture, si les débats au Sénat, se sont déroulées avec le sérieux et le respect qui caractérise notre assemblée, nous avons souffert de délai extrêmement contraint le texte de l'Assemblée nationale ayant été publié seulement hier soir, nous étions ce matin même en commission pour examiner le rapport à peine quelques heures avant le début de la séance, le budget de la Sécurité sociale et pourtant cela a été dit le plus gros budget de l'État et il mérite que l'on s'y attarde, c'est pourquoi, comme chaque année, le groupe RDSE regrette mais comprend le dépôt d'une motion tendant à opposer la question préalable nous comprenons ce choix effectivement faisons nous aussi le compte de peu de mesures du Sénat retenu par le gouvernement mais par principe le RDSE préférera Poursuivre la discussion, considérant que dans un contexte d'inflation des ordonnances toute opportunité pourrait être saisie pour autant reconnaissons également que le gouvernement n'a pas créé les conditions favorables d'une nouvelle lecture certains apports votés par le Sénat aurait effectivement pu être conservés par le gouvernement, notamment la pérennisation du dispositif TODE défendue de longue date par le RDSE et d'autres groupes ou encore l'annulation du transfert aux Urssaf du recouvrement de plusieurs types de cotisations ou encore des mesures de prévention en direction de la jeunesse Bernard Jomier la rappeler toutefois, nous partageons des points de ce Plfss, dans la situation de pénurie de praticiens que l'on connaît, dans l'attente des premiers résultats, espérons-le, positif du numerus apertus à Perthus il est nécessaire de trouver des solutions de court terme, c'est une nécessité absolue pour alléger la charge de travail des médecins qui reste est enclenché le virage de la prévention, nous saluons donc les rendez-vous de prévention des âges de la vie, tout comme l'accès facilité au dépistage des infections sexuellement transmissibles, le cumul emploi-retraite plus avantageux permettra par ailleurs aux médecins qui le souhaitent de prolonger leur activité, enfin et surtout, le partage des tâches permettront de libérer du temps médical tout en améliorant l'accès aux soins via les certificats de décès délivrés par les infirmiers l'élargissement du nombre de professionnels habilités à administrer les vaccins, ainsi que l'accès Direct aux infirmiers en pratique Avast avancer sous réserve, et j'insiste, de confier l'application de cette mesure aux équipes coordonner sur le terrain, je veux parler des MSP des ESP ou des ces BTS par ailleurs, nous constatons que l'ajout d'une 4ème année de troisième au au 3ème cycle des études de médecine générale, les débats ont porté leurs fruits, lors de l'examen de cet article en séance, j'ai défendu avec insistance l'importance de garantir aux étudiants l'encadrement par des maîtres de stage des universités et la possibilité de réaliser une partie du stage en milieu hospitalier, si je souhaitais qu'il soit réserve aux hôpitaux de proximité, je me satisfait de ces précisions indispensables qui rappelle avec force que cette année supplémentaire et une année de formation mais juste une année de formation pour autant le PLFSS n'a pas vocation à changer en profondeur le système de santé qui en a tant besoin les médecins libéraux seront en grève jeudi et vendredi, rejoignant la longue liste des professionnels de santé à bout de force dont les urgentistes, pédiatres, sages-femmes, pharmaciens ou encore les laboratoires d'analyses, je salue ici leur travail et leur engagement il y aurait tant à dire Madame la Ministre, sur le manque d'anticipation des politiques de santé sur les aspirations des jeunes générations qui ont bien changé sur le manque de projections à moyen terme qui pourrait être l'objet d'une loi pluriannuelle très attendu sur l'indispensable révolution de la prévention ou encore sur la place trop importante de la tarification à l'acte, en somme une transformation en profondeur, a mené avec les premiers concernés, accompagné d'un grand soir de la décentralisation est seule en mesure de relever le défi, une gouvernance territoriale composée de tous les acteurs du soin des collectivités, des associations de patients à l'échelle d'un territoire pour répondre aux besoins et non à l'offre, comme le lait se plaît à le dire, le ministre-Bruno pour toutes ces raisons, le groupe RDSE votera contre à la question préalable et appelle de ses voeux une grande loi de sa mère. Si cher collègue, la parole est à Madame Corinne Imbert pour le groupe Les Républicains pour dix minutes.

Madame le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure générale, Madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Alors que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 arrive à la fin du du processus législatif, il est maintenant temps d'en tirer des enseignements nécessaires tout d'abord je tiens à remercier à nouveau la rapporteure générale, les rapporteurs et l'ensemble de mes collègues sénateurs qui ont travaillé sur ce texte, qui ont beaucoup travaillé sur ce texte, en effet, une fois de plus, le Sénat a montré sa capacité à enrichir et à améliorer le texte, qui lui était proposé, loin du tumulte de l'actualité, l'ensemble des groupes politiques qui composent cette assemblée ont su apporter lors de cette semaine d'examen en séance publique des propositions cohérentes, constructives et argumentées. Au-delà des désaccords politiques qui nous sépare sur le fond et en cette période trouble où la parole du politique est souvent mise à mal, je pense qu'il est nécessaire de rappeler la qualité de débat que l'on trouve au sein de cet hémicycle, il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, que c'est uniquement dans l'hémicycle du Sénat que le débat sur la branche maladie, et donc sur la santé, a eu lieu en première lecture au Sénat, nous sommes employées à enrichir ce texte de manière pragmatique, j'en veux pour preuve les différentes mesures votées dans cet hémicycle, nous avons pris nos responsabilités. Ma mon plus grand regret, une nouvelle fois le Sénat n'a pas été entendu par le gouvernement et par la majorité présidentielle et j'y reviendrai, alors que l'Ondam 2022 avait été supprimé à l'Assemblée nationale en première lecture le Sénat a été indulgent en réintégrant l'Ondam 2022 dans le texte, le débat s'est cependant crispé rapidement quand, dès le début de l'examen du texte, vous avez déposé, madame la ministre, un amendement relevant l'Ondam 2022 de 600 millions d'euros régularisant ainsi une dépense réalisée entre le 1er juin et le 15 septembre dernier mais que vous avez été incapables d'afficher dans le projet de loi initial fin septembre 2022, que dire de cette nouvelle augmentation de 500 millions d'euros inscrite dans le texte à l'issue d'un nouveau 49 3 à l'Assemblée nationale, au total, c'est une augmentation, comme l'a rappelé la rapporteure générale de 10,1 milliards d'euros pour l'Ondam 2022 par rapport à l'Ondam voté dans la dernier loi de financement de la Sécurité sociale, nous comprenons mieux que vous ne souhaitiez pas que le comité d'alerte joue son rôle. Nous avons rejeté la trajectoire financière proposée par le gouvernement jusqu'en 2026 loin d'être démagogique cette suppression fait suite à l'absence de plan stratégique au manque de sincérité de cette trajectoire financière, nous avons du mal à croire à un redressement de la trajectoire aussi spectaculaire car il ne repose que sur un effet recettes anticipées mais revenons au travail du Sénat en première lecture, pour 2023 travail marquée par de la constance et de la cohérence de la part de notre groupe, comme souvent ces dernières années, nous avons voté la mise en place d'une contribution la d'arrêter les organismes complémentaires d'assurance maladie, au bénéfice de la branche maladie à hauteur de 300 millions d'euros, loin de vouloir acculer les aucun, nous souhaitons que l'ensemble des acteurs de santé participent de manière proportionnelle aux défis posés par la pandémie récente mais vous le refuser. Nous avons supprimé le transfert de charge de 2 milliards d'euros entre les branches famille et maladie ce transfert que vous maintenez constitue un moyen artificiel de diminuer les moyens dévolus à la politique familiale et traduit un manque d'ambition chronique en faveur d'une politique familiale, vous vous en été dans cette voie. Fidèle à notre tradition de défense de l'agriculture française, nous avons pérennisé le système spécifique d'exonération de cotisations et de contributions sociales patronales pour l'embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d'emplois du secteur agricole, vous faites le choix de le prolonger le dispositif quelques années je vous en accordera nous avons par ailleurs modifier la mesure d'ajout d'une 4ème année d'internat en substituant à la rédaction du gouvernement par celle de la proposition de loi du président, Bruno Retailleau, proposition de loi adoptée au Sénat en octobre dernier, cette rédaction nous apparaît plus solide que pour le plan sur le plan logistique et plutôt que de valoriser une initiative parlementaire, le gouvernement s'est entêté à introduire cette mesure dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, je préciserai sur ce point que la version du texte issu du 49 3 à l'Assemblée nationale et qui nous est soumis aujourd'hui permet à titre exceptionnel. Pardon que le stage de quatrième année puisse être réalisée par dérogation en milieu hospitalier ou extra-hospitalier en rajoutant cette possibilité, vous avez dénaturé l'objectif initial de la mesure et nous ne pouvons que le regretter, au-delà du fond, la forme nous interpelle également cette mesure telle que rédigée ne relève techniquement pas d'un texte financier mais d'un texte santé qui modifie les études médicales et l'organisation des soins ces dernières années, de nombreuses mesures qui ne relevait pas du Champ d'une loi de financement de la Sécurité sociale ont été introduites par les gouvernements, alors même que le Sénat lui-même, quant à lui est plus exigeant en matière d'irrecevabilité, nous attendons une loi santé mais il est vrai que nous attendions aussi grand âge et autonomie et peut-être que nous allons entendre attendre encore un moment afin de faire face aux tensions sur l'offre de soins, nous avons voté une mesure visant à mieux encadrer l'intérim médical et paramédical en début de carrière, mais vous le refusez également sur l'épineux dossier qui oppose le gouvernement et les biologistes votre méthode avouez lieu n'a pas été très élégante vis à vis de avec le rapporteur général, nous avons proposé la mise en place d'une contribution exceptionnelle de 150 millions d'euros sur la seule année 2023 cette solution constitue un compromis raisonnable qui aurait été accepté par les biologistes vous le refusez vous en état poursuivent dans votre voix, sous prétexte d'une rentabilité record pour le secteur de la biologie médicale. Nous ne contestons pas cet état de fait, mais n'oublions pas que ces mêmes biologistes ont été en capacité d'investir énormément pendant la pandémie afin de faire face à l'explosion de la demande, n'oubliez pas, sur ce sujet, que c'est l'État qui a été le prescripteur et que c'est aussi lui qui a fixé les différents tarifs, nous avons également mieux encadrer l'implantation des cabines de téléconsultation et leur axe ça accessibilité en effet l'uberisation de la médecine ne peut pas constituer une solution de repli aux difficultés rencontrées en termes d'accès aux soins concernant l'hôpital, il était le grand oublié du texte initial, une loi de financement de la Sécurité sociale sans un financement de l'hôpital, il fallait quand même le faire heureusement vous avez présenté de modification à la hausse de l'Ondam 2022, j'allais dire il était temps, et enfin grâce au Sénat et malgré votre avis défavorable exprimée au sein de cet hémicycle et je vous remercie de l'avoir souligné, Madame la Ministre, le texte sécurise le garant, la garantie de financement de l'hôpital pour 2000 22 et prévoit un nouveau dispositif pour 2023 nous avons supprimé l'Ondam 2023 également pour cause de sincérité douteuse et par manque d'éléments nous permettant d'apprécier la situation dans son ensemble, les ajustements à la hausse de l'Ondam 2022 aurait dû vous inciter à la réflexion. Nous avons intégré également une clause de retour devant le Parlement, en cas de dépassement de l'Ondam de plus de 1 % en cas d'exercice en cours d'exercice par rapport au montant voté en loi de financement de la Sécurité sociale et, en cas de rétablissement de l'objectif dans la suite de la navette. Le Parlement ne peut se résoudre à laisser ces pratiques perdurer dans un souci de transparence et de lisibilité des comptes publics, le ministre de l'action et des Comptes publics nous a répété à plusieurs reprises lors de nos débats que chaque Euro comptait oui bien sûr, chaque Euro compte Madame la Ministre, pourtant vous avez refusé la proposition du Sénat de revenir devant le Parlement 100 de dépassement, ce sont 2 5 milliards d'euros. Nous avons voté la création d'une conférence nationale des générations de l'autonomie destinée à documenter les besoins des personnes âgées et des personnes handicapées afin d'entraîner la décision relative au financement des priorités qui appelle ses constats, c'est un sujet qui vous est cher mais néanmoins vous n'y adhérez pas les mesures relatives à la branche autonomie demeurent insuffisantes lors du passage du texte au Sénat, nous avions voté un certain nombre d'amendements visant à améliorer le contrôle des Ephad, ces amendements n'était que la traduction législative des préconisations issues de la mission d'information sur le contrôle des États dont le rapport a été présenté en juillet dernier par Bernard Bonne et Michel Meunier, vous annonciez vouloir vous emparer du sujet vous avez conservé un abonnement de notre collègue Bernard Bonne, plus que des paroles, nous attendons maintenant des actes, enfin nous avons institué une convention nationale pour l'emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraite et prévoyant les termes d'une réforme paramétrique, dossier cher à notre collègue René-Paul Savary, l'emploi des seniors est trop souvent minimisé dans notre pays. Or, il a des répercussions importantes dans de nouveaux domaines dans l'économie, la cohésion intergénérationnelle la transmission du savoir, la santé de nos aînés, regardez l'évolution de notre démographie, la question du travail des seniors demeure prépondérante concernant la pérennisation de notre système de santé, nous attendons que les promesses du gouvernement se matérialisent autour d'un texte ambitieux et pragmatique. Voilà, Madame la Ministre, un tour d'horizon des principales mesures votées par la Chambre haute, ces mesures ne sont ni démagogique ni rien irréalisable, elle s'appuie sur un travail sérieux mené lors de dizaines d'auditions de rendez-vous ces dernières semaines, ma question est donc simple : je reprenais je reprendrai pour cette occasion, une partie, une partie je dis bien du titre d'une chanson de Charles Trénet que reste-t-il, que reste-t-il du texte du Sénat sans suspense et cela a été dit, il ne reste rien ou si peu, et c'est vrai le 49 3, évoquée par nombre de mes collègues change tout, j'allais dire il chamboule tout, nous vous tendons la main en choisissant la voie de la raison et vous préférez une posture nombriliste qui n'augure rien de bon pour l'examen du futur texte au Parlement, vous l'aurez compris, madame la ministre, alors que les professionnels de santé, les professionnels du médico-social sont à bout de force, le constat est décevant et toute cette semaine de travail balayés d'un revers de la main, nous laisse un goût amer. Aussi, le groupe Les Républicains votera la motion proposée par la commission des affaires sociales, je vous remercie.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure générale, mesdames et messieurs les rapporteurs, madame la présidente de la commission, mes chers collègues ce PLFSS apporte pour moi des avancées pour les hôpitaux et nos concitoyens pour l'hôpital avec une augmentation de l'Ondam 2 3 7 % hors Covid cela pour le personnel et l'investissement entre 2012 et 2000, du fait, l'augmentation de l'Ondam était de 2 % je me permets de le rappeler. Concernant l'augmentation de cet Ondam 57 milliards entre 2017 et 2023, c'est beaucoup,

à augmenter les salaires des soignants cent quatre-vingt-trois euros et presque trois cents euros pour les aides-soignantes pour une somme de 13 milliards par an dans les hôpitaux, il y a un manque de personnel, c'est vrai, mais souvent beaucoup de postes sont financés ne trouvent pas preneur pour les médecins, infirmiers, les aides-soignantes, comme l'a indiqué le ministre un grand plan national de formation d'infirmier des soignantes et aussi de médecins mais malgré l'ouverture du numerus clausus n'a eu. On pas avant plusieurs années pour les soins, la quatrième internat dans les zones sous-denses mais ça aussi, c'est seulement en 2027. Et je le répète, la rémunération de nos interne pour cette dixième année doit être suffisante et devrait être égale à une consultation mensuelle à hauteur de l'équivalent de 10 consultations par jour, soit 5000 euros par mois dans le médico-social, et surtout, on n'est pas nous aurions espéré beaucoup plus de propositions d'emploi vu la grande dépendance qui nous attend et des pensionnaires actuels puisqu'il y aura de 200000 personnes ah j'ai été pendant de plus entre 2020 et 2030, c'est donc une déception de ce Plfss, mais nous avons écouté attentivement le Ministre de l'économie, qui nous a promis, dans cet hémicycle 50000 emplois pour le quinquennat et vous avez, Madame le Ministre, renouveler Il y a des avancées pour les familles avec l'âge des des conjugaisons Alizée la pas à domicile en hausse l'augmentation du complément mode de garde, la détection précoce du trouble du du rôle de développement, l'augmentation des pensions alimentaires minimale et pour la prévention 3 visites préventives a déjà des âges clés de la vie, dépistage des infections sexuellement transmissibles et du VIH, la pilule du lendemain gratuite pour toutes les femmes sans ordonnance et encore les vaccins sur prescription des pharmaciens, des infirmières et des sages-femmes. L'expérimentation aussi d'un accès Direct Direct aux infirmiers en pratique avancée dites à pas collaboration avec le médecin et aussi mobilisation des médecins retraités, avec exonération des cotisations retraite, tout cela me paraît utile, j'ai voté à titre personnel pour l'objectif d'équilibre des comptes de la branche retraite en prévision de déficit de 12 milliards d'euros en 25 et 15 en 2026 mais cela bien sûr après le dialogue avec les partenaires. Sociaux et ne pouvait pas figurer dans ce Plfss madame le reporteur souhaite maintenir. Le suivi de l'Ondam à l'année, moi j'y suis favorable, j'aurais souhaité que l'amendement du Sénat concernant Agirc-Arrco soit retenue, mais malgré tout, pour moi ce PLFSS à des avancées. Il me paraissait possible, d'abord une CMP conclusive pour ce Plfss 2023, cela n'a pas été le cas et dans cet esprit, les parlementaires pourraient aussi consacrer un peu plus de temps pour essayer de s'entendre sur ce texte, les indépendants s'abstiendront ou voteront contre, la question préalable merci.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, le désaccord entre la majorité relative à l'Assemblée et le Sénat en CMP, qui nous a conduits qui nous conduit à rediscuter ce texte nous a surpris, tant il semblait que la majorité sénatoriale s'était mise quand même au diapason avec le coeur, de vos projets, notamment en vous proposant de repousser l'âge de de départ à la retraite, a décidé néanmoins de repousser de quelques semaines c'était fiance, arguant de l'existence d'une concertation dont on sait d'avance le sort qui lui sera réservé ainsi après 4 49 3 le gouvernement aime rappeler qu'il n'obéit au jeu de la démocratie que lorsqu'il en fixe lui-même le cadre et les règles ah si le texte que nous retrouvons ici est un vrai camouflet pour la démocratie parlementaire, dont le seul tort est de vouloir jouer son rôle législatif si nous saluons les quelques avancées que le gouvernement a consenti à conserver dans ce PLFSS Post 49 3 coms alors important quand même, la compensation par l'État des exonérations de la prime de partage de la valeur des précisions apportées au rendez-vous de prévention correspondant en grande partie à ce que nous avions souhaité l'ajout d'une feu d'une phase transitoire après la fin de garantie de garantie de financement pour permettre aux hôpitaux publics de renouer avec leur activité ou bien encore, effectivement, la suppression de l'Arctique, repoussant l'âge de départ à la retraite, presque reste que nous déplorons que beaucoup d'ajouts du Sénat était quasi systématiquement supprimés, y compris ceux à enjeu très modeste, et ce sans justification par contre majeur, la chambre haute avait rejeté avec raison le transfert de plus de 2 milliards d'euros de charges de l'assurance maladie à la branche famille et que c'est dans plus qu'utile à la mise en place de politiques en faveur des familles modestes beaucoup plus ambitieuses que celles contenues dans ce PLFSS qui se restreint et seul mais aussi qui se restreint aux seules familles monoparentales alors qu'un enfant sur 5 est en situation de pauvreté en France, le Sénat avait aussi apporter des premières réponses aux impayés, tout ça, les assistantes maternelles en attendant l'instauration d'une garantie de salaire de la branche, mais c'est déjà trop, le Sénat avait supprimé l'article 44 qui permettait une extrêmement une extrapolation à partir des indus constatés et ainsi exiger des pénalités aux établissements de santé sur des dossiers non contrôlée un renversement de la charge de la preuve pour les établissements sur lesquels pèsera la charge de prouver la non-pertinence de cette extrapolation ces avancées ont été balayées, même si, enfin, le gouvernement a consenti une rallonge de l'Ondam hospitalier que nous avions défendu en vain au Sénat, et ce, pour une meilleure prise en charge des surcoûts Covid la rectification partielle de l'Ondam 2022 ne suffit pas à masquer un Ondam 2023 qui ne rattrape pas le retard des Budgets précédents, d'autant que l'inflation persiste et pèse sur l'investissement et de fonctionnement que la Covid amène des milliers de personnes toujours par an dans les hôpitaux publics et que les mesures d'urgence du rapport Brown sont prolongés, alors qu'elle devrait dès à présent pérenniser, nonobstant les avancées que nous avons cité le PLFSS 2023 souffre toujours d'un manque d'ambition pour relever les défis de la transformation de notre système de santé s'affranchissant enfin de logique comptable à très court terme

merci, cher collègue, la parole est à monsieur Martin lévrier. Pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour quatre minutes Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame, le rapporteur général, mes chers collègues en nouvelle lecture après échec de la commission mixte paritaire, les députés ont adopté sans vote la partie recettes du PLFSS après un recours à l'article 49 3 de la Constitution par madame la première ministre le nouveau texte, sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité est ainsi quasi identique à celui adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale aujourd'hui, bien que la majorité sénatoriale dépose une motion tendant à opposer la question préalable considérant que subsistent des points de désaccord sur des questions décisives, nous pouvons nous réjouir que l'Assemblée nationale n'est pas retenu l'amendement des réformes des retraites présentée par notre collègue René-Paul Savary, en effet, si les pistes retenues sont intéressantes : le gouvernement s'est engagé dans une concertation avec les partenaires sociaux pour déterminer les critères devant présider à une réforme, il est nécessaire d'atteindre l'issue de ces discussions pour trouver les meilleurs moyens de préservation de notre système de de retraite auquel nous sommes tous attachés de la rallonge de 543 millions d'euros destinés aux hôpitaux pour couvrir les surcoûts liés au Covid en 2022 de la conservation des 2 améliorations apportées par notre groupe en 1er lieu l'expérimentation pour une durée de 3 ans du versement au médecin, en complément de la rémunération à l'activité d'un forfait, financé par les fonds d'intervention régional un territoire ultramarin, il prendra part, afin de garantir la diversité des territoires investi dans ce dispositif, ainsi que leur représentativité, en second lieu, l'extension de la condition de durée minimale d'exercice dans un cadre autre que des missions d'intérimaires pour les professionnels de santé, mise à disposition auprès de d'un établissement de santé en France dans le cadre d'un contrat conclu par une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger. En responsabilité, le Sénat avait rien réintroduit l'annexe B qui a pour vocation de donner une visibilité et une stratégie pour l'avenir, cette mesure a été conservé à l'inverse des articles tout aussi pertinent avait été supprimé dans notre hémicycle et ont été réintroduits au cours de la navette, je pense notamment à l'article 24 24 pardon 24 terre qui permet l'expérimentation de l'accès Direct aux infirmiers en pratique avancée en structures d'exercice coordonné un décret devant préciser après avis de la Haute autorité de santé, les modalités de cette expérimentation et je pense bien évidemment à l'article 47 le vote en hémicycle a suivi la commission en rejetant les amendements de suppression de cet article, mais la majorité sénatoriale n'étant pas à un paradoxe près a ensuite fait voter la suppression de ce même article est éliminé de fait l'Ondam 2023, fixée à 244,1 milliards d'euros, faisant fi de tous les efforts financiers du gouvernement en faveur de notre système de santé. Bien qu'elle veuille mettre fin au débat, la droite sénatoriale pourra se réjouir de la conservation de l'article 8 qui acquiesce relatives à la taxe soda modulée en fonction du taux de sucre contenu dans les boissons concernées et de la conservation de l'amendement sénatorial visant à inciter les entreprises à se saisir des dispositifs de rachat de RTT. Cela étant, nous ne pouvons que regretter qu'un texte si important pour les Français, Madame la Ministre, l'a très bien résumé dans son discours de présentation ne puisse, pour la 6ème année consécutive, poursuivre son cheminement de la navette parlementaire pour ce faire, il faut une volonté partagée, or la majorité sénatoriale, en rejetant l'Ondam, en première lecture et de telle manière, ne laissait pas présager une forte envie de discussion notre attachement au débat parlementaire, l'emportant sur toute considération c'est sans surprise que nous voterons contre, la question préalable, je vous remercie. Si. Merci, cher collègue, la discussion générale est Close, nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Madame Élisabeth Doineau, au nom de la commission des affaires sociales a déposé une motion distribuée sous le numéro 6 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion, la parole est à madame la rapporteure générale pour la motion et pour dix minutes maximum. ça va être court, madame la président ça devrait être court, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, chers collègues, ce matin, réuni la commission des affaires sociales a décidé de proposer d'opposer la question préalable à à l'ensemble de la chambre haute, et donc je vais rapporter peut être quelques exemples, quelques raisons. Qui nous ont amenés à à prendre cette décision, en réalité, même si nous avons des des points d'accord et ça été rappelé dans l'expression de certains de nos collègues, il y a tout de même une certaine frustration à voir que le travail d'une semaine ici au Sénat a été balayé très rapidement par le gouvernement, on a donc considéré qu'il manquait un certain nombre d'éléments que nous avions défendu pendant quelques jours ici alors considérant que que si un accord est intervenu entre les 2 assemblées sur certains articles du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, des points de désaccord subsistent sur des aspects essentiels, considérant que le texte considéré comme adopté en nouvelle lecture, reprend le montant de l'Ondam pour 2023, que le Sénat a rejeté en première lecture en considérant qu'il était sous-évalué, considérant de surcroît qu'aucune des mesures de régulation, de renforcement du contrôle du Parlement en cas de dépassement de l'Ondam n'a été intégrée dans ce texte, considérant que la trajectoire financière quadriennal présenté par le gouvernement est incompatible avec l'objectif d'apurement de la dette sociale au 31 décembre 2033, considérant que le transfert de 2 milliards d'euros de charge de la branche maladie vers la branche famille ne se justifie pas et risque même de pénaliser comme ça a été dit par mon collègue rapporteur de branches, l'action de cette dernière branche en faveur des familles, considérant qu'il est indispensable que le Parlement se prononce sur le montant des dotations que les régimes obligatoires de base de sécurité sociale verse au fond aux organismes et aux agences qui le subventionne, considérant qu'il est nécessaire d'affirmer dès à présent, la nécessité d'améliorer l'emploi des seniors et de corriger les déséquilibres structurels de la branche vieillesse et de mobiliser l'ensemble des parties prenantes à cette fin dans les meilleurs délais considérant enfin que l'emploi systématique par le gouvernement de la procédure définie à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution ne permettra pas l'intégration de nouvelles propositions du Sénat en lecture définitive le Sénat décide donc qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Merci madame la rapporteure générale, quel est l'avis du gouvernement, madame la ministre. Sans surprise, l'avis du Gouvernement est défavorable. Merci, alors je vais passer la parole à Madame poncer mon jeu pour explication de vote chers collègues. Merci madame la présidente, alors le texte que nous nous propose de discuter revient au Sénat, après un nouveau 49 3 devant l'Assemblée nationale, mais aussi en supprimant une grande partie des amendements votés au Sénat si nous approuvons, nous l'avons dit quelques avancées, comme le maintien de la compensation par l'État des exonérations de la prime de partage de la valeur, la rallonge de l'Ondam, l'inscription d'une phase transitoire, face à la fin de la garantie de financement pour l'hôpital public reste que la question préalable au, delà de considérant que le groupe écologiste ne partage pas, point un désaccord profond sur la méthode qui a quel que soit des accords et des désaccords, que l'on peut avoir avec les amendements qui ont été adoptés au Sénat durant la première lecture bien sûr, je rappelle à titre d'exemple, notre opposition résolue à l'amendement relatif aux retraites reste que nous nous trouvons face à un gouvernement qui méprisent le travail parlementaire et il n'est pas envisageable que le Sénat délibère de nouveau, sachant que le gouvernement in fine et n'entend pas partager le pouvoir législatif des apports même d'enjeu mineur de la chambre haute, ont ainsi été balayé sans explication, les notes comme ceux d'autres groupes cette importation au Sénat de l'esprit du 49 3 brutalise le Parlement et présente un vrai danger en bafouant la démocratie parlementaire, il affaiblit, c'est une forme d'antiparlementarisme ainsi, ils ne sont pas que nous soyons dans des conditions favorables pour enterrer un sereinement une deuxième lecture et il est difficilement acceptable d'entamer notre travail dans la perspective que le Parlement sera encore déconsidérée, du fait de notre désaccord sur plusieurs considérons de fond le geste, le groupe écologiste solidarité et territoires s'abstiendra sur la question préalable, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame ah pour. Merci madame la présidente, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste ne votera pas cette motion tendant au rejet de la question préalable, même si nous avions déposé nous-mêmes une motion en première lecture, que vous auriez pu voter parce que finalement, quelle perte de temps, la majorité sénatoriale et le gouvernement n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le contenu du budget de la Sécurité sociale pour 2023, mais en réalité, on le sait, c'est un jeu de dupes d'un côté, le gouvernement campe sur ses positions et refuse toutes les modifications apportées apportées par le Sénat, y compris celle adoptée à la quasi-unanimité, comme le refus de transférer à l'Urssaf le recouvrement des cotisations des retraites complémentaires des cadres de l'Agirc-Arrco ou sur le refus de transférer 2 milliards d'euros de la branche maladie à la branche famille, de l'autre, la majorité sénatoriale, défend l'hôpital public alors qu'elle a adopté l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie pour 2023 qui est inférieur aux besoins des établissements, hé bien en deçà, rappelons-le, de l'inflation en réalité le gouvernement et la droite sénatoriale marchent ensemble. Pour attaquer nos retraites et se sont donnés rendez-vous à la rentrée 2023 hé oui pour allonger la durée de cotisation à 43 annuités si vous voulez bien me laisser finir après je vous écouterai et puis vous pourrez dire ce que vous avez à dire pour allonger la durée de cotisation à 43 annuités pour reculer l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans pour maintenir la décote jusqu'à 67 ans et pour supprimer les régimes spéciaux de retraite, bref autant de reculs sociaux qui vont pénaliser principalement les femmes, les précaires, les seniors celles et ceux qui ont des métiers pénibles et qui vont favoriser. Vous avez le sentiment des jeunes qu'ils n'auront pas même ce retrait merci, cher collègue. Alors je vais consulter le Sénat sur la motion tendant à opposer la question préalable, je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte en discussion en application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire et de droit et le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos. je donne le résultat du du scrutin, nombre de votants 343 exprimés 329 pour la motion 264 contre 65 la motion est adoptée et, en conséquence, le texte est considéré comme rejeté alors je vais suspendre la séance quelques instants pour permettre à chacun de s'installer pour l'examen du prochain point à l'ordre du jour, la séance est suspendue.

La séance est reprise, l'ordre du jour appelle l'examen des crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances et article 46 quater du projet de loi de finances pour 2023 la parole est à monsieur Arnaud Bazin, rapporteur spécial de la commission des finances a pour cinq minutes et je vais demander à chacun de rejoindre sa place et de de faire un peu de silence a pour notre collègue merci. Merci madame Merci madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2023 proposent ouvrir 30 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au titre de cette mission, cela représente une hausse conséquente de plus de 2 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2022, soit environ 8 % ça te hausse s'explique principalement par l'indexation à l'inflation du montant des prestations sociales financées par la mission, l'allocation aux adultes handicapés, la prime d'activité auquel il faut des désormais ajouter le RSA dans les départements où son financement a été recentraliser à elles seules, ces prestations représentent plus des 3 quarts des crédits de la mission ainsi le coût de la prime d'activité en 2023 dépassera le seuil symbolique de 10 milliards d'euros, ce qui est bien sûr le signe de la dynamique du marché du travail mais aussi de la faiblesse des salaires, les dépenses de d'allocation adulte handicapé, quant à elles dépasseraient les 12 milliards d'euros, la mission regroupe une grande variété d'actions qui reflètent la diversité de la politique d'action sociale pour le temps qui m'est un parti, je souhaite m'appesantir sur l'enjeu de l'aide alimentaire. Cette politique ne représente qu'une faible part des crédits de la mission avec 117 2 millions inscrits au PLF 2023, mais le sujet est crucial dans la période actuelle, en 2020 année marquée par la crise sanitaire, on estimait que 5 6 millions de personnes ont fait appel à l'aide alimentaire, le problème s'intensifient depuis l'inflation est très forte sur les produits alimentaires et fragilise considérablement nos concitoyens les plus modestes, la situation est également préoccupante pour les associations d'aide alimentaire, celles-ci sont en quelque sorte victime d'un effet ciseau entre un afflux de demandes qui ne faiblit pas et des moyens de plus en plus contraints en 1er lieu l'envolée des prix d'électricité alourdi fortement leurs charges de fonctionnement, tandis que la hausse des prix des carburants affecte les bénévoles se rendant sur le site de distribution surtout les tensions mondiales sur les marchés agroalimentaires sont à l'origine de nombreux lots fructueux dans les marchés passés pour leur compte par FranceAgriMer pour l'achat de denrées, je me permets une brève ainsi sur ce sujet de ses achats en principe éligible à un remboursement par l'Union européenne dans le cadre du FSE plus en pratique, les contrôles effectués en la matière sont si pointilleux qu'une partie significative des produits achetés finalement déclaré inéligible au remboursement, la simplification des procédures est absolument indispensable et cela fait maintenant plusieurs années, près de cinq, je crois que nous lançons l'alerte sur ce sujet avec Éric Bocquet dans ce contexte, il est indispensable de prendre des mesures de soutien efficace à cet égard nous nous félicitons certes que ce projet de loi de finances prévoit de renforcer de 60 millions d'euros, les crédits de l'aide alimentaire, nous avons cependant des divergences quant à la méthode retenue puisque cette enveloppe est destinée à la création d'un fonds pour les nouvelles solidarités alimentaire dédié à financer des projets de transformation des structures en lieu, en lutte contre la précarité alimentaire et soutien aux filières agricoles durables, il constitue en quelque sorte une issue au débat qui a eu lieu suite à la Convention citoyenne pour le climat autour de l'introduction d'un chèque alimentaire propositions que nous ne soutenons pas car elle tourne le dos au modèle français associatif fondé sur le couplage aide alimentaire et accompagnement social. Nous considérons qu'il conviendra de se montrer davantage pragmatique et d'utiliser cette enveloppe nouvelle pour soutenir directement le fonctionnement des structures, voire pour compenser de possibles aux infructueux dans l'esprit de l'enveloppe de 40 millions d'euros, qui avait pu être adopté cette année en et les faire sur une initiative de notre commission des finances, je suis loin de partager les orientations du gouvernement en matière de politique de cohésion et de solidarité, ce sont les revenus du travail qui permettent de sortir les personnes de la pauvreté et non d'échec ponctuel distribuées par l'état de temps à autre, même si le gouvernement a pris 2 fâcheuse habitude ces dernières années, mon collègue Éric Bocquet reviendra sur ce point, néanmoins en responsabilité et afin d'assurer le financement nécessaire de la prime d'activité et de l'allocation adulte handicapé, je vous propose d'adopter les crédits de cette mission. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Éric Bocquet, rapporteur spécial de la commune. Sur des finances pour cinq minutes aussi. Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes intéressés à la dynamique importante des crédits de la mission depuis 2019. Si nous tirons le bilan de la période récente, que constatons-nous chaque année depuis 2019 des enveloppes supplémentaires ont été ouvertes en urgence sur la mission d'abord en réaction au mouvement des Gilets jaunes avec une majoration de la prime d'activité qui représente un coût pérenne pour l'état d'environ 4 4 milliards d'euros par an ensuite pendant la crise sanitaire, avec le versement au printemps, puis à l'Automne 2020 et de 2 aide exceptionnelle de solidarité en faveur des bénéficiaires des minima sociaux et les aides au logement d'un montant de 150 euros avec une majoration de 100 euros par enfant à charge et représentant un coût de près de 2 milliards d'euros, enfin, en réaction à la forte accélération de l'inflation qui fragilise considérablement le pouvoir d'achat de nos concitoyens les plus modestes, de nouveaux dispositifs d'urgence ont ainsi successivement été financés sur la mission d'abord l'indemnité inflation fin 2021 qui cumule le défaut d'une aide à la fois limitée à cent euros très peu ciblé, elle s'adresse à toutes les personnes percevant moins de deux mille euros de revenus mensuels, sans considération des revenus du foyer et enfin très coûteuse pour le budget de l'État 3 8 milliards d'euros, dont 3,2 milliards financés par la mission. Plus récemment, et les faire 22 2022, une aide exceptionnelle de rentrée de un virgule 2 milliards d'euros, a ensuite été voté, nous avons dans cette commission assurément des visions très divergentes en matière de politique économique et budgétaire, je pense cependant que nous pourrons tous nous accorder sur un point : cette politique du chèque entre guillemets n'est pas une politique sociale, elle permet uniquement aux plus pauvres de nos concitoyens de passer le mois sans leur donner la moindre perspective et ne résout rien au problème de fond, le budget de la mission ne peut pas, à lui seul absorber les chocs sociaux qui trouvent leurs racines dans nos fragilités structurelles je pense en particulier à la question récurrente de la faiblesse des salaires, des points à quelques points positifs dans ce budget, je pense par exemple à la déconjugalisation de la H prévu à compter du premier octobre 2023, cette mesure était très attendue, on ne peut que regretter le temps perdu en la matière avant que cette réforme soit enfin arraché au gouvernement, à la faveur de la campagne présidentielle, cette mesure vient conclure un quinquennat qu'ont contractés en matière d'A. H puisque le la réévaluation la revalorisation pardon de son montant à taux plein de près de 80 euros a été contrebalancée par de discrètes mesures d'économie une revalorisation importante de la H a eu lieu en 2018 puis en 2019, relevant le montant mensuel de la location de près de quatre-vingt-dix euros pour le porter à un peu plus de 900 euros en 2021 sur le quinquennat cela représente un effort global de 3 milliards d'euros, même si elle est maintenue en dessous du seuil de pauvreté, mais en parallèle de discrets coups de rabot ont été décidées pour modérer l'évolution de la dépense, réforme du plafond de ressources des personnes en couple, suppression du complément de ressources sous-indexation de la revalorisation légale annuelle et caetera, ces mesures d'économie, il y a une capter plus du tiers de la dynamique créée par leur par la revalorisation de la H, soit environ un milliard d'euros sur les 5 ans. Pour de nombreux, nombreux bénéficiaires cette revalorisation a donc été largement théorique, en tout état de cause, son montant resterait nettement sous le seuil de pauvreté peut également être cité la poursuite de l'augmentation des crédits dédiés à la politique de lutte contre les violences faites aux femmes, les rapporteurs spéciaux relève la poursuite de l'augmentation des crédits en 2023 les crédits demandés s'élève en effet à 54 5 millions d'euros en autorisations d'engagement, soit une augmentation de 15 % par rapport à la loi de finances initiale 2022 le volume de l'enveloppe reste cependant bien modeste, eu égard à l'ampleur des enjeux et aux difficultés rencontrées par les associations de défense des droits des femmes qui sont également frappés comme beaucoup d'autres de plein fouet par l'inflation, à titre personnel, je m'en étais remis à la sagesse de la commission des finances sur l'adoption des crédits, la Commission comme vous l'indiquiez à l'instant, mon collègue Arnaud Bazin a décidé de vous proposer leur adoption. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean Sol, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales pour 3 minutes. Madame la présidente, mesdames les ministres, messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues, les crédits de paiement de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances s'élève à 29 virgule 9 milliards d'euros pour 2023, en hausse de 8,3 % par rapport à 2022 sous l'effet notamment de la revalorisation des prestations sociales et de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés c'était toutefois vrai la semaine dernière, mais un amendement du gouvernement déposé vendredi pourrait ramener cette hausse à 7 % nous espérons obtenir cet après-midi mesdames les ministres de plus amples explications sur la diminution de 568 millions d'euros des crédits dédiés à la prime d'activité et au revenu de solidarité active. Le budget de la mission, pour 2023 à Paris comme un budget de transition où l'on entrevoit des chantiers du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté, l'insertion et l'emploi. La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, arrive en fin de cycle et les crédits consacrés à cette action diminue de 327 6 millions à 252 millions d'euros en 2022, et dès 2023 les actuelle convention État département arrivant à échéance en cours dans mes mes nouveau pacte des solidarités prendrait la suite avec des axes nouveau concernant la lutte contre la grande marginalité et la transition écologique et solidaire, le gouvernement va lancer plusieurs expérimentations relatives au RSA qui ont vocation à converger vers le projet France dans des conditions qui ne se dessine pas encore avec évidence ne suivront également avec attention le projet de solidarité à la source, qui pourrait permettre de fiabiliser le versement des prestations sociales, s'agissant de la prime d'activité en particulier une amélioration du versement à bon droit, de la prestation est indispensable, selon la Cour des comptes en euros de prime d'activité sur 5, soit 2 milliards d'euros au total seraient versés à tort à titre définitif, par ailleurs, la commission a porté attention à la traduction budgétaire des avancées de la loi du 7 février dernier sur la protection des enfants, s'agissant des mineurs non accompagnés, alors que les flux d'entrée semble repartir à la hausse, la contribution de l'État aux dépenses des départements continuent à baisser de 93 millions d'euros en 2022 à 90 millions en 2023 sur tous les crédits inscrits en loi de finances sont sans rapport avec les dépenses réelles de l'État en 2022 sur les 28 millions d'euros qui ont été ouverts en compensation des dépenses supplémentaires à la charge de l'aide sociale à l'enfance, seuls 3 millions d'euros seront répartis entre les 11 départements ayant accueilli plus de MNA au 31 décembre 2021 par rapport au 31 décembre 2020, le mode de calcul de cette contribution doit être révisé car il était en complet décalage avec la réalité du terrain tous ces réserves, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable dire. Chers collègues, je ne peux pas donner des secondes et des minutes supplémentaires dans dans ce cadre là, je suis désolé, vous, si vous voulez revenir samedi ou dimanche, vous savez que le temps est très contraint alors dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque unité de discussion qu'on prend le temps d'intervention général et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de 10 minutes pour intervenir et la parole est à monsieur Philippe mouiller pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Madame la présidente, madame la ministre, Ministre mais c'est le rapporteur, mes chers collègues, s'il y a un domaine où l'effort de la nation ne doit pas faiblir, c'est bien celui de la solidarité, et cela d'autant plus vrai en cette période difficile, les crédits de la mission augmente de 8 % mais dans le contexte d'une inflation qui s'établit actuellement à 6 virgule 2 pour 100, il faut souligner également que la hausse correspond principalement à la déconjugalisation de la âge à la revalorisation des prestations sociales et à l'augmentation de la prime d'activité avec la crise sanitaire, économique et social, puis la soudaine baisse du pouvoir d'achat, la hausse du coût de l'énergie, chacun a pu mesurer combien de filet de protection sociale sont précieux, qu'il s'agisse d'un système de soins du chômage partiel de l'aide alimentaire ou dans la continuité des droits sociaux, malheureusement, malgré tout cela, environ 9,3 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France, le gouvernement a multiplié les mesures d'aide ponctuelle pour faire face aux urgences aide exceptionnelle de solidarité prime de rentrée majoration du chèque énergie primes d'inflation, cependant, ces aides ne remplace pas une réforme structurelle de lutte contre la pauvreté, comme l'ont souligné nos rapporteurs cette politique de chèques et d'aujourd'hui, certains de nos concitoyens, mais qu'en sera-t-il demain, quelles perspectives leur ouvre ton notre modèle social montre ici ses limites et le budget de l'État n'est pas inépuisable. Concernant les réformes envisagées, je voudrais former quelques observations et interrogations, le gouvernement a lancé plusieurs expérimentations relatives au RSA dans le sillage de 3 départements d'outre-mer, qui sont 2 heures déjà engagés dans cette voie, la loi de finances pour 2022 expérimente la recentralisation du RSA, la Seine-Saint-Denis et les Pyrénées-Orientales rejoint le dispositif qui prévoit que l'État reprenne le financement et la gestion du RSA sur une durée de 5 ans en contrepartie d'un renforcement des politiques d'insertion mise en Oeuvres localement cependant : la Cour des comptes juge inefficace de dissocier les responsabilités financières et opérationnelles et je souhaiterais avoir votre sentiment, Madame le Ministre, sur ce sujet et connaître les premiers retours d'expérience, une autre expérimentation prévoit de renforcer le contrôle et l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, la Cour des comptes a en effet pointé les défaillances alarmante du dispositif d'accompagnement en matière de retour à l'emploi, seuls 40 % des allocataires du RSA bénéficient de l'accompagnement social prévues par le dispositif, et seul un tiers des allocataires ont un emploi, 7 ans après leur entrée dans le dispositif, nous sommes favorables à un suivi qui soit enfin efficace, il faudra également s'appuyer sur le principe des droits et des devoirs pour les bénéficiaires qui adhère à leur parcours et qui soient donc moteur de leur insertion je souhaiterais maintenant formuler plusieurs remarques sur la politique en matière de handicap concernant l'allocation pour dites handicapé d'une hausse de 750 millions d'euros, tient compte des de mesures que nous avons voté dans la loi sur la protection du pouvoir d'achat, la revalorisation de 4 % pour, tenez compte de l'inflation et la déconjugalisation ces dernières mesures obtenues après un long combat parlementaire bénéficiera à 160000 de nos concitoyens, pour un gain moyen de 300 euros mensuels, elle permettra surtout d'assurer l'indépendance financière de la personne handicapée, celle-ci sera effective le premier octobre du 1023 et peut être même avant, comme vous l'avez indiqué en audition, Madame le Ministre, en matière d'emploi, on peut se réjouir qu'en 3 ans, le taux de chômage des personnes handicapées soit passé de 19 à 14 %, il reste cependant presque 2 fois plus élevé que dans la population générale, certaines entreprises s'engagent par une convention que quitte pas faire davantage de place au handicap, ils sont pas ailleurs que dernièrement les tensions du marché du travail incite les entreprises à embaucher des chômeurs en situation de handicap, pourriez-vous nous en donner quelques confirmations je dirais enfin que quelques mots sur la protection juridique des majeurs qui bénéficient actuellement à près de 1 1000000 de personnes souffrant de troubles psychiques en situation de handicap ou en perte d'autonomie, compte tenu du vieillissement de la population, ce dispositif pourrait concerner jusqu'à 2 millions de personnes en 2040, certes les crédits consacrés à cette protection sont en hausse de 9 % afin notamment d'augmenter les salaires et restaurer l'attractivité de la profession de mandataire à la protection juridique des majeurs, cependant les moyens nécessaires sont largement supérieur aux crédits votés actuellement près de 6500 mandataires se partagent plus de 390000 mesures par an ce que représente une charge de 60 mesures par mandataire et ce nom est difficilement compatible avec la qualité du service nécessaire pour assurer une réelle protection des personnes les plus vulnérables de notre société, c'est pourquoi je présenterai tout à l'heure un amendement pour transférer des crédits en conclusion, notre groupe, constate l'évolution des crédits de la mission et sera favorable, merci, madame. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Colette Mélot, pour le coup plus indépendants pour quatre minutes. Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues autour de 2 milliards d'euros de hausse, soit 8 % pour la mission Solidarité, insertion et égalité des chances dans le budget pour 2023. C'est à la fois un signe positif est aussi un marqueur de problèmes plus profonds pour notre société, nous traversons des périodes de crise importante la pandémie de Covid 19 a été pour beaucoup de Français le signe de la province à Pau appauvrissement pardon les menant parfois à des situations extrêmement difficiles, la guerre en Ukraine et les tensions énergétiques que nous subissons un Europe constitue un nouveau défi, beaucoup se demandent comment ils vont passer l'hiver, ainsi que les hivers prochains les risques de cette crise sur notre compétitivité sont visibles, le groupe, les indépendants, dès le 5 octobre dernier lors d'une question d'actualité au gouvernement, a alerté sur ce sujet qui laisse craindre de nouvelles délocalisations et des fermetures d'entreprises, la conséquence première seraient des licenciements et de nouvelles difficultés pour les Français, nous devons absolument préserver notre tissu entrepreunarial et faire en sorte que nos entreprises puissent rester sur notre territoire avec des emplois qu'elles créent le travail et surtout sa juste rémunération sont des moteurs au sein de notre société et doivent permettre de vivre correctement les réponses conjoncturelles via la multiplication des aides exceptionnelles sont importantes en ces temps de crises multiples cependant je partage l'avis qu'il faut penser à des évolutions structurelles, nous devons donner des perspectives aux Français et de l'espoir dans l'avenir, comme l'ont rappelé, dans leur rapport, les rapporteurs spéciaux dont je salue le travail nos discussions en commission des affaires sociales ont aussi révélé certaines failles de notre système, dans mes travaux j'appréhende de nombreux sujets via le prisme de la prévention, je crois qu'il faut également le faire sur les sujets de la solidarité de l'insertion et de l'égalité des chances, la lutte contre la pauvreté, c'est aussi de trouver des solutions afin qu'elle ne s'installe pas ce qui me paraît essentiel sur ce point, je crois beaucoup en la formation et un un encadrement qui doit permettre de reprendre pied dans la vie active et de ne pas laisser un cercle vicieux s'installer alors que nous allons négocier les nouvelles générations de conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, je pense qu'elles doivent être adaptées au plus près des problématiques de chaque territoire pour être efficace, je suis particulièrement attentive à la situation de nos jeunes, nous avons entendu leurs difficultés très importantes après la pandémie et maintenant face à l'inflation et au coût de l'énergie dans ce cadre, je salue les crédits supplémentaires via le financement d'un fonds pour les nouvelles solidarités cependant comme beaucoup il me semblerait important dans la situation actuelle de soutenir plus directement et donc plus rapidement des les associations dédiées à l'aide alimentaire, les bénévoles font un travail extraordinaire, malgré les contraintes toujours plus forte, et malheureusement le nombre croissant de personnes devant y recourir, d'après l'Insee, cela concerne entre 2 et 4 millions de personnes, je souhaiterais aussi évoqué le rapport alarmant de l'UNICEF et sur ce point, il y a beaucoup à faire concernant l'enfance un dernier point pour terminer, il faut signaler que les crédits concernant la hache pour 2023 seront les premiers après la réforme de la déconjugalisation nous devons redonner des perspectives aux Français et lutter contre la pauvreté, de manière préventive, il y a tant à accomplir afin de répondre aux problématiques structurelles de notre système, cependant, la hausse des crédits de cette mission est une bonne nouvelle et le groupe les indépendants votera en faveur. Merci, cher collègue, la parole est à Madame, Mélanie Vogel pour le groupe écologiste solidarité territoire pour quatre minutes. Merci madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, la mission nous examinons aujourd'hui devrait contenir les grandes actions de l'État visant à éradiquer la pauvreté et l'exclusion et la discrimination dans notre pays, certaines propositions budgétaires sont évidemment bienvenus, je pense à l'augmentation de l'allocation ajoute handicapé la reconduite des 5 millions de budget alloué à la lutte contre la précarité menstruelle depuis l'adoption de l'amendement de ma collègue Raymonde Poncet mange via la loi de finances 2021, l'augmentation du budget alloué aux 39 19 le lancement de l'expérimentation territoire 100 pour 100, accès au droit, ces mesures vont nature naturellement dans le bon sens, mais la réalité politique, c'est qu'elles n'émanent principalement, pas de vous, elles sont en réalité l'émanation de victoire que nous avons remporté contre vous, l'augmentation de l'enveloppe de la hache et due à sa déconjugalisation, qui a été obtenu après une campagne acharnée des associations contre votre gouvernement le budget dédié à la lutte contre la précarité menstruelle et le maintien d'un dispositif que nous avions fait adopter, il y a 2 ans, contre l'avis du gouvernement, l'augmentation du budget du trente-neuf 19 se situe dans la lignée de votre renoncement à préserve tissé sa gestion suite également à une forte mobilisation, ce n'est donc pas ici l'expression d'un projet mais d'arbitrage ponctuels liés à 2 ponctuels défaite du reste, il n'y a pas vraiment dans cette mission de politique volontariste pour réduire la pauvreté, l'exclusion et la discrimination le manque de moyens dédiés à la solidarité en France est affligeant, quand on sait qu'il y a près de 10 millions de pauvres une inflation galopante et des bas salaires qui stagnent pour lutter efficacement contre la pauvreté, il aurait fallu ouvrir le RSA aux jeunes de moins de 25 ans rehausser le RSA et lâche au niveau du seuil de pauvreté, supprimer des contreparties au RSA pour lutter contre le non-recours et garantir à chacun le minimum vital, au lieu de ça, l'assurance chômage assurera moins bien le RSA sera conditionné, vous vous obstinez dans une réforme des retraites anti-redistributive et injuste, le budget de la prime d'activité est un aveu de son échec à faire sortir les travailleurs et travailleuses pauvres de la précarité, le manque de moyens dédiés à l'égalité femmes-hommes est aussi frappant Georges je relirai donc cette demande des associations féministes 0 virgule 1 % du PIB pour lutter contre les violences subies par 50 % de la population sur l'égalité professionnelle tellement reste à faire, notamment en menant des politiques visant à faire l'égalité salariale, non pas seulement dans les entreprises, mais entre les secteurs, ensuite nous notons des baisses de financement justifier de façon obscure, une baisse de 50 % de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine au motif d'un faible recours c'est bien connu, en baissant des aides déjà faible, on améliore le recours à celle-ci baisse là encore du budget dédié à la stratégie interministériel de prévention et de la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, n'empêchera les enfants pauvres d'être pauvre en leur retirant l'argent mais aussi l'extension programmée de la formation des métiers de la santé et du soin, avec la suppression des autorisations d'engagement, c'est vrai qu'on n'a aucun besoin en santé, c'est bien connu et puis lorsque vous augmentez des Budgets, on sait pas exactement trop comment ça va se passer, je pense par exemple au fond pour une alimentation alimentaire durable, qui est une bonne chose, la manière dont les 60 millions d'euros vont garantir que les produits concernés seront réellement durable et peu clair, or l'alimentation c'est un déterminant majeur de la santé et c'est quasiment exclusivement dépendant du niveau social, plus on est pauvre, moins on a accès à des produits sains, plus on est malade, et tout ceci est dans un système où l'alimentation fournie aux plus pauvres et qui les rend malade rend aussi malade notre planète pour toutes ces raisons, et ayant pesé le pour et les contre le geste s'abstiendra sur les crédits de cette mission. Mais si la parole est à monsieur Xavier Iacovelli pour le groupe. Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour quatre minutes. Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, dans ce projet de loi de finances 2023 la mission Solidarité, insertion et égalité des chances se dote de moyens conséquents pour la mise en oeuvre de plusieurs chantiers prioritaires dans la continuité de ce qui a été entrepris dans les précédentes lois de finances en terme de petite politique sociale de nombreux sujets d'importance sont concernés par cette mission, je pense notamment au financement attribue en matière de protection de l'enfance inhérent à son bon fonctionnement et son organisation, le groupement d'intérêt public France Enfance protégée sera mise en oeuvre au 1er janvier 2023, ce nouveau Jeep s'appuiera sur une gouvernance associant l'État, les départements, mais aussi les représentants des associations, nous l'avions voté en début d'année et je me félicite que cette année de se clôture par l'examen de crédits permettant son financement, je tiens ici à souligner les moyens mobilisés pour la protection de l'enfance, afin de répondre à la diversité des situations difficiles auxquelles ils doivent faire face, 4 millions permettront de financer le plan de lutte contre les violences faites aux enfants, afin de financer notamment l'utilise l'unité pardon d'accueil pédiatrique, enfants en danger 140 millions pour la mise en oeuvre de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance à travers la contractualisation avec les départements afin de sécuriser leur parcours des enfants protégés de fluidifier l'accompagnement scolaire mais également de faciliter l'accès au logement et aux droits des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance je souhaite revenir sur un constat que j'avais fait devant vous depuis maintenant 2 ans chaque année des milliers de jeunes sont victimes de sorties sèches, faute de contrat jeune majeur et d'accompagnement des départements, les chiffres sont d'ampleur 70 pour 100 des jeunes de la de sortent sans diplôme 100 des sans domicile fixe de moins de 25 ans ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance ainsi, c'est pour moi essentiel que sa mise en oeuvre des c'est des mesures pour faire face à cette situation, et c'est ce que nous avons fait lors de l'examen de la loi relative à la protection de l'enfance, aujourd'hui, le budget que nous avons qui nous est soumis prévoit 50 millions pour fléchés pour prévenir les sorties sèches des jeunes majeurs de la dessus je ne peux que me satisfaire de voir ce financement assuré sa mise en place et sa mise en oeuvre ce projet de loi de finances porte également un financement à l'aide alimentaire abondé en 2023 de 60. Millions supplémentaires, améliorer la qualité de l'offre et s'assurer que tous les moyens soient déployés pour lutter contre la précarité alimentaire, ce devait être au coeur de notre action, la mission Solidarité prévoit. également le financement de mesures de lutte contre la précarité menstruelle qui concerne environ 1,7 1000000 de femmes l'enveloppe de 4,7 millions assurera la distribution de protection aux populations précaires, la collecte et la redistribution par des associations, mais aussi la sensibilisation de la population, la mission porte également sur le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes, grande cause du quinquennat avec notamment une hausse de près de 15 % des crédits pour répondre aux enjeux multiples, en terme d'accueil et d'orientation des victimes et leur mise en sécurité à travers plusieurs mesures, la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, comporte également le financement de l'allocation adulte handicapé, dont l'augmentation des crédits depuis 2017 marque l'engagement du gouvernement les crédits permettront de financer la déconjugalisation de la que nous avons voté cet été, nous portons aujourd'hui également avec mes collègues Hassani et Mohamed Souani un amendement visant à harmoniser les modalités d'accès à la hache à Mayotte et le territoire national, en proposant d'étendre la décongèle agace déconjugalisation pardon de la H sur le territoire mahorais, mais également de supprimer l'obligation de résidence d'un an pour pouvoir y prétendre. La mission illustre la volonté du gouvernement d'assurer pleinement l'égalité des chances, elle démontre l'ampleur des moyens mis en oeuvre. Pour poursuivre les actions des solidarités engagé ces dernières années, elle porte enfin une réalité derrière des mots, des petits pas et des grandes avancées pour protéger nos concitoyens dès leur plus jeune âge, de la violence de la précarité. Et d'exclusion notamment enfin sa saison je d'envergure, les crédits proposés nous semble adéquate pour assurer la mise en oeuvre d'une politique publique ambitieuse dans le domaine et c'est pourquoi le groupe RDPI c'est cher quand même tiendra pleinement les mesures et l'orientation de cette mission. La parole est à madame Annie Le Houerou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour six minutes chers collègues. Madame la présidente, mesdames les ministres, chers collègues. Depuis ce début d'année, la guerre en Ukraine et ses conséquences de la crise énergétique angoisse les Français, selon les derniers chiffres du cabinet IRI publié dans Le Monde, l'inflation atteint 11 96 % et 11 96 % et dépasse même les 12 % sur le seul rayon alimentaire en novembre, dont 16 9 % sur les produits frais, les inégalités sociales se creusent 20 pour 100 des personnes les plus modestes dispose en 2019, 2 8 7 % des richesses alors que les 20 % les plus aisés en personne en perçoivent 38 % la mission Solidarité, insertion et égalité des chances que nous examinons aurait pu être l'occasion de mettre en place des mesures sociales fortes et ambitieuses pour lutter efficacement contre ces inégalités pour 2023, les crédits alloués à la mission s'élève à 29,9 milliards d'euros, en progression de 8,3 pour 100, il finance principalement la chez la prime d'activité, le programme 300 quatre consacré à l'inclusion sociale et à la protection des personnes, voit ses crédits augmenter à hauteur de 10 08 % cette hausse qui paraissent significatives est en grande partie liée au financement de la réponse à l'urgence engendrées par la crise économique et sociale actuelle et sont loin de couvrir l'inflation dans le cadre de ce programme, l'action 14 dédié à l'aide alimentaire est en hausse de 106,7 pour 100, mauvaise nouvelle, car le nombre de bénéficiaires augmente l'aide alimentaire en France concerne 5 5 millions de personnes, un chiffre sous-estimé par rapport aux besoins réels, la demande d'aide alimentaire restant une démarche difficile et mal connu, sur ces 5 5 millions de personnes les le réseau des Banques alimentaires permet d'des des 2 millions de personnes face à la flambée des prix, mais aussi à l'explosion du nombre de bénéficiaires, la Fédération française des banques alimentaires nous alerte et craint de ne pas faire face à la demande, le groupe socialiste, écologiste et républicain proposera une augmentation des crédits alloués à l'aide alimentaire et en particulier pour le soutien aux initiatives de solidarité alimentaire territorialisée l'action 19 qui concerne la stratégie interministérielle, il y a de la, de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes s'élève à 252 millions pour 200 pour 2023, soit une baisse de 23 % par rapport à 2022, nous déplorons cette baisse regrettable et inquiétante quand on sait que 3 millions d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté, soit un enfant sur 5 dans notre pays, il y a donc plus qu'urgence à agir pour que chaque enfant en France vivent et grandissent dignement, nous proposerons donc un amendement pour augmenter les crédits alloués à cette action et pour donner à la politique de protection de l'enfance, les moyens de ses ambitions : nous proposons également un amendement pour abroger les règles restrictives d'Aix d'accès au RSA jeune et ainsi à l'ouvrir aux 18 25 ans cette mesure constituerait un filet de sécurité efficace pour ces jeunes qui subissent un taux de chômage à plus du double de la moyenne, du fait de problèmes de formation de mobilité, une réponse aux étudiants qui viennent rallongé les files d'attente de l'aide alimentaire, s'agissant du programme 157 qui concerne le handicap et la dépendance 14 milliards d'euros, ils sont consacrés pour 2023, une hausse qui tient compte de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé et de la revalorisation de celle-ci, à hauteur de 4 pour % actée dans le projet de loi, mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat, mesures que nous avons largement soutenu néanmoins le montant moyen servie aux allocataires de la H atteint selon l'adresse 759 euros sur une base de un virgule 28 millions d'allocataires. Cela signifie que la grande majorité des allocataires de la hache vit en dessous du seuil de pauvreté, évalué à 1102 euros alors que cette allocation est censé leur permettre de vivre dans la dignité, nous proposerons donc d'augmenter cette allocation pour qu'elle atteigne le seul le seuil de pauvreté s'agissant du programme 137 qui coordonne les actions relatives à l'égalité entre les femmes et les zones, il est en hausse de 54 avec 154,4 millions d'euros de crédits alloués l'action 25 de ce programme finance la prévention et la lutte contre les violences et la prostitution pour 2023, les crédits alloués à cette mission s'élève à 29 millions d'euros, soit une hausse de 17,54 6 millions d'euros sont alloués à la lutte contre la prostitution, dont 200000 euros pour accroître le nombre de bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion professionnelle, la FIS cède cette aide s'élève à 330 euros par mois, là encore, comme pour la H ce montant est trop fait pour aider les personnes en situation de prostitution à en sortir et à mener une nouvelle vie, nous proposons donc de revaloriser cette aide à hauteur du montant de revenu de solidarité active, c'est-à-dire 598 euros Nous saluons cette hausse globale du programme 137 consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais elle ne permet pas de répondre aux besoins nécessaires pour lutter contre les inégalités de genre ni pour créer par exemple un observatoire des féminicides qui a tant attendu, il conviendrait de redoubler d'efforts de financement au vu de l'ampleur des besoins et d'une priorité du quinquennat les res les ressources nécessaires aux associations qui Havre de son dans ce domaine sont trop limitées, c'est pourquoi nous demandons une augmentation des crédits à hauteur de 1 milliard qui correspond au budget supplémentaire nécessaire est évalué par les associations qui se battent au quotidien pour lutter contre les violences faites aux femmes, globalement, les crédits alloués à cette mission Solidarité, insertion, égalité des chances demeurent largement insuffisants et ne permettront pas à nos concitoyens les plus vulnérables de vivre dignement et d'espérer un jour sortir de cette précarité en guise de conclusion je vous vous citerai la phrase de Michel en 1871 s'il y a des misères de dans la société, c'est que la société dans laquelle nous vivons et mal organisé, on ne peut pas admettre qu'il y ait encore des gens qui crèvent la faim quand d'autres ont des millions Merci, cher collègue,

avec près de 30 milliards d'euros, les crédits de la mission progresse de 2 milliards d'euros par rapport à 2022, l'examen des crédits en faveur des personnes les plus fragiles, dans un contexte social extrêmement préoccupant, avec un fort taux de chômage avec plus de 10 millions de personnes pauvres et un taux d'inflation de plus de 6 % doit nous alerter les prix flambent et les pertes en pouvoir d'achat ce considérable pour une large majorité de la population, les indicateurs sont au rouge, pourtant, le gouvernement refuse de regarder cette réalité en face et refuse d'augmenter le SMIC de rétablir l'impôt sur la fortune ou de taxer les superprofits l'augmentation des inégalités sociales dans notre pays entre les plus riches et les plus précaires, porte un coup de canif à notre pacte social face à la crise de la pandémie, le gouvernement a été capable de débloquer 200 milliards d'euros pour les entreprises, et aujourd'hui, alors que des millions de familles peuvent basculer dans la précarité ou la grande précarité, seulement 2 milliards d'euros supplémentaires seront versés aux personnes handicapées, aux jeunes sans emploi et aux personnes vulnérables les crédits de la mission progresse, principalement en raison de la revalorisation anticipée des prestations sociales de 4 % intervenue au 1er juillet 2022 alors que le nouveau de l'inflation sur l'année 2022 approche les 5 cela veut dire que les ménages les plus précaires ont perdu du pouvoir d'achat en 2022, le niveau de l'inflation est qualifiée par la Banque de France de jamais vu depuis les années 1980 cela mérite un investissement public à la hauteur des besoins, ce qui n'est malheureusement pas le cas, notre groupe ayant déposé des amendements sur cette mission, je concentrerai mon propos sur les jeunes et les moyens de contrôle des agences régionales de santé, comment pouvons-nous nous satisfaire des crédits de la stratégie interministériel de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes quand tu l'Insee indique que dans notre pays près de 3 millions d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté, selon l'UNICEF, que 8000 enfants vivent dans des bidonvilles l'état doit assurer à toutes et tous les moyens de vivre dignement et en particulier à nos jeunes, nous savons que des milliers de jeunes de l'aide sociale à l'enfance sont obligés de dormir à l'hôtel, en raison de la suffisance des moyens d'État ces jeunes subissent la violence des réseaux de prostitution et de raquette, il faut donc plus de moyens pour mieux les protéger pour nos anciens, ce n'est guère meilleure : le gouvernement se vante d'augmenter les crédits de personnel de contrôle des pas des agences régionales de santé après l'affaire Orpea mais les cinquante inspectrices et inspecteurs qui seront recrutés en 2023 ne remplaceront pas les 2000 postes supprimés depuis 2010 dont 400 entre 2014 et 2021 en 20 ans la politique de réduction de personnel a entraîné une baisse de 30 % des effectifs des corps d'inspection et une baisse de 39 pour 100 des médecins inspecteurs le renforcement des contrôles nécessiterait de revoir à la hausse les moyens des agences régionales de santé pour compenser ces pertes, mais aussi pour renforcer les effectifs des conseils départementaux chargés du financement des Epad l'avancée concernant la déconjugalisation de la H pour laquelle nous nous sommes battus nous et que nous saluons ne contrebalance malheureusement pas les mesures, les mesures négatives que je viens d'évoquer pour l'ensemble de ces raisons, notre groupe votera contre les crédits de la mission, pour 2023 je vous en remercie.

Ah, le président a même litre messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission Solidarité, insertion, égalité des chances est au coeur d'une mission humaine pourtant les politiques publiques, solidarité et de cohésion sociale envers les personnes les plus vulnérables, c'est l'une des plus importantes de missions du budget de l'État, comme l'a souligné d'ailleurs la présidente Catherine Deroche des crédits demandés au titre cette mission s'élève à, pour 1900 2023 29,9 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une hausse de 8,3 % par rapport, loi de finances pour 2022 importante dynamique constatée cette année sur les dépenses de mission porté par l'inflation et la revalorisation des pensions, illustrent la mise à contribution majeure de cette mission pour faire face à l'urgence sociale, on ne peut que soutenir les dépenses d'intervention de la mission au bénéfice des personnes plus fragiles, sans occulter cependant que l'infraction quand le ressenti par les populations les plus fragiles dépasse le taux d'inflation constatée, toutefois, comme le souligne le rapporteur des crises successives, mettre en lumière la vulnérabilité de notre modèle social lui-même, le budget de l'État ne pouvant seule absorber les chocs sociaux les interventions répétées, un cours de gestion, souligne le défaut de rôle stabilisateur de notre système de prestations de solidarité, Madame la Ministre, quels enseignements tirez-vous de ces crises successives et quelle réponse pérenne aux urgences sociales, hein des vous porté

le programme 157 Handicap et dépendance contribuera également à soutenir les établissements et services d'aide par le travail à hauteur d'un milliard et demi qu'on a une on suivent 6,4 % notamment par l'augmentation du SMIC et 2023 verra la réalisation des mesures bienvenue au plan de transformation des actes dans un contexte économique des plus difficiles pour nos concitoyens touchés par la hausse du prix de l'énergie et des denrées alimentaires qui s'ajoute à la crise post- Covid je voudrais souligner, à la question majeure de l'aide alimentaire en effet au lendemain des collectes de dons pour les banques alimentaires auxquels nous sommes nombreux sur ces bancs, à avoir participé dans nos territoires, nous avons pu mesurer l'inquiétude sur les capacités de générosité des Français, l'augmentation des ménages les plus précaires, les associations d'aide alimentaire de plus en plus sollicités moi le profil des bénéficiaires évoluer étudiants personne seuls travailleurs modestes 7 personnes sur 10 sont des femmes, la demande n'augmenter de 9 % on peut mieux semestres 2022 pour les banques alimentaires et de 15 % pour les Restos du coeur, selon les chiffres de la Commission, l'approvisionnement constitue également une inquiétude en raison de la hausse des prix de l'énergie qui touche singulièrement les associations et des tensions sur les marchés agricoles depuis le début de la guerre en Ukraine, augmentation des fois européenne dédiée à l'aide alimentaire, le FSE plus doté de 647 millions d'euros sur la programmation 2000 22027 et fragilisée par l'inflation et la multiplication de l'OM fluctuer, privant les associations de volumes de denrées de 67 millions d'euros depuis 2021 certes comment compenser en loi de finances rectificative pour 40 millions d'euros, quelles mesures comptez-vous mettre en oeuvre pour améliorer l'approvisionnement et simplifier les procédures et qui font peser un cadre normatif très contraignant sur les associations le font pour les nouvelles solidarités alimentaire qui doit être créée en 2023 avec un volet national pour les territoriales pour développer les raisons des solidarités alimentaire et les guerres avec les producteurs locaux est encore incertain, pouvez-vous nous préciser le calendrier et les modalités de fonctionnement en fait à ce qui concerne le programme 137, égalité entre les femmes et hommes représentant une part modeste la mission, je tiens à souligner la hausse des crédits de 14 % par rapport à 2000 22 et leur doublement depuis 2019 la priorité donnée à la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, l'accueil et l'aide à la mobilité des victimes, le renforcement du réseau d'écoute la plateforme téléphonique que son total Nappi au programme bon groupe parlementaire soutiennent pleinement ces mesures dans la proposition de loi devant les les Valérie Létard a été adoptée le mois dernier a ainsi le type de ma collègue Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes, nous avons déposé des amendements appelant à revaloriser la subvention allouée au Centre d'information sur les droits des femmes et les familles et l'ensemble des métiers, financé par le programme aussi dans ces conditions, le groupe Union centriste votera les crédits de cette mission, qui vise à lutter contre la précarité, réduire les inégalités et protéger les personnes les plus vulnérables, je vous remercie. madame la présidente. Mesdames les Ministres Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans cette période de crise économique et sociale que nous traversons, il est important d'avoir un regard particulièrement exigeant sur cette mission, les chiffres, nous les avons devant les yeux et nous les connaissons, plutôt que de se réjouir dans un budget s'élevant à 29,9 milliards d'euros pour 2023, j'aimerais comprendre pourquoi le programme 137 pourtant, sur l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas plus important d'ailleurs, vu la diversité des sujets de cette mission je m'attarderai plutôt sur l'égalité femmes-hommes, les enjeux sont immenses : comment expliquer que, dans notre société encore aujourd'hui des femmes meurent parce qu'elles sont des femmes depuis le début de l'année 2022 il y a eu 121 féminicides dont 62 conjugaux, les moyens accordés sont certes en hausse mais demeurent insuffisants même Emmanuel Macron vendredi dernier, avouer, je le cite, qu'on pouvait faire mieux pour lutter contre les violences conjugales, il y a quelques semaines, je rendais visite à l'association Halte aide aux femmes battues, j'ai rencontré un personnel associative bénévoles incroyable engagé et prêt à tout pour aider ces femmes brisé toutes les associations de violences faites aux femmes : vous voulez clame depuis plusieurs années déjà le milliard, ce à quoi vous répondez par une augmentation des crédits alloués du trente-neuf dix-neuf, alors même que la Fédération nationale solidarité femmes qui gère le numéro d'appel a fait état d'une hausse de 14 % des appels par rapport à 2019 où est donc votre logique budgétaire et votre promesse de faire de la cause des femmes votre priorité la crise inflationniste ne distingue pas les gens, certes, mais force est de constater que l'emphase la enfin l'inflation impact plus grandement les femmes que les hommes, elles représentent près de 64 % des recourant à l'aide alimentaire et 72 % de ceux qui recourent au colis et aux épiceries sociales ajoutons à cela que les femmes représentent environ 3 quarts des bas salaires, en effet, de toutes les personnes touchant le SMIC en France 62 % sont des femmes, c'est très révélateur révélateur de notre modèle social cela demande une nouvelle fois que nous sommes loin de répondre à l'extérieur à l'exigence d'égalité homme femme pourtant garanti par notre Constitution depuis 40946 mesdames les ministres, le combat contre les inégalités salariales et sociales n'ait pas dépassé et mérite d'être accentuée par plus d'efforts, plus de moyens et plus d'ambition, je m'abstiendrai. Cher Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, hein : janvier dernier le président de la République déclarer : nous devons lutter contre un enracinement de la pauvreté, qui a signé une peur du quotidien et autres toute perspective d'avenir, c'est dans cet esprit que la mission Solidarité, insertion et égalité des chances se mobilise des crédits indispensables pour affronter les crises et assurer aux plus fragiles d'entre nous une certaine dignité, un 2023, les crédits de la mission augmentent et atteignent un peu plus de 29 milliards d'euros, notamment pour accompagner les mesures contre l'inflation, telles que la revalorisation de 4 % des aides sociales ou la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés, mais dans ce contexte social préoccupant, la question du Nord au cours de prestations sociales et prégnante aussi il me paraît plus que jamais indispensable d'aller chercher celles et ceux qui ne savent pas celles et ceux qui renoncent face à la complexité ou l'illectronisme des campagnes mieux ciblées et plus s'impose 1 2021 25 pour 100 des plus jeunes n'ont pas eu accès à une aide à laquelle ils avaient droit l'expérimentation des territoires 5 pour accès au droit permettra, je l'espère, d'enrichir notre arsenal de lutte contre le nord au cours mais je pense que nous devons nous diriger vers une automatisation des premiers versements quand cela est possible, vers des déclarations et des guichets uniques pleinement décentralisé et contrôlable, les politiques publiques de la solidarité s'en trouverait renforcée, mes chers collègues, vous me permettrez 3 remarque sur des programmes spécifiques de la mission concernés la location du 15 handicapés, nous nous félicitons de Andréa Ricoeur de la déconjugalisation de la H, même si celle-ci n'interviendra qu'en octobre 2023,

proposé aux femmes qui doivent être accompagnées pour une nouvelle vie, or les femmes victimes de violences conjugales en milieu rural sont les grandes oubliées de la lutte contre les violences faites aux femmes, elles souffrent d'un isolement à la fois géographique et moral qui les fragilise un plus encore une enquête régionale montre ainsi 50 % des féminicides survenus hein Nouvelle Aquitaine aurait lieu dans ces zones rurales où ne vit pourtant qu'un tiers de la population de la région, 600000 euros déduit pour 2023 à ces actions dans la réalité, ne sommes pas à mon sens tout à fait à la hauteur de la protection due à ces femmes, dernière remarque alors que les banques alimentaires d'assurer le week-end de collecte plus difficile que prévu et que le rapport de l'IGF de novembre 2022 attestent d'une hausse des produits alimentaires de 10 % à 12 % en décembre, l'urgence est bien là, les boucliers associatifs et des collectivités locales ne peuvent prendre le relais quand la vague est trop forte, or la question du chèque alimentaire durable et sur la table depuis le 3 novembre 2022 le fonds pour une aide alimentaire durable 60 millions d'euros, souhaitée par la Première ministre devait être gérés à travers des projets locaux, nous demandons que cette mesure annoncée puisse aller vite, je souhaiterais également que ces chèques puissent être utilisés pour payer la restauration collective et les cantines scolaires, permettant ainsi aux enfants les plus fragiles d'avoir au moins un repas équilibré par jour au-delà de ces remarques notre groupe votera cette mission budgétaire, je vous remercie. Voilà. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Catherine Bell Rithy pour le groupe Les Républicains et pour cinq minutes.

Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la mission Solidarité, insertion et égalité des chances du PLF 2023 et doté de 29 8 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 29,9 milliards d'euros en crédits de paiement ces crédits sont respectivement en hausse de 1 8 milliards d'euros et de deux 3 milliards d'euros par rapport aux crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2021 cette mission regroupe 4 programmes importants l'inclusion sociale et protection des personnes ou les crédits de la prime d'activité augmente d'un milliard Handicap et dépendance dont les crédits augmentent de 6 % et supporte notamment le coût de la déconjugalisation de l'allocation ou z'autres handicapés égalité femmes-hommes, dont l'augmentation de 14,95 % faire notamment renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et améliorer l'accès aux droits, ce qu'il faut saluer conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales dont la dotation supporte en partie la hausse du point d'indice de la fonction publique et la valorisation du schéma d'emplois pour 2023 la généralisation de ces augmentations s'explique par le rôle d'avant-garde de cette mission budgétaire face à la crise sanitaire et sociale que nous avons traversé, sur laquelle nous ne reviendrons pas ici, en revanche, les dépenses exceptionnelles alimente d'autant plus cette augmentation dans le contexte de la crise économique actuelle, marquée marquée par une hausse généralisée des prix la hausse budgétaire de cette mission, poursuit donc son ascension en 2023 à partir d'objectifs très hétérogène, tantôt structurelle et liée à des objectifs de long terme de nos politiques publiques telles que la lutte contre la précarité, la recentralisation du Revenu de Solidarité Active l'égalité femmes-hommes et la protection de l'enfance, tantôt ponctuelle et destinée à protéger le pouvoir d'achat des Français tantôt circonstanciel et dépendant d'aides exceptionnelles, telles que la revalorisation anticipée des minima sociaux de 400 millions et l'aide exceptionnelle de rentrée de plus d'un milliard Acton tout d'abord que les crédits alloués à la prime d'activité et à l'allocation aux adultes handicapés représentent l'essentiel des crédits de la mission, pour 76 virgule 8 % la prime d'activité qui a remplacé la prime pour l'emploi, ainsi qu'une partie du revenu de solidarité active soutient le pouvoir d'achat des travailleurs modestes à hauteur de 10 milliards pour près de 4 6 millions de foyers, l'allocation aux adultes handicapés bénéficient quant à elles d'un dynamisme liée aux viennent ici Isman démographique et à l'extension de la reconnaissance du handicap, mais il faut souligner le poids de la déconjugalisation de cette allocation enfin adopté en revanche l'augmentation générale et continue des crédits de cette mission subit le coût des mesures exceptionnelles qui requiert une vigilance accrue. Plan d'urgence en matière alimentaire d'enfance de violences conjugales, s'y ajoutent notamment l'indemnité inflation des 1000 euros à toute personne percevant de moins de deux mille euros de revenu Net mensuel et des aides exceptionnelles dont on ne dressera pas la liste ici ici 4, dispositif exceptionnel se sont succédés en moins de 2 ans, or ces dépenses ponctuelles sont directement imputables à une politique du chèque, laquelle ne parvient pas à dissimuler ce que nos collègues rapporteur Arnaud Bazin et Éric Bocquet honte éloquemment appeler des fragilités à double titre d'une part, fragilité du rôle de l'État qui ne saurait se borner à absorber de manière exceptionnelle, mais surtout perpétuel des chocs sociaux et économiques, d'autre part, fragilité de l'intervention de l'État qui s'est trop souvent abstenu de politiques structurelles, en particulier à l'égard du chômage, du sous-emploi et de la faiblesse des salaires. En conclusion, nous voudrions donc insister sur la vigilance du au budget de cette mission, dont l'augmentation marquerait l'apparition d'un État amortisseurs et dont les politiques publiques se réduiraient au poids budgétaire d'une politique du chèque. Il faut, bien au contraire tourner nos travaux vers la Laboral, l'élaboration de politiques de long terme, nous voudrions souligner l'effort budgétaire à poursuivent concernant l'égalité femmes-hommes, d'une part et d'autre part, le financement du futur groupement d'intérêt public France Enfance protégée: celui-ci a fait l'objet des amendements salutaire des commissions des finances et des affaires sociales du Sénat, je vous remercie. Merci, cher collègue, alors nous allons donné la parole à mesdames les ministres, je vous rappelle que vous avez un temps global de dix minutes maximum ah vous partagez et que bien entendu je couperai la parole à la à la dernière donc le le décompte par à dix minutes et je donne la parole à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Merci madame la présidente d'Amel les ministres. Messieurs les rapporteurs mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ce premier examen des crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, mobilise 3 ministères, cela montre l'importance des politiques qu'elle finance qui permettent de mener des actions concrètes en matière de lutte contre la pauvreté, de réduction des inégalités, de protection des personnes vulnérables en conciliant le court et le long terme dans un contexte où le coût de la vie pèse sur nos concitoyens, nous avons fait le choix de protéger ceux d'entre eux qui sont les plus fragiles avec les crédits de cette mission, en hausse de 7,8 % pour 2023, soit plus de 2 milliards d'euros supplémentaires et le programme 304 inclusion sociale et protection des personnes, voit son budget augmenter de près de 1 milliard cette hausse se permet de financer la revalorisation de 4 % des prestations sociales que vous aviez voté à nous dernier ainsi que la montée en puissance de la prime d'activité mais elle acte aussi la création du fonds pour l'aide alimentaire durable doté de 60 millions d'euros, qui vise à réduire l'impact environnemental, tout en faisant de l'aide alimentaire, un outil central de lutte contre la pauvreté

la période de forte inflation nous oblige par ailleurs à des mesures d'urgence une enveloppe exceptionnelle a été débloqué à hauteur de 10 millions d'euros pour financer 300000 colis alimentaires permettant à un étudiant de se nourrir pendant une semaine, autre grande priorité à laquelle je suis évidemment attachés l'accompagnement des personnes handicapées ce PLF accroît de 6,4 % soit 845 millions d'euros les moyens dédiés à leur accompagnement sur le programme 175 Handicap et dépendance parmi les grandes dépenses financées, il y a bien évidemment l'allocation adulte handicapé, pour un total de 12 milliards et demi d'euros avec une hausse de 750 millions d'euros pour tenir compte de la revalorisation de 4 % mais aussi de l'individualisation de l'individualisation à venir de la autre axe majeur, un milliard et demi d'euros dédié à la garantie de rémunération des travailleurs handicapés à Neshat ce budget nous permet de conduire une réforme structurelle pour fluidifier les parcours professionnels des personnes accompagné en Esat et nous entendons encore l'amplifier ce budget finance enfin l'emploi accompagné dispositif auquel je crois beaucoup et qui est un levier indispensable pour viser l'amélioration de l'emploi des personnes en situation de handicap, il apporte le soutien nécessaire à l'insertion et à leur maintien dans leur poste de travail, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je veux, pour finir, insister sur l'importance des politiques financées par cette mission, leur impact est immense dans la vie des Français les plus vulnérables, mais ces politiques ont aussi beaucoup de sens pour les agents publics, ces hommes et ces femmes qui les déploie sur le terrain, au quotidien, il est indispensable pour le pays que le secteur social et médico-social dispose de personnel qui soit formé à ces enjeux très précis et qu'ils soient en nombre suffisant, c'est pourquoi la mission Solidarité accueil des moyens supplémentaires dédiés en cohérence avec ce qui est fait en PLFSS il s'agit de pérenniser des postes cruciaux par exemple ceux des renforts dédié à la crise Covid Covid afin de pouvoir capitaliser demain sur des compétences précieuses en matière de pilotage et de gestion des crises, il s'agit également de recruter des équipes au sein des ARS, notamment pour renforcer les missions de contrôle en Ephad, nous partageons tous ici la conviction que notre système de soins et de solidarité repose d'abord sur les hommes et les femmes qui s'engagent auprès de leurs compatriotes les plus vulnérables, je vous remercie. Merci, la parole est à madame Isabelle Rome ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes de la diversité et de l'égalité des chances. Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs, monsieur le président de la commission des finances, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, programme de l'égalité avec un E majuscule le programme 137 dont j'ai la responsabilité s'articule autour de 3 axes forts : la lutte contre les violences d'égalité économique et professionnelle et la culture de l'égalité, permettez-moi tout d'abord de me réjouir de la hausse du budget dédié au ministère dont j'ai la responsabilité, cette progression s'élève à 7 3 millions d'euros dans le cas du projet de loi initial, ce qui représente 15 % supplémentaires par rapport à 2022, pour atteindre 57 9 millions d'euros, l'augmentation du p 137 s'inscrit dans un continuum depuis 2017 au total en 5 ans le programme 137 aura progressé de plus de 95 % c'est la traduction en acte de la grande cause des 2 quinquennat du président de la République, ces moyens supplémentaires permettront notamment de renforcer les aides aux associations dans le cas du PLF 2023 un effort budgétaire important d'un million six sera ainsi consacré au réseau de la FNC idée ff pour atteindre 6,3 millions d'euros, 600000 euros de crédits supplémentaires permettront de développer la démarche de l'les vers, si important dans nos territoires ruraux joue périphérique 3 6 millions deux euros de crédits nouveaux seront consacrés à l'intensification de la prévention et lutte contre les violences, permettez moi aussi de m'arrêter sur le 39 19 la plateforme d'écoute et d'orientation, des victimes dont le gouvernement a étendu les horaires, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un effort supplémentaire de 2 9 millions d'euros permettra de soutenir l'action de la FNSF et du dispositif d'écoute en parallèle les actions de prévention et de lutte contre la prostitution seront renforcées, notamment via une augmentation de 200000 euros afin d'accompagner la hausse du nombre de bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion professionnelle, le gouvernement propose un abonnement sur pour ouvrir la compensation du Ségur aux structures associatives de la branche de l'action sanitaire et sociale dont font partie les associations oeuvrant dans le Champ de l'égalité femmes-hommes, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, le financement de l'ensemble des actions en faveur de l'égalité femmes-hommes dépasse le simple cadre du programme 137, comme l'indique le document de politique transversale, ce sont 3 3 milliards qui sont alloués à la politique d'égalité du gouvernement, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, je me réjouis que le Sénat se saisissent avec autant de détermination de la grande cause des quinquennat du président de la République, un enjeu qui dépasse les clivages partisans, je vous remercie. Merci la. Parole est à madame Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargé de l'enfance. Madame la présidente, monsieur le Ministre Mesdames les Ministres monsieur les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, l'enfant, c'est une priorité du gouvernement c'est une politique éminemment interministérielle la première ministre a d'ailleurs réuni la semaine dernière le 1er comité interministériel de l'enfance, avec l'ensemble des ministres concernés, nous avons déterminé 40 mesures structuré en 3 axes : lutter contre les violences faites aux enfants, garantir l'égalité des chances et agir pour le développement et l'avenir de tous les enfants. Sur le plan financier, évidemment, les crédits de l'enfance sont portés par de nombreux ministères, mais aussi par les départements et les collectivités locales, c'est pourquoi je porte dans le PLF 2023 3 sujets : le 1er celui de créer un jaune budgétaire sur l'enfance, le gouvernement a d'ailleurs porté par amendement à l'Assemblée Nationale ce projet, cela me semble indispensable pour enfin avoir une vision complète de l'ensemble des financements mobilisés par l'État mais aussi par les collectivités locales, la seconde priorité, c'est le maintien des crédits de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance, incluant le renforcement de la prise en charge des jeunes majeurs à hauteur de 190 millions d'euros, 2023 sera une année d'évaluation et d'élargissement de la contractualisation à des acteurs essentiels que sont l'éducation nationale et la justice nous réfléchissons par ailleurs à la contractualisation avec des territoires particulièrement exposés, comme les territoires d'outre-mer ou de la couronne francilienne. Nous avons porté le l'augmentation des emplois avec les autres ministres sur le terrain pour améliorer le pilotage de l'action de l'État et des contrôles, c'est le 3ème axe qui eux que je sollicite, c'est une priorité, l'État doit prendre sa place dans l'accompagnement des départements, et plus particulièrement dans le contrôle des établissements de protection de l'enfance, c'est donc 31 emplois qui sont demandés dans les services des dettes qui s'ajouteront aux 20 employes sollicité sur une autre mission pour la protection judiciaire de la jeunesse, ce projet de loi de finances a ainsi pour objectif de consolider et renforcer la politique de l'enfance, aux côtés des départements des autres collectivités territoriales et bien sûr des nombreux acteurs engagés dans cette politique. Merci, merci, madame la Ministre et bravo pour avoir suivi le timing, hein, sincèrement. Alors, nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, figurant à Ali Thabet, alors je vous rappelle que pour cette mission, la conférence des présidents a fixé la durée maximum de la discussion à 2 heures 30 et que celle-ci été porté exceptionnellement hier à 3 en conséquence, si nous n'avions pas terminé l'examen de cette mission à 19 heures 20, celui-ci se poursuivrait à la fin d'émission de cette semaine et nous passerions à l'examen de la mission santé en revanche, si nous terminions avant le terme de cette durée, l'examen de la mission suivante pourrait commencer sans attendre, je vous remercie et nous passons à l'amendement 730 présenté par le gouvernement, monsieur le Ministre. Merci madame la la présidente, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, avant d'ouvrir l'examen des amendements de fond déposés sur cette mission Solidarité, je vous propose d'en ajuster le niveau global pour une question de sincérité, il me semble en effet important de tenir compte des dernières prévisions sur lesquelles le gouvernement s'appuie et des dernières évolutions acté notamment en lien avec les collectivités locales, je vous propose ainsi de faire évoluer les crédits pour 2023 de cette mission à hauteur de 470 millions d'euros, un niveau substantiel, mais qui traduit un certain nombre d'évolutions que je souhaite détaillé tout d'abord une actualisation des prévisions de la CNAF en matière de recours à la prime d'activité et au revenu de solidarité active de telles actualisation sont somme toute classique et celle-ci est en l'occurrence, liée à l'amélioration de la situation du marché du travail observée ces derniers mois, dont nous pouvons je pense toutes et tous nous féliciter, il ne faut bien sûr y voir ni triomphalisme alors que nous venons de continuer à avancer collectivement vers le plein emploi, ni remise en question des droits des individus, les autres évolutions vont, quant à elle, dans le sens d'une augmentation des crédits avec par exemple l'entrée du département de l'Ariège dans l'expérimentation de recentralisation du RSA pour un montant de 40 millions d'euros ou encore la compensation d'une partie des revalorisations salariales décidées en février 2000 22 et supporté par les départements, c'est une soulte de 14 millions d'euros que nous avons discuté avec les départements dans le cadre du comité des financeurs, que nous inscrivons dans ce texte, et enfin une revalorisation salariale de 3 % pour tous les opérateurs relevant de la branche de l'action sanitaire et sociale donc le secteur privé non lucratif financée par cette mission, revalorisation qui est équivalente à celle de l'augmentation du point d'indice dans la fonction publique, donc, pour 38 millions d'euros toutes ces ouvertures de crédits sont indispensables pour que l'État puisse tenir ses engagements en matière de prestations sociales de revalorisation salariale ou de recrutement d'agents publics, l'amendement qui vous est proposé montre donc bien à mon sens, tant la responsabilité que l'ambition de ce gouvernement au moment de finaliser le budget de l'État pour 2023. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente. Mesdames les Ministres Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'impact à la baisse des crédits, vous l'avez cité monsieur le Ministre de l'Ordre de 470 millions d'euros principalement due à la révision des prévisions que nous ne sommes pas en mesure d'expertiser mais qui engagent votre gouvernement en tout état de cause, le RSA, la prime d'activité étant des droits ouverts, j'aurais tendance à dire que, peu importe les montants inscrits de toute façon ces droits devront être servi, cependant je souhaitais vous interroger sur les 14 millions d'euros que vous avez évoqué au titre de la soulte due au département après la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social, si cette somme semble conforme à ce qu'attendent les départements ceux-ci souhaitent toutefois connaître les modalités de la répartition de cette somme, si vous pouvez nous l'a précisé, de toute façon ce sera un avis de sagesse de la commission. Merci monsieur le ministre. Oui, je peux répondre immédiatement la le mode de répartition de cette somme leur appartient, puisque nous avons décidé avec ma collègue, Charlotte Caubel lorsque nous avons réuni le comité des financeurs qui leur appartiendrait de définir dans le cadre de l'assemblée des pas des départements de France, la répartition de de l'enveloppe, je crois qu'il y avait un débat entre un mode forfaitaire ou un mode ou réel de la répartition de cette enveloppe. Merci, alors je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement qui a reçu un avis de sagesse de la commission qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est donc adopté 34 amendements faisant l'objet d'une discussion commune: l'amendement 422 Monsieur Merci madame la présidente, mesdames les ministres, en France, on compte plus de 3 millions de personnes nouvellement de chaque année, un quart des deuils se complique ou deviennent pathologiques des conséquences sanitaires, sociales, économiques du seuil sont lourd pour les nuits comme pour la société dans cet amendement propose de développer une politique publique de prévention des risques liés au deuil et de le doter de nouveaux crédits permanents d'offrir un accompagnement psychologique adapté aux personnes en deuil qui le souhaitent de former les professionnels, à un meilleur accompagnement. Vous pouvez continuer monsieur Ro. Et le 2ème, c'est un amendement de repli. Très bien, merci l'amendement 534 madame Le Houerou madame Meunier, merci madame la présidente. Monsieur le Ministre Mesdames les Ministres, cet amendement vise à doter dignement notre politique de protection de l'enfance, par des moyens derrière lui donnant les moyens de ses ambitions, les dépenses par rapport aux montants d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement proposé par le gouvernement dans l'action, 19 ont diminué, et ça ne peut être acceptée, d'autant que la protection de l'enfance va mal et on lui demande de plus en plus, la loi de 2022 demandent à juste titre d'accompagner les mineurs jusqu'à l'âge de 21 ans par les conseils départementaux, l'inscription en priorité pour obtenir un logement social, etc, or le besoin principal remonté par les acteurs du terrain, que ce soit en maison d'enfants à caractère social ou ou dans les familles d'accueil, nous disent le besoin de moyens supplémentaires moyen d'investissement bien sûr mais surtout moyens humains, des éducateurs, des éducatrices notre amendement repose aussi sur la conviction que ces 250 millions d'euros de dépenses supplémentaires proposées sont des dépenses qui, finalement, ce seront des dépenses d'investissement puisque dans l'avenir, nous aurons moins de dépenses de santé publique, par exemple, ou de politiques d'insertion ou d'accueil des jeunes laissés à l'abandon, donc nous proposons ce prélèvement de 150 millions sur l'action 17 du programme 124. Merci l'amendement 424 monsieur c'est exactement le même que les 2 premiers sets même hein propose donc d'abonder ce nouveau programme de 201 millions d'euros en minorant l'action 17, financement des agences régionales de santé du programme ça 24 conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales et l'action homme pris 11 prime d'activité autre dispositif du pouvoir me 3 5 4 inclusion sociale et des personnes chacune de 100 millions 500 1000 euros à un acte d'engagement, rien qu'au CP. Merci l'amendement 533 madame Meunier c'est. Un amendement de repli si on peut dire, puisque c'est un amendement qui propose de doter de 125 millions donc la moitié de ce que je viens de dire, sur la stratégie interministériel de prévention de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Merci le cent cent 35, c'est ma Meunier même Le Houerou. Défendu, je le prends, madame la présidente, le 535 abonde un nouveau programme intitulé font de prise en charge psycho-trauma causé aux enfants suite à des violences sexuelles et à des violences intrafamiliales à hauteur de 100 millions d'euros, la prise en charge des psycho-trauma chez l'enfant, suite à des violences sexuelles ou des violences subies dans le cas familiale est une politique d'ambition, la création d'un tel font de prise en charge ne doit pas être perçu comme une charge nouvelle mais comme de futurs économies je viens de le dire pour des Budgets de la Nation et des comptes sociaux, les conséquences des traumatismes sont abondamment décrit chaque année en France 165000 enfants sont victimes de viols et de violences intrafamiliales seulement 4 pour 100 dépose plainte et moins de 1 % des plaintes aboutissent aux assises, autrement dit, l'impunité est quasi totale, la réparation est quasi inexistante en tout cas fortement retardé faute de repérage attends pourtant le traumatisme lait traumatisme sont réversibles et plus ils sont pris à temps et précocement et plus ils ont de chances d'être soigné, guéri, en tout cas trouver une certaine résilience si on on reste impuissant face aux risques vitaux encourus, il y a également un risque pour la santé mentale et la santé physique de ces jeunes futurs adultes il est défendu il donc il bon un nouveau programme intitulé cellule de conseil et de soutien pour les professionnels, destinataire de révélations de violences sexuelles de la part des enfants à hauteur de et on l'a entendu, notamment à Nantes dernièrement aux assises nationales sur les violences, ce sont des révélations qui se poursuivent tout au long de la vie. Et l'amendement 539 madame Meunier. Il s'agit là aussi d'un amendement concernant le repérage systématique le fond de repérage systématique des violences sexuelles auprès de tous les enfants, par tous les professionnels à hauteur de 5 millions d'euros, et ça c'est un amendement qui nous a été soufflée par la syphilis, la commission inter-ministérielle, les victimes des infractions sexuelles, abus sexuels, violence sexuelle caractère familial. Merci, alors nous avons 3 amendements identiques alors le premier le 385 Monsieur

de personnes souffrant de troubles psychiques 30 % des personnes en situation de handicap et 22 % ce sont des personnes en perte d'autonomie, donc la moitié des mesures de protection 497000 en 2020 sont exercées par 8300 mandataires dont 80 % sont salariés de services associatifs aujourd'hui près de 6500 mandataires judiciaires de protection des jeunes majeurs des services associatifs se partagent plus de 390000 mesures par an dont 60 chacun, donc le nombre est difficilement compatible avec le maintien de au niveau de qualité pour les personnes concernées donc afin d'agir concrètement pour la protection donc juridique et faire à ces constats d'urgence cet amendement propose d'abonder de 95 millions d'euros, la dotation versée par l'État au service associatif cette revalorisation devant entériner le recrutement de 1000 800 professionnels pour passer de 60 à 45 mesures géré par mandataire judiciaire de protection des jeunes majeurs, permettant ainsi de baisser la charge de travail, mais surtout de maintenir la qualité du service, donc il est proposé d'attribuer ces 95 millions de crédits

sur l'action 12 et de 47 plein du 5 millions sur l'action onze merci. Merci monsieur Roux pour le 416 il est bien défendu,

Oui, madame la présidente, effectivement, cet amendement défendu mais je voulais rajouter quelques points pour le défendent davantage pourquoi parce que l'exemple de mon département, la Haute-Saône, illustrent parfaitement les conséquences mise en cause par ce ce cet amendement si on prend le cas de la Haute-Saône ou une désaffection du métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs était effective de par la surcharge de travail et par l'absence de valorisation des responsabilités en effet ces mandataires sont aujourd'hui rémunérés sous le le fait de la grille de la classe de la convention 66 qui elles-mêmes ignorent le métier de mandataire et donc ils émargent en tant qu'éducateur spécialisé, ce qui fait, qui sont sous-rémunérés, rien que pour vous donner un exemple : depuis 2019 sur les 14 mandataire que comptent les services de la Haute-Saône dix ans démissionner et sur les recrutements, un seul a pu se faire à travers un mandataire qualifié, ce qui signifie qu'il y a eu beaucoup de temps et beaucoup d'argent dépensé pour former de nouveaux mandataires les tribunaux nous annonce mandatement qui va augmenter la révision régulière des mesures permet certes d'adapter des mesures de protection à l'évolution des situations mais cela génère un flux entrée sortie mal pris en compte avec du retard dans la tarification, les mandataires Hosono à suivre, à ce jour 53 personnes en moyenne et nous ne connaîtrons qu'en juillet de l'année prochaine, le montant du budget accordé donc si nous ne pouvons embaucher pour prendre en charge les mesures supplémentaires à qui d'ici là. Pour conclure, les personnels motivés à la base dans le choix de leur métier, par l'aide aux personnes vulnérables sont en souffrance de ne pouvoir avoir les moyens de mener à bien leur mission, c'est la raison pour laquelle j'ai cosigné je voterai cet amendement merci madame. Merci le 548 madame Le héros. Oui merci madame la présidente, c'était également un abonnement qui concernent la protection juridique des majeurs : la moitié des mesures de protection sont exercées par 8300 mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont près de 80 pour 100 sont salariés des services associatifs, les projections actuelles montre un besoin d'anticiper les conséquences, notamment du vieillissement de la population aujourd'hui donc près de 6500 mandataires judiciaires, la protection des majeurs se partagent 390000 mesures par an soit 60 mesures par mandataire donc les crédits ne permettent pas de d'assurer en fait le besoin qui était évalué à 1800 professionnels supplémentaires devraient être recrutés pour faire face aux besoins est passé de 60 à 45 mesures donc ben voilà c'est le l'objet de l'amendement, c'est de rétablir ces crédits. Merci l'amendement soixante Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, on est dans la même logique, une demande de crédit supplémentaire avec un montant différent, peut être un peu plus raisonnable, auteur au regard des enjeux simplement par cette intervention, c'est surtout pour appeler la crise de la situation qui est extrêmement difficile sur le terrain, beaucoup de maires nous ferons monter des difficultés pour avoir des interlocuteurs beaucoup de prise en charge qui sont décalés, parfois même incapacité d'avoir des contacts dans les structures associatives pourtant qui essaie de faire un maximum d'efforts, mais elles sont submergés par la situation et à la fois on a évoqué lui sont de la population, mais c'est également la situation économique et sociale qui est aujourd'hui de plus en plus difficile qui entraîne bien en complément des problématiques plutôt psychique et bien des difficultés sur le territoire et donc la nécessité de la mise en place de professionnels pour pour accompagner ces majeur a protégé, voilà, donc c'est vraiment un cri d'alarme de la profession, c'est également quelque part un cri d'alarme des élus locaux et avec un grand principe général plus nous prendrons en considération les besoins sur le terrain tu au moins ça coûtera à notre société, nous sommes dans un texte budgétaire et je crois qu'il faut l'entendre merci.

la période Covid nous a fait prendre conscience des inégalités criantes en terme d'accès à une à l'alimentation durable et de qualité, l'inflation cette année est venu exacerber cette situation préoccupante, selon les dernières données de liste de l'Insee, donc l'augmentation des prix alimentaires, approche approche les 12 % selon les produits, les effets sur la santé d'un manque d'accès d'accès à une alimentation de en quantité ou qualité suffisante sont aujourd'hui bien connus, avec pour conséquence une double peine pour les ménages en situation de précarité ce fonds vise à soutenir des dynamiques multi-partenariale, alors que l'ingénierie, l'investissement sont souvent soutenus par des appels à projets ce fonds vise à soutenir des frais de lancement, mais aussi de fonctionnement ingenierie frais d'administration et surtout toutes les dépenses liées aux besoins d'animation et de formation pour de véritables effets de participation des personnes. Madame Le Houerou le 549. à 149 concerne la revalorisation de l'ensemble des métiers, financé par le programme égalité entre les femmes et les hommes, les associations financées par ce programme se retrouvent exclus du périmètre de revalorisation salariale, je crois que ça a été revu depuis, pour autant, je pense qu'il faut impérativement revaloriser ces métiers pour permettre également à à ces métiers d'être attractif et rémunérer correctement parce que les métiers du social, et particulièrement pour prendre en charge les personnes et les femmes victimes de violence sont.

au sein de différentes structures majoritairement associative, je pense par exemple aux accueils de jour spécialisé, mais aussi aux lignes d'écoute pour les victimes, sans oublier les permanences juridiques et sociales déployée partout France, le programme 137, égalité entre les femmes et les hommes, vise à soutenir l'ensemble des métiers permettant à c'est 800000 femmes de recevoir l'aide précieuse dont elles ont besoin, en février 2022, les associations financées par ce programme ont été exclus du périmètre des revalorisations salariales des métiers du social et du médico-social, porté par l'État lors de la conférence des métiers, or l'absence de mesures de revalorisation pour l'ensemble de ce secteur menace à terme la qualité et la continuité de l'accompagnement de ces femmes et de ces victimes, à cela s'ajoute le manque d'attractivité des métiers du secteur social, toutes catégories confondues, ça entraîne des sous-effectifs inquiétant donc ça été déjà expliqué donc cet amendement vise donc à revaloriser l'ensemble des métiers, financé par le programme égalité entre les femmes et les hommes en généralisant la prime du Ségur social je vous remercie. Merci l'amendement 710 Madame Cohen. que s'agissant de la grande cause du quinquennat le gouvernement ne maintiennent pas la progression des crédits en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes des années précédentes, quoique déjà insuffisante mais qui était, je vous le rappelle, pour 2022 de 22 % et pour 2021 de 37 % ce regret est d'autant plus vive que dans le détail des actions budgétaire la ligne pour l'égalité entre les femmes et les hommes diminue en réalité de 1 7 % % alors que dans les mots, je crois que nous sommes toutes et tous convaincus du poids de l'éducation pour faire progresser l'égalité : seulement 4 millions d'euros sont prévus pour financer des projets territoriaux destinés notamment à déconstruire les stéréotypes sexistes et promouvoir la participation des filles dans les domaines où elles sont peu représentées voir invisibiliser par contre 11 4 millions d'euros sont prévus au profit de l'entreprenariat des femmes et du développement de la culture, de l'égalité dans les entreprises, 2 poids, 2 mesures, pourquoi un tel une telle différence pour nous ces combats ne sont pas contradictoires, donc notre amendement d'appel vous invite à à revaloriser l'ensemble des métiers qui sont financés par le programme égalité entre les femmes et les hommes en généralisant la prime du Ségur de 183 euros pour un montant de 16 millions d'euros, et je vous rappelle que, aujourd'hui, les femmes sont toujours payé 15 % de moins en moyenne que les hommes à poste équivalent, il est temps en 2022, de faire un geste dans cette mission que l'on examine pour combler ce retard, je vous remercie.

l'Établissement et service d'aide par le travail des ESAT peut bénéficier d'une aide versée par l'nos fonds d'accompagnement de la transformation des établissements et service d'aide par le travail, Fateh Sat pour soutenir leur transformation en 2022, le montant des crédits dédiés à flot font s'élevait à 15 millions d'euros inscrit dans le cadre du plan de relance, or ces crédits ne sont pas reconduits en 2023, du fait de la fin du du plan de relance, et si nous proposons d'augmenter de 15 millions d'euros, la dotation allouée à l'action, allocations, aides en faveur des personnes handicapées du programme Handicap et dépendance afin de poursuivent leur transformation entamée dans de bonnes conditions pour les travailleurs ah Merci beaucoup, le 541 Madame le héros. suite aux circulaire du 11 et 13 mai 2022 les établissements ISAT peuvent bénéficier d'une aide versée par le nouveau fonds pour soutenir leur transformation, le montant des crédits dédiés aux Fateh that s'élevait à 15 millions d'euros dans le cas du plan de relance, or le bleu budgétaire ne nous permet pas de de voir que ces crédits seront reconduits pour 2023, 2 questions se posent à celle du montant dévolu à la mise en oeuvre en 2023 des projets déjà sélectionnés, ainsi que la poursuite de la réforme de la transformation des ESAT afin de de poursuivre la transformation entamée dans de bonnes conditions pour Les Travailleurs en Esat, cet amendement vise donc à ce qu'une enveloppe au moins équivalente à celle de 2022 soit reconduite en 2023, il s'agit d'une demande Hamid a minima, puisqu'avec 15 millions d'euros, le Fath that est censée couvrir les 1500 du territoire national, or il ne représentent que 10000 euros par structure, ce qui ne permettra pas de répondre aux besoins. Merci le 553 monsieur Madame la présidente, madame le Ministre, mes chers collègues, le Conseil économique et social et environnemental, rappelait dans un rapport récent acidulé, la place des jeunes dans les territoires ruraux que malgré des résultats supérieurs à la moyenne nationale au Baccalauréat, la proportion des jeunes qui poursuivait des études supérieures était 2 fois moindre que les jeunes vivant en milieu urbain, notamment à cause de l'assure, mais également à cause d'éloignement des centres d'enseignement supérieur, en outre, le taux des jeunes de 18 24 ans ne poursuivant ni études ni formation et était de 4, plus élevé que la moyenne nationale. Ces constats appellent à ne plus dissocier le développement des territoires et l'accompagnement des jeunes dans la préparation de leur avenir et de l'avenir de de ces territoires, aussi proposer une action nouvelle qui est celle de généraliser au niveau national, expérimentation menée par l'association Bocage en région Centre, intitulé Les jeunes s'en mêle et financé grâce au pays, ce dispositif, pardon, consiste en la mise en place d'un maillage fin de référent jeune capable d'aller à rencontre des jeunes et de les accompagner dans leurs projets universitaires mais mais aussi associative de repérer ceux qui sont en difficulté qui seraient piloté en quelque sorte par des structures neutre où siégeraient divers acteurs de de la société locale, chef d'entreprise me l'emploi, et il est proposé de mettre en ce dispositif de l'élargir à titre expérimental dans 2 régions où se trouve une population de jeunes inférieurs à la moyenne nationale et c'est la raison pour laquelle il propose une enveloppe de 13 millions d'euros, je vous remercie. Merci l'amendement 554 madame Liban. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre le présent amendement a pour objet de permettre à l'accompagnement, dès 2023 du développement de 10 résidences de répit partagé à titre de mesure nouvelles financé à hauteur de 10 millions d'euros, soit un 1000000 d'euros par structure de 60 places médico-social d'hébergement temporaire 30 places étant consacré à l'accueil des personnes en situation de handicap et 30 à celle des des personnes âgées en perte d'autonomie accompagné d'au moins, au moins, d'au moins autant des dents au titre de la branche autonomie gérée par la CNSA une résidence Rebbie partager propose l'accueil temporaire à vocation médico-social de la personne aidée en présence d'un ou plusieurs aidants familiaux bénéficiant conjointement d'une offre de tourisme et vacances adaptées à leurs attentes et besoins réciproques, bien que la stratégie nationale 2020, 2022, agir pour les aidants, effet de ce dispositif, une priorité sa mesure 12 de renforcement et diversification des solutions de répit il est constaté l'absence de développement réel de ces solutions pourtant fortement attendue par l'ensemble des parties prenantes dont au 1er chef les associations des dents, prenant acte de ce Plfss 2023, le conseil de la CNSA une même attente alertant sur le manque de mesures en direction des aidants et de leurs proches, et en particulier la possibilité pour eux de bénéficier de solutions de répit, plus d'une dizaine de territoire et au 1er chef leurs conseils départementaux, toujours en lien avec les associations représentatives des personnes et des aidants sont porteurs de ces projets novateurs de résidence de répit partagé, Docteur, Madame la Ministre, ce qui vous est au moins aussi cher qu'à moi, celui des Landes aussi par cet amendement, nous vous proposons la création au sein de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, d'un nouveau programme Fonds d'appui territoriale, au développement des résidences de répit partager composée d'une action unique abonder des crédits de l'action de 13 du programme 304 inclusion sociale et protection des personnes, à hauteur de 4 millions d'euros en a eu en CP, des crédits de l'action de 13 du programme 150 et nous vous demandons de lever le gage. Si cher collègue, c'est parfait, amendement 509 madame la présidente, Guillon. Madame a président le bilan 500 599 oui. J'ai eu un doute, j'ai entendu ça non, non, voilà ça 90, merci madame la présidente, mes chers collègues, en 2021, le gouvernement a lancé un plan interministériel pour mieux lutter contre la prostitution des mineurs qui concerne entre 7 et 10000 jeunes en France suite à un travail d'ailleurs fouillé que la procureure Champ-Renault avait mené et que nous avions auditionnées au sein de la délégation aux droits des femmes, ce phénomène de prostitution de mineure présents sur tout le territoire, touche surtout des jeunes filles âgées de 15 à 17 ans, avec un point d'entrée dans la prostitution, de plus en plus tôt, se situant entre 14 et 15 ans pour plus de la moitié d'entre elles, le plan qui a été déployé sur les années 2021 2022 vise à sensibiliser et à informer les mineurs à renforcer les repérages des jeunes impliqués accompagner ceux en situation prostitutionnel, ainsi qu'à renforcer l'action judiciaire contre les clients et les proxénètes, des actions doivent être déployés au cours des de l'année 2023, hélas, hélas, pardon, le projet de loi de finances ne prévoit pas de moyens financiers fléché spécifiquement sur la lutte contre la prostitution des mineurs, les moyens financiers employé pour l'année 2022 était issu d'un report de crédits non consommés en 2021, le plan ayant été tardif monter le poulailler au cours de sa première année cependant, ces crédits doivent être doivent à présent être renouvelée et garanti pour 2023, comme je vous le disais, ce sont 7-t-il Bill mineurs qui se trouve en danger tant physiquement que psychologiquement, c'est pour cela que je vous invite à voter cet amendement qui vise à s'assurer que ce plan de lutte contre la prostitution des mineurs dont l'importance ne peut être ignorée, hé bien doté de crédits nécessaires à son bon déploiement pour l'année à venir, je vous remercie. Merci l'amendement 550 Madame Le Houerou. le taux de non-recours aux aides sociales et minima sociaux est estimée à environ un tiers des potentiels bénéficiaires, c'est autant de personnes en situation de grande précarité qui ne peuvent disposer de leurs droits, d'après Helena Réville, chercheuse à l'université de Grenoble c'est non recours sont expliquées par la complexité du chemin pour demander des aides, c'est un parcours du combattant, il faut d'abord s'adresser aux caisses d'assurance maladie, constituer un dossier puis se tourner vers des organismes complémentaires et à chaque étape il y a des incompréhensions qui font que le dossier ne va pas au bout, ainsi, si nous avons pu réaliser le prélèvement à la source pour les impôts, nous pensons qu'il est nécessaire d'engager une automatisation et de la réaliser pour le versement du RSA. Merci l'amendement 711 madame Gréaume. Merci par cet amendement d'appel, nous proposons d'investir pour généraliser les contrats jeunes majeurs au majeurs qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance, dont la plupart sont en très grande difficulté, les départements ont réduit ces dernières années, la durée, le montant des contrats jeunes majeurs, vu les crédits insuffisants et les baisses de dotations, les départements ont besoin de l'État pour les soutenir dans cette action en effet environ 36 % des ex de l'ASE bénéficient d'un contrat jeune majeur de durée variable et montants différents face à ces inégalités, nous estimons qu'il revient à l'État de garantir un statut social pour tous les jeunes majeurs de 18 à 21 ans et à assurer la généralisation des contrats jeunes majeurs à l'ensemble des majeurs de l'aide sociale à l'enfance telle et le sens de cet amendement d'appel merci. Merci l'amendement 712 madame hein pour ce. Merci madame la présidente, cet amendement d'appel visent donc à étendre le RSA aux jeunes de moins de 25 ans, d'après la dernière étude de l'Observatoire des inégalités, la moitié des plus pauvres au moins 30 ans le taux de chômage atteint, parmi eux, eux, selon le président des Restos du Coeur, la moitié des bénéficiaires à moins de 25 ans, un sentiment que partage la Fondation Abbé Pierre et le Secours catholique, mais également les associations étudiantes vivre avec 580 euros par mois, ce n'est pas un idéal pour personne et ceci à n'importe quel âge il faudrait évidemment aller plus loin avec un véritable statut social pour l'ensemble des jeunes lors de la pandémie de Covid 19 l'ancien 1er ministre Jean Castex, occupé par la gestion des retards de métro et de manque de conducteurs de bus avaient refusé de m'y mettre en oeuvre cette proposition une tribune publiée dans le JDD, demandant l'extension du RSA pour les 18 25 ans avait pourtant été signé par plusieurs associations, dont la Fondation Abbé Pierre, les apprentis d'Auteuil, la Fédération des associations générales et l'Union nationale des étudiants de France, aujourd'hui il est encore possible de ne pas sacrifier les jeunes qui sont l'avenir de notre pays aussi assurons leur un revenu minimum pour lutter contre la précarité, telle est donc le sens de notre amendement, je vous remercie. Merci l'amendement 329 de la commission des affaires sociales présenté par monsieur le rapporteur Jean Sol. créé par la loi du 7 février 2022 relatives à la protection des enfants, résulte du gros groupement du GIP Enfance en danger Giped de l'Agence française de l'adoption du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et du conseil national de la protection de l'enfance à compter du 1er janvier 2023 le nouveau Jeep exercera au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de la politique publique de protection de la, de l'enfance d'adoption nationale et internationale et d'accès aux origines personnelles, il contribuera à l'animation à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire, la loi prévoit que le Giped de financé à parts égales par l'État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive, répondant à une demande et des départements, l'article 46 quater du PLF inséré à l'Assemblée nationale permet cependant à titre dérogatoire que la part de l'État dans ce financement soit supérieure à celle des départements en 2023 toutefois le coût supplémentaire qui devrait en résulter pour l'état n'a pas été répercutée dans les crédits de la mission afin que le report de la montée en charge de la contribution des départements ne compromettent pas la capacité du GIP à exercer ses missions cet amendement de la commission des affaires sociales vise à abonder de un virgule 4 millions d'euros les crédits dédiés à leur financement. l'aide financière à l'insertion sociale, à la sortie de la prostitution à hauteur du RSA en effet au 1er rang des violences faites aux femmes, nous comptons la prostitution depuis l'adoption de la loi de dix de de 2016, les moyens financiers dégagés pour faire vivre l'ambition abolitionniste de la France ne sont pas au rendez-vous et cela se ressent sur le terrain, on propose par cet amendement, de faire passer le montant de la FIS à hauteur du RSA, quoi de plus normal pour des femmes déjà très fortement précarisé dans mon département en Loire-Atlantique, l'accompagnement vers le parcours de sortie de prostitution est assurée par le mouvement, le nid, il emploie une travailleuse sociale pour accompagner les personnes en en situation de prostitution vers la sortie, ce salaire coûte 44000 euros par an et le ni perçoit une subvention entre 20 et 22000 euros de l'État, on voit vite l'insuffisance de la situation pour l'association, qui s'interroge sur le renouvellement de son agrément, alors même que les sorties de de parcours fallait les les parcours réussi de sortie de prostitution sont nombreux les moyens mérite d'être développé s'agissant du montant de la FIS pour les personnes en situation de prostitution, comme pour les associations qui accompagnent les femmes. Merci l'amendement 714 même Cohen. Oui, cet amendement d'appel vise à augmenter de 500000 euros, le financement des associations qui accompagnent les personnes sortant de la prostitution et l'aide financière à l'insertion professionnelle, merci aux personnes s'engageant dans un parcours de sortie de la prostitution en effet la mission Solidarité prévoit une très légère augmentation de l'enveloppe allouée à l'aide financière pour l'insertion sociale, destiné aux personnes en parcours de sortie de prostitution de plus 0,3 % alors que le nombre de bénéficiaires a triplé entre 2018 et 2021, le montant de la FIS qui est, je le rappelle, de 363 euros reste très faible et insuffisamment incitatif, comme le note le rapport spécial du Sénat de nos collègues, Arnaud Bazin et Éric Bocquet notre amendement propose donc d'augmenter les crédits destinés à la prévention, à la lutte contre les violences et la prostitution de 500000 euros afin d'adresser un signal, y compris aux victimes de ce système prostitutionnel qui est mortifère, j'en profite pour demander la pleine application de la loi du 13 avril 2016 renforçant la lutte contre le système prostitutionnel et la compagnons des personnes prostituées afin de donner des moyens à la hauteur des besoins aux commissions départementales chargées de mettre en place les parcours de sortie de la prostitution, la situation est inacceptable au regard de l'enjeu prioritaire que représente la lutte contre la prostitution et la marchandisation des corps telle et le sens de cet amendement d'appel, je vous remercie. Merci l'amendement 668 madame Vogel. ou résidences sociales en France, ce dispositif permet de sécuriser leurs droits sociaux lorsqu'ils effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine, plus de 6 mois, c'est-à-dire de continuer à percevoir une prestation comparable au minimum vieillesse, ce qui est impossible avec l'ASPA qui elle suppose de résider en France sous prétexte que le recours à cette aide est en baisse, le gouvernement fait dans ce budget, le choix de baisser les crédits alloués pour notre part, nous considérons au contraire qu'il est nécessaire de maintenir les moyens budgétaires alloués l'an dernier et invitant le gouvernement a plutôt lutter contre les non-recours évidemment l'objectif n'est pas de réduire le budget de l'action 17 du programme 124 hein, c'est simplement pour respecter l'article 40 de la constitution, que nous avons construit la maman comme ça et l'objectif c'est bien d'alerter le gouvernement sur le besoin de maintenir les crédits dont il est question, identiques à ceux votés en 2022, je vous remercie. Merci l'amendement 542 Madame Le Houerou. Il concerne donc également les le budget pour accompagner les femmes victimes de violences dans son rapport de 2020 intitulé où est l'argent pour mieux protéger les femmes victimes de violences, examinant donc les moyens dont dispose la politique publique afférentes, la Fondation des femmes propose la création d'un observatoire national des féminicides cet amendement ajoute donc au budget consacré à l'égalité entre les femmes et les hommes 500000 euros, dans le but de créer cet observatoire et de lui permettent de fonctionner immédiatement la mise en application de cette proposition nous paraît indispensable, d'abord parce que, aujourd'hui, le décompte des meurtres conjugaux réalisé et réalisé par le collectif Féminicides Par compagnon qui a permis de mettre en lumière la réalité dramatique et implacable des féminicides commis sur notre territoire, cette mise en lumière à participer à une mobilisation exceptionnelle de la société en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et autour des familles de victimes, ensuite, comme l'ont révélé les investigations du monde une part significative des féminicides aurait pu être évité en 3ème lieu donc il s'agit également de prévoir une structure capable de répertorier mais également d'analyser les meurtres des femmes en raison de leur sexe permet de répondre partiellement aux conséquences de la disparition de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales l'année dernière, ensuite, nous devons également à la mémoire de trop nombreuses victimes l'engagement ferme et entier de toute la société dans un seul but éradiquer les violences faites aux femmes, la proposition est donc de créer cet observatoire et qui s'insèrent pleinement dans les une réponse donc aux objectifs que je viens de citer. Merci l'amendement 500 même de Marco. Merci madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, alors que 19 % des jeunes de 15 à 24 ans sont au chômage et que 20 % des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté, il n'existe aucun filet de sécurité pour les moins de 25 ans ainsi près de 800000 jeunes de bénéficier d'aucune couverture minimale, cet amendement vise à étendre l'accès au Revenu de solidarité active aux jeunes de 18 à 25 ans, ce revenu étant le dernier filet de sécurité de notre pays en matière de protection sociale, les jeunes de 18 à 25 ans peuvent voter ce salarié payé des cotisations et des impôts mais ils ne peuvent pas accéder au RSA un plan, un jeune une solution lancé par le gouvernement n'est pas à la hauteur de nombreux jeunes se retrouvent sans emploi ni formation et surtout sans aucun revenu des contrats précaires ne sont pas la solution, l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans permettra d'accompagner notre jeunesse dans sa formation et son insertion professionnelle pour conclure, mes chers collègues, lutter contre la précarité de notre jeunesse, ce n'est pas de l'assistanat, c'est investir pour l'avenir. Merci madame la présidente, mai 2022 indique à partir de l'enquête Santé européennes de 2019 que de 5 millions de Français demeurent sans complémentaire santé, les personnes les plus pauvres sont toujours les plus concernés par l'absence de complémentaire santé, selon l'article précité, la situation économique et sociale des individus reste le principal déterminant de la souscription d'une complémentaire santé et surtout du niveau de garantie souscrit les familles monoparentales, les personnes en dehors du marché de l'emploi, les retraités les plus pauvres sont particulièrement impacté parmi les causes de l'absence de complémentaire santé, on compte un tiers de non-recours aux droits de la CSS, notamment en raison de difficultés administratives, la CSS en mutualisant les anciens dispositifs de la CMU-C et de l'ACS avait pourtant pour objectif 1er de faciliter l'accès des bénéficiaires potentiels cet amendement se propose d'accentuer les efforts déployés afin de lutter contre le non-recours à la complémentaire santé solidaire dans une logique de prévention et d'aller vers les populations les plus fragilisées à titre d'exemple, le programme que cet amendement vise à créer, pourrait permettre d'automatiser la filiation à là c'est et de financer de vastes opérations de phoning auprès des personnes éligibles, il s'agit ici d'un amendement d'appel d'une d'une somme de d'un Euro symbolique mais qui permet de créer une mission dédiée à lutter enfin contre le non-recours à la complémentaire santé solidaire. Merci l'amendement 574 madame pour ces Mondiaux. Merci madame la présidente, donc par cet amendement d'appel, nous demandons la mise en place d'un véritable plan d'éradication du sens prisme qui était d'ailleurs une promesse de du de dès la première année de son mandat, le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal logement en 2022 indique que le nombre de sans-domicile-fixe élèverait au moins en France à 300000 personnes d'après un rapport d'information fait au nom de la commission des finances du Sinn du Sénat sur la politique d'hébergement d'urgence, la crise sanitaire a accentué les limites déjà existantes de la politique d'hébergement, l'année 2020 ayant mobilisé le secteur de l'hébergement d'urgence à un niveau inédit, s'il n'y a aucun chiffre officiel sur le nombre de sans-papiers parmi les structures d'hébergement d'urgence, plusieurs acteurs du secteur, estime qu'ils constituent un public majoritaire afin de combattre l'embolie du système d'hébergement d'urgence, le directeur de l'Office français de l'Immigration et de l'intégration, Didier, défend le fait de faciliter la régularisation des familles qui stagne depuis de nombreuses années dans l'hébergement d'urgence, c'est une forte mobilisation des élus locaux a permis de convaincre le gouvernement de renoncer à la fermeture de 14000 places d'ici l'année prochaine, permettant du de ce fait, de stabiliser le parc d'hébergement à à hauteur de 197000 places, cela n'est pas suffisant, cet amendement nécessiterait l'abondement de sommes considérables pour un programme dédié aux sans-abrisme et conviendrait non seulement de créer des places d'hébergement mais aussi et surtout de libérer des places par des sorties plus rapide, vers le logement donc cet amendement invite à amorcer un plan pluriannuel de grande ampleur. Merci l'amendement 667 même mange. Alors, cet amendement est un amendement d'appel pour demander au gouvernement de publier le rapport sur le revenu universel d'activité, je voudrais d'abord rappeler la jeunesse de ce rapport fin 2018 Emmanuel Macron lançait en grande pompe la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté depuis là, 10 stratégie s'est réduit à la à la principale mesure qui a consisté à distribuer des petits déjeuners à l'école, c'est important, je n'en disconviens pas, mais ça n'éradique pas la pauvreté pour les enfants, je rappelle un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté en France, alors en 2019 le président annonçait la fusion des minima sociaux, on a revenu universel d'activité, un projet qui, selon l'exécutif devait répondre au problème de la pauvreté, mais qui n'a à ce stade, toujours pas abouti et n'a en réalité que braquer contre lui les principaux acteurs de lutte contre l'exclusion face à ce projet, constatant son incapacité à formuler des réponses utiles et partager pour lutter contre la pauvreté et d'exclusion, la dernière initiative du gouvernement fut de missionner l'adresse pour rédiger un rapport sur le revenu universel d'activité qui, bien que remis en mains propres au 1er Ministre de l'époque n'a jamais été rendu public par le gouvernement, franchement qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut justifier que sur une question si fondamentale pour l'organisation sociale de notre société, un rapport remis au Premier Ministre soit gardé confidentielles, y compris pour le Parlement, attaché au débat et à la confrontation des idées, nous demandons simplement qu'il soit publié la haute administration, a produit un travail, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que si, qu'on soit d'accord ou non avec le projet que l'on partage ou non le contenu du rapport lui-même, il en va de la transparence et de la bonne santé démocratique que les rapports demandés en plus remis soit soit publié pour éclairer les décideurs, les décideurs publics et et paraît que par excellence, le Parlement. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Bien, merci, madame la présidente, nous allons alternativement à mes collègues : Arnaud Bazin présenter les avis donc avec votre permission de le président je donnerai la vie sur les 3 premiers 422 puis 423 et 24 qui sont des amendements de repli portant sur le même objet, merci madame, alors le 422 qui porte sur la politique d'accompagnement du deuil, le présent amendement vise à ouvrir à un montant de 522 millions d'euros pour la politique d'accompagnement du deuil, bien qu'il s'agisse d'un problème grave, bien évidemment, cette politique publique ne s'inscrit que difficilement dans le Champ de la mission et des administrations chargées de la mise en oeuvre de ces différents programmes, elle nous semble davantage relever de de l'assurance maladie, voilà pour le 422 le 423 donc même objet, mais cette fois-ci, le montant proposé à 160 millions d'euros et le 424 8 sur un montant de 200 millions d'euros, donc : demande de retrait sur ces trois amendements. Merci. Merci madame la présidente, madame le Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je prends maintenant le 534 qui vise à renforcer 250 millions d'euros, les crédits de la stratégie pauvreté la baisse constatée en 2023 est soulignée par les auteurs de l'amendement, tient au fait qu'en 2023, c'est une année de transition avec la fin des contrats État département dans l'attente de la conclusion d'une nouvelle génération de contrat, nous avions critiqué dans nos travaux de contrôle, cette forme d'impréparation et la nécessité de proroger par 2 fois, les contrats en cours, il aurait été préférable d'anticiper davantage pour lancer la nouvelle génération dès cette année pour le reste, cet amendement dont la finalité n'est pas précise en dehors du constat d'un manque de moyens, doit, selon nous, être considéré comme un amendement d'appel, c'est pourquoi nous en demandons le retrait. Je prends ensuite le 533. Qui vise à renforcer de 125 millions d'euros, les crédits de la stratégie pauvreté bon même chose se aux yeux un amendement drape d'appel avec une demande de retrait. Trente-cinq avec la création d'un fonds de prévention de l'inceste, de 100 millions d'euros, nous observons que la prévention de l'inceste et d'ores et déjà dans ce, dans un des axes de la stratégie de la protection de l'enfance, dont les crédits ont déjà progressé de 70 millions d'euros au PLF c'est donc aussi une demande de retrait le 538 création d'une cellule nationale de conseil et de soutien pour les professionnels, destinataire de révélations de violences sexuelles de la part d'enfants et doté 10 millions d'euros. ces crédits ont été des crédits ont déjà été ajoutés pour permettre un tel soutien à hauteur d'un 1000000 et demi d'euros, nous proposons de d'attendre pour voir si des moyens supplémentaires sont vraiment nécessaires pour les renforcer, le cas échéant l'an prochain, c'est également une demande de retrait sur le 539 vise le fond, le financement d'un fonds de repérage systématique des violences sexuelles auprès de tous les enfants, par tous les professionnels et qui serait doté de 5 millions d'euros, cette lutte contre les violences sexuelles, je viens de le rappeler, fait déjà l'objet d'un des axes stratégiques de protection de l'enfance, donc les crédits ont progressé de 70 millions d'euros, c'est également une demande de retrait.

Alors pour le 385 de notre collègue Chassaing, donc le présent amendement vise à renforcer de 95 millions d'euros, les moyens de la politique de protection juridique des majeurs, certes le PLF intègre la budgétisation à hauteur de 40 millions d'euros en année pleine d'une revalorisation des mandataires dans le cadre du Ségur et les crédits de cette action atteignent 800 millions d'euros, plus 70 millions les auteurs de l'amendement font valoir que le nombre de mandataires est insuffisant pour permettre une prise en charge des mesures de protection dont la dynamique est très importante dans des conditions satisfaisantes, ce constat est corroborée par les auditions que nous avons pu conduire lors de nos travaux, ces ces dernières années, nous souhaitons ainsi demandé l'avis du gouvernement afin de savoir quels moyens pour être dégagée pour remédier à ce problème structurel.

voilà le présent d'amendement vise à renforcer donc de 95 millions d'euros, les moyens de la politique de protection juridique des majeurs, certes le PLF intègre la à la hauteur de 40 millions d'euros en année pleine, tout cela a déjà été dit donc là aussi nous demandons l'avis du gouvernement pour connaître les moyens décidé pour remédier à ce problème structurel. Voilà, idem pour le soixante même de monde donc avis du Gouvernement sur l'amendement 60 présentée par notre collègue. Le 537 vise à ouvrir 20 millions d'euros pour le financement d'un fonds de soutien pour les initiatives de solidarité alimentaire territorialisée, l'amendement est satisfait, puisque le projet de loi de finances prévoit déjà 60 millions d'euros supplémentaires pour financer un nouveau fonds pour les nouvelles solidarités alimentaire dont la gestion serait déconcentré, nous considérons comme notre part et et j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure à la tribune qu'il serait préférable d'utiliser ces crédits nouveaux pour financer directement les associations qui sont considérablement fragilisé par la crise énergétique et par la problématique de l'eau infructueux et également de l'inflation sur tous les produits alimentaires certes prévoir de la qualité des circuits courts, peut être un chèque alimentaire tout ça pourrait être débattue mais aujourd'hui, l'urgence de l'urgence et que les associations puissent continuer à tourner dans le modèle français français associatif et ce, ce à quoi nous vous engageons donc ce sera une demande de retrait. Sur le 549 et c'est un amendement d'appel qui vise à revaloriser les personnels du programme 137, celui-ci ne finançons pas de dépenses de personnel, il vise en réalité les opérateurs financé par le programme s'agissant de revalorisation salariale de structures associatives, privées qui ne sont donc pas décidé par l'État, il ne semble pas qu'une augmentation des crédits soit opérante faudrait au sein des associations pour en appliquer la revalorisation con parce que l'accomplissement des missions convention avec l'État, ce qui pourrait être source de complexité, voire d'inéquité entre salariés, il convient également de noter qu'un tel amendement représenterait à lui seul près de la moitié des crédits du programme qui ont déjà connu une progression importante ces dernières années, 15 % de plus en PLF 2023, c'est donc une demande de retrait, mais mon collègue à titre personnel, lui, est favori, le 594 revalorisation de 16 millions d'euros pour les métiers, financé par le programme égalité entre les femmes et les hommes identiques identique même mêmes observations demande de retrait

Voilà pour le 509 donc, cet amendement prévoit de reconduire les financements octroyés pour la modernisation des établissements et services d'aide par le travail, les ESAT dans le cadre du plan de relance du fait de la fin du plan de relance, il n'existe en effet plus de crédits dédiés dans le présent PLF toutefois la mise en oeuvre des projets retenus se poursuivra en revanche en 2023, cet amendement est l'occasion d'interroger le gouvernement sur le bilan du Fatah that l'opportunité de reconduire un tel font en 2023, comme cela était prévu sur la mission Travail et emploi s'agissant du fond de transformation des entreprises adaptées, nous demandons donc l'avis du gouvernement, sur cet amendement. 509 ensuite. 41541 voilà est identique, donc, même chose à avis du gouvernement, ensuite on a de 553 qui est un peu différent donc déploiement de référent jeunesse en zone rurale, cet amendement propose de financer le déploiement à titre expérimental, durant 5 ans, dans 2 régions où la part des jeunes et moins importante au sein de la population totale du département de procéder au déploiement de référent jeunesse si l'idée est intéressante, elle fait écho à d'autres dispositifs financés par la mission enseignement scolaire notamment les cordées de la réussite en outre les référents jeunesse reste à définir l'amendement nous semble donc relever d'un appel au ministre qui pourra développer sur les politiques déjà en cours, donc c'est une demande de retrait. Merci. pour 12 millions d'euros destinés au développement territorial de solutions temporaires de répit, partagé entre les aidants et leurs proches en situation de handicap, maladie chronique ou perte d'autonomie liée à l'âge. Il nous semble que l'État doit participer aux côtés des départements à un soutien renforcé aux aidants, dont le l'appui essentiel et précieux et qui sont trop souvent laissés pour compte, c'est donc un avis favorable de la commission des finances qui prévoit de renforcer, à hauteur de 7 millions d'euros les moyens du plan interministériel, doté de 14 millions d'euros pour lutter contre la prostitution des mineurs, les moyens de ce plan nous paraissent relever davantage de la direction de protéines de la protection judiciaire de la jeunesse et donc du ministère de la justice, plutôt que de la mission que nous examinons néanmoins cet amendement à l'occasion d'interroger le gouvernement pour faire le point sur la mise en oeuvre du plan, son éventuelle articulation avec la stratégie, protection de l'enfance en partie porté par la mission, elle est sur la nécessité de renforcer ses moyens je sollicite donc l'avis du gouvernement le 550 qui porte sur le versement automatique du RSA mais qui est dotée de 5 millions d'euros est à nos yeux un amendement d'appel qui est l'occasion de l'interroger le gouvernement sur la traduction concrète de la promesse de solidarité à la source, mais sinon, c'est une demande de retrait. Merci. Le 711 le présent amendement propose ouvrir 5 millions d'euros au titre de la généralisation du dispositif de contrat jeune majeur visant à accompagner les jeunes sortant de l'âge, il nous semble que ce type de dispositif en lien avec les compétences départementales doit faire l'objet d'une approche différenciée selon les territoires, plutôt que d'un dispositif uniforme piloté par l'État, la prévention des sorties, c'est je l'âge a constitué l'un des principaux axes des contrats État département dans le cadre de la stratégie, pauvreté et doivent le rester pour la prochaine génération de contrat, donc c'est une demande de retrait pour la commission, à titre personnel favorable cet amendement vise à ouvrir le débat sur l'extension du RSA aux personnes âgées de moins de 25 ans, au vu du montant demandé 5 millions d'euros, il ne peut s'agir que d'un amendement d'appel, une telle mesure elle avant tout et cas en tout état de cause, pardon, de la loi demande de retrait, sauf à titre personnel, c'est la schizophrénie et le 329 présentée par notre collègue sol cet amendement vise à de 1 virgule 4 millions d'euros, la contribution de l'État au financement du nouveau Jeep France Enfance protégée : en effet, comme le souligne le rapporteur pour avis les conséquences budgétaires de l'article 46 quater inséré dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale n'ont pas été tirés sur les crédits de la mission pour mémoire cet article permet de déroger au principe de financement paritaire entre l'État et les départements en 2023, d'où il résulte nécessairement un relèvement de la contribution de l'État, ce sera un avis favorable. Merci.

le montant de la FIS nous paraît donc insuffisante pour vivre décemment, comme l'a souligné d'ailleurs récemment un rapport de l'IGAS sus-cité par les auteurs, ils incitent les auteurs à accepter des emplois très peu qualifiés, pour trouver un complément de revenu au détriment du succès de leur parcours de formation, la lutte contre la prostitution étant un enjeu de pub public de politique publique majeure son portage est insuffisant, il faut renforcer le montant de la de la FIS c'est aussi contribuer à inciter davantage de victimes à s'orienter vers un parcours de sortie de prostitution, nous ne voyons pas pourquoi l'État ne compte qu'on ne consacrerait pas pour le financement des prestations dont il a la charge, un effort au moins similaire à celui qu'il impose aux départements pour les personnes en voie d'insertion pour toutes ces raisons, nous donnant un avis favorable à cet amendement. Le 714 c'est aussi hein n'amendements qui porte sur les moyens de lutte contre la prostitution, avec un budget renforcé de 500000 euros, comme c'est un amendement d'appel, c'est l'occasion d'ouvrir le débat, c'est une demande de retrait le 668 augmentation des crédits destinés au financement de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans les pays d'origine, l'avait fait la FS, pardon, il nous semble que cet amendement n'est pas opérants, car FS est un droit ouvert dont les conditions d'attribution sont déterminés par l'article L 117 3 du code de l'action sociale et des familles, le montant inscrit au présent PNF n'est donc qu'une prévision, c'est donc une demande de retrait. Merci pour 542. Sur l'amendement 542 le président maman vise à ouvrir 500000 euros de crédits supplémentaires pour le financement d'un observatoire national des féminicides si la cause est de première importance, la mission interministérielle pour la protection des femmes, le Miprof du ministère de l'Intérieur publie déjà des études sur le sujet, hein, si on sait qu'en 2021 122 femmes ont été tuées par leur ex-compagnon en compagnon, il ne nous paraît pas eux, donc utile, efficace de multiplier les structures, l'amendement nous semblent satisfaits : demande de retrait pour le 500, cet amendement vise à ouvrir le débat sur l'extension du RSA aux personnes âgées de moins de 25 ans, au vu du montant demandé donc un euro il ne peut s'agir que d'un amendement d'appel, une telle mesure relève en tout état de cause, la loi donc demande de retrait favorable à titre personnel et pour le 573 amendement qui vise à ouvrir le débat sur le non-recours à la complémentaire santé solidaire aux personnes âgées de moins de 25 ans, là aussi au vu le montant demandé un Euro, il ne peut se dire que, d'un amendement d'appel, une telle mesure relève en tout état de cause, avantages du PLFSS selon nous demande de retrait. Merci 574. Oui, c'est un amendement qui voudrait obtenir l'éradication du sans-abrisme mais il est inscrit un montant d'un euros, il s'agit là aussi d'un amendement d'appel, une telle mesure relève en tout état de cause, davantage de la politique du logement, que de la mission ou de la mission cohésion des territoires que de notre mission, c'est donc une demande de retrait. Le 667 demande une publication d'un rapport sur le revenu universel d'activité, donc il vise manifestement à ouvrir le débat sur cette question, vu le montant inscrit également c'est un amendement d'appel mais le projet de semble avoir été abandonnée au profit du projet de solidarité à la source, donc je renouvelle le questionnement au gouvernement sur ce sujet. Merci beaucoup, alors l'avis du gouvernement, je ne sais pas qui prend la parole en 1er, monsieur le Ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, donc on va se succéder pour répondre aux pour donner l'avis du gouvernement sur les différents amendements, je vais essayer d'être le plus clair possible mais je vais répondre immédiatement pour les amendements 422 423 424 sur la question de l'accompagnement du deuil qui évidemment un sujet de préoccupation pour le gouvernement qui oeuvrent constamment à améliorer cet accompagnement, c'est notamment pour cette c'est notamment pour cela que nous avons mis en place un congé pour deuil parentale pour accompagner la douleur des des parents qui vivent le drame de la perte d'un enfant, par ailleurs, l'accompagnement des personnes endeuillées doit être fait, bien en amont du décès et c'est pour cela que l'accompagnement des aidants, des personnes en fin de vie est un axe important du plan en cours de développement des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie et en second lieu concernant les professionnels confrontés à l'accompagnement des personnes en deuil. Différentes formations existent déjà dans le cadre de la formation continue donc compte tenu ces événements, nous suivons l'avis de la des rapporteurs : avis négatif concernant l'amendement numéro 533

534. Oui, Monsieur le Ministre, à vous pouvez faire tous vos amendements à vous, oui, à condition de les prendre tous dans l'ordre comme ça et puis donc la ministre se rendra après OK, c'est ce qui est en train de ça. Excusez-moi, madame la présidente, alors concernant le 533 sur l'abondement des crédits, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la la pauvreté, la première ministre, il a annoncé le 3 novembre dernier à cette stratégie de lutte contre la pauvreté va succéder un un pacte national des solidarités qui va s'appuyer sur le le le la stratégie précédente et son n'évaluation il comportera 4 axes : les 2 premiers sont ceux qui étaient, qui ont bien fonctionné dans la stratégie précédente, à savoir la lutte contre les inégalités de destin et la reproduction sociale, de la pauvreté, le second c'est l'insertion par l'emploi, le troisième qui me tient particulièrement à coeur et vous le comprendrez, c'est celui contre la de la lutte contre la grande exclusion et enfin de faire de cette transition écologique une transition solidaires et donc de travailler en profondeur sur la question de la réduction pour les foyers modestes des charges contraintes que représente l'alimentation, l'axe alimentation l'hébergement et la mobilité. En attendant la mise en place de ce pacte de solidarité qui interviendra à partir de 2024 et donc nous recontre actuel Liseron avec les collectivités en 2023 l'année 2023 sera donc une année de transition, c'est pour cela que facialement les crédits, les crédits baissent parce qu'en fait l'idée c'est de remettre en cohérence les calendriers des différentes contractualisation certaines collectivités devront donc contractualisé en 2023 pour 6 mois pour accompagner ces départements donc, dont les crédits vont baisser sur l'année 2023, on a mis en place une enveloppe complémentaire, notamment pour renforcer les crédits à l'insertion et au total, ces contrats de lutte contre la pauvreté représenteront 94 % de ce effectivement contractualisé en 2021, donc la baisse n'est pas celle que vous mentionnez donc pour ces raisons je suis défavorable à votre amendement concernant les amendements 385 416 et 658 l'augmentation des crédits, la protection juridique des majeurs, je pense qu'on poursuit avec ce projet de loi de finances pour 2023 le même objectif, celui d'améliorer la qualité de la prise en charge des personnes protégées, l'un des moyens, en effet, consiste à diminuer le nombre de personnes prises en charge par mandataire judiciaire, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a augmenté le budget de 7 virgule 1 millions d'euros pour 2023, afin notamment de prévoir l'embauche de 200 mandataire supplémentaires, cette mesure a un caractère progressif, compte tenu des délais nécessaires pour la formation et le recrutement de ces nouveaux mandataires des métiers qui ne font pas exception dans le Champ, dont j'ai la responsabilité en terme d'attractivité, c'est en 2023 qu'elle connaîtra donc son plein effet, il nous semble indispensable d'évaluer l'effet des nouveaux recrutements avant d'aller plus loin, par ailleurs, les métiers du secteur social au sens large, connaissent une véritable crise d'attractivité, je viens de le dire qu'qui ne n'épargne pas la protection juridique et il nous semble nécessaire d'aborder cette question de façon plus globale, plusieurs travaux en cours doivent permet de structurer en profondeur le secteur de la protection judiciaire des majeurs, avec en particulier la la refonte de la formation initiale des mandataires avec l'instauration d'une filière dédiée univers cet universitaire Izé autour d'une licence professionnelle, mais également l'intégration de la protection judiciaire majeur dans la politique d'accompagnement global des personnes vulnérables pour toutes ces raisons, nous donnons un avis défavorable à l'ensemble de ces amendements concernant ensuite. Juste de monsieur, oui monsieur mise je, je rappelle que nous sommes dans un temps contraint et que, si vous voulez revenir samedi ou dimanche, moi je suis prévu pour présider dimanche soir donc, pas de souci, il faut peut être juste un tout petit peu raccourcir, voilà les explications, c'est 48 peut être pas favorable ou défavorable, ça besoin quand même de réponse mais peut être quelque chose d'un peu plus court, merci. OK, OK, je, je vais donc accélérer 537 sur le fonds de soutien aux initiatives de solidarité de citoyenneté alimentaire, les rapporteurs, l'ont dit, on a mis en place et la première ministre, il a annoncé un fonds de 60 millions d'euros dédié dédié à cette question, votre amendement et est satisfait. Vous m'interrogez sur la façon dont nous allons dépenser cet argent préalablement, je rappelle que les crédits au total pour l'aide alimentaire pour 2022 ont été triplé entre les 2 projets de loi de finances rectificative 55 millions d'euros cet été 40 millions d'euros supplémentaires avec le dernier projet de loi de finances rectificative qui permettent de soutenir directement les réseaux d'aide alimentaire, donc les grandes associations et donc leur permettent de faire. Face aux contraintes liées à l'inflation problématique d'approvisionnement et de crise énergétique, il bénéficie d'ailleurs par ailleurs des des dispositifs qui ont été mis en place pour faire face à cette crise de l'énergie, donc avis défavorable du gouvernement sur cette question, concernant l'amendement 500 qui concerne le fond d'appui territoriale, au développement des résidences de répit, partagez-vous dire que évidemment le répit est un sujet de forte préoccupation pour le gouvernement, qui l'avait d'ailleurs inscrit dans la précédente stratégie nationale, agir pour les aidants 2020, 2022 dans cette stratégie, donc on avait un cadre pour le, pour développer l'offre de répit et d'accueil temporaire on a par ailleurs missionner l'IGAS pour évaluer cette cette stratégie et à la question de la solution. nous attendons les conclusions les conclusions de la mission de l'IGAS, je suis désolé, c'est difficile de répondre de façon rapide et donc pour ces raisons, nous vous proposons de rejeter cet amendement, l'amendement 550 concernant le versement automatique du du RSA, là aussi, nous partageons vos préoccupations, c'est l'objectif du chantier de solidarité à la source, que j'ai engagé qui va viser à s'appuyer sur les informations dont disposent les différentes administrations sur les situations des personnes pour s'adresser à elle et donc d'aller vers les potentiels bénéficiaires nous commencerons dès 2023 avec une expérimentation territoires 0 non-recours qui avait été prévu dans la loi 3DS et qui permettra d'expérimenter ce cette lutte contre le non recours dans une dizaine de départements des trucs, le 712 sur les crédits supplémentaires pour étendre le RSA aux moins de 25 ans ça ne vous étonnera pas que le Gouvernement émet un avis défavorable à ce sujet, puisque un certain nombre de dispositifs existent déjà pour les moins de 25 de de moins de 25 ans, pardon, ils ont accès notamment à la prime d'activité, ils peuvent bénéficier de l'accompagnement vers l'emploi du plan, un jeune une solution et depuis le début de l'année 2022 ils ont accès au contrat d'engagement, jeune, le gouvernement est pleinement mobilisé pour venir en soutien à la jeunesse, néanmoins, nous pensons que, il faut que nous fassions en créant les conditions d'une meilleure insertion sociale et professionnelle, d'où l'ensemble de ces dispositifs et d'où le travail que nous faisons actuellement dans le cadre de la réforme France travaille donc avis défavorable sur cet amendement sur le 668 la question du maintien des crédits dans la lutte contre le non recours à l'aide à la vie familiale et sociale si le montant qui figure dans le projet de loi de finances et le résultat d'une projection, il n'est en aucun cas limitatif donc toutes les personnes qui peuvent légitimement bénéficier de cette aide n'auront aucune difficulté à l'apercevoir en 2023 donc, le gouvernement est défavorable à cet amendement concernant le d'un monde mon numéro, je vais dire une bêtise. l'amendement 673 avis défavorable à cet amendement, vous souhaitez augmenter donc les moyens mobilisés pour lutter contre le non-recours à la complémentaire santé solidaire toutes ces démarches de lutte contre le non recours feront partie là aussi des travaux solidarité à la source et lutte contre le non recours de façon de façon générale, on a mis en place un certain nombre de mesures, notamment d'aller vers pour en direction des des populations les plus fragiles pour les aider à bénéficier de cette, de cette aide sur le 574 création d'un nouveau programme, dans le but de supprimer la situation des sans-abri, cet amendement relève plus de la mission cohésion des territoires donc qui porte les crédits dédiés au logement et à l'hébergement d'urgence, nous rejetons cet amendement et enfin le 667 sur la création d'un nouveau programme portant sur la publication du rapport sur le revenu universel d'activité, je vous l'ai dit, nous sommes engagés dans le projet de solidarité à la source, porté par le président de la République, c'est une réforme ambitieuse et qui va bien au-delà du revenu universel d'activité, c'est pour cela qu'on n'a pas repris, effectivement, les conclusions du rapport Lenglart on a néanmoins demandé à l'adresse de travailler à de nouvelles projections dans le cadre du projet de solidarité à la source et donc pour ces raisons, nous sommes défavorables à votre amendement.

ça va être plus logique. Merci donc globalement ce je tiens à rappeler que, en matière de d'enfance comme je l'ai dit, je n'ai pas le monopole de toutes les lignes budgétaires puisque mon collègue ma collègue sur le handicap, mon collègue sur la pauvreté, l'école, la justice l'aide alimentaire, tout le monde contribue au bien-être de nos enfants sur la protection de l'enfance comme je l'ai expliqué cette année est une année de transition, j'ai obtenu le maintien de la fin, je vous propose le maintien de la contractualisation à hauteur de 140 millions d'euros auxquels s'ajoutent 50 millions dédiés aux jeunes majeurs, on avait déjà eu 50 millions sur le budget 2022, on propose de maintenir 50 millions sur le budget 2023, étant entendu qu'aujourd'hui les départements ont des difficultés à évaluer leurs besoins et qu'on pourra toujours rectifier le cas échéant ses besoins venait à augmenter, ce qui est important pour moi, c'est d'améliorer la gouvernance La gouvernance nationale, j'y reviendrai avec logique, mais aussi la gouvernance territoriale dans le cadre des conseils départementaux de protection de l'enfance nous travaillerons cette question de contractualisation avec des objectifs extrêmement précis, nous évaluerons ce qui a été fait en 2022 2021 pour pouvoir améliorer nos demandes pour le budget 2000 L'objectif c'est donc d'une efficacité des dépenses s'agissant du comme il a été dit-il, sera créée au 1er janvier 2 2023 le financement à parité connaît une exception sur cette année de transition, nous considérons qu'aujourd'hui que le programme 300 Kate et calibrée pour financer les mesures nouvelles qui sont relativement limités, il sera ajouté éventuellement, si nécessaire, nous n'avons pas encore commencé à à dépenser, évidemment, mais surtout, il nous faut laisser un peu de temps à ce pour voir s'il arrive à mettre en oeuvre toutes ces mesures nouvelles, s'agissant des préconisations de la civile, je tiens à dire que il ne faut pas oublier que non seulement il y a le programme de 300 quatre mais bien sûr l'Ondam et le firent contribue largement à la politique de prévention et de lutte contre les victimes et de prise en charge des les victimes de violences sexuelles sur les Apaid, nous avons quand même hein, au total 16 millions d'euros qui sont donnés à enfin qui sont prévus entre les 2 Budgets firent Ondam et le budget qui vous est présenté aujourd'hui aujourd'hui 7 4 millions d'euros avec un virgule 3 millions de mesures nouvelles, donc, pour les Hug pète ces unités tout à fait, dédié à la prise en charge des enfants victimes à la fois à la détection, l'accompagnement judiciaire et, bien sûr, la prise en charge la formation des professionnels reste évidemment un axe important qu'y compris dans les Budgets qui vous est proposé la plateforme téléphonique. Madame la ministre, s'il vous plaît,

sont sur le il y a, il y a des amendements sur le financement. Bon, en tout cas, si je résume je suis défavorable à l'ensemble des, des, des amendements et je vous fais des réponses groupés pour aller le plus vite possible. J'essaie d'avoir une réponse concrète, excusez-moi mais bon en regroupant parce que les sujets sont sont un peu mélangé sur les recommandations de la civile je répète que nous mettons effectivement dans ce budget 7 4 millions pour les yeux, dont 1,3 1000000 de mesures nouvelles sur la plateforme téléphonique dédiée, nous faisons, virgule 5 millions d'euros, dédié à une campagne de communication sur les jeunes majeurs comme je l'ai dit, les 50 millions sont passés de la stratégie pauvreté à la stratégie, protection de l'enfance, évidemment nous serons particulièrement vigilants et nous travaillerons avec les départements, dans le cas des CD DPE sur les insertion des jeunes dans les territoires ruraux, comme l'a dit mon collègue les dispositifs et pris en charge, notamment par le ministère du Travail, nous serons particulièrement attentifs à la à la façon dont le contrat d'engagement, jeune et l'accompagnement des jeunes majeurs se fait dans les territoires ruraux, le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'enseignement supérieur, contribue aussi à l'accompagnement des jeunes en ruralité sur la prostitution, un plan de 14 millions d'euros a été déployé, aujourd'hui nous allons de 2 millions supplémentaires pour financer l'amélioration des repérages dans les maraudes numériques et le développement de structures spécialisées, voilà, voilà donc l'ensemble des des amendements ne me paraît sans objet et je demande le rejet.

permettent la revalorisation de l'ensemble des métiers, financé par le programme 137 pour permettre la généralisation de la prime du Ségur aux salariés du programme 137 hé bien en fait, c'est justement ce qu'a prévu l'amendement du gouvernement que vous avez adoptées et qui visent à permettre la compensation du Ségur aux structures de la branche sanitaire et sociale non médicaux sociales dont font justement partie les structures oeuvrant dans le Champ de l'égalité femmes-hommes, je vous propose donc de retirer cet amendement.

et 714 relatifs au parcours de sortie de la prostitution et à la FIS aide financière à l'insertion sociale, donc juste pour vous indiquer que toute cette toute cette politique est financé par le programme 137 à hauteur de 2 5 millions d'euros pour les têtes de réseau et la FIS plus de un 1000000 d'euros au niveau local accompagner les personnes en situation de prostitution en 2022 au titre des mesures nouvelles se sont ajoutées 2 millions d'euros pour financer les parcours de sortie et la FIS et je précise que, s'agissant justement du montant de la FIS, il a été revalorisée de 4 % à compter de juillet 2022, et que cette mesure est intégré dans le PLF 2023 dans le cas d'une mesure nouvelle, hauteur de 200000 euros donc je propose soit le retrait de cet amendement, ou à défaut je serai défavorable S'agissant des de l'Observatoire des féminicides, c'est le l'amendement 542. Donc défavorable compte tenu du fait que, il y a une étude sur les morts violentes, publié chaque année par le ministère de l'Intérieur, des retours d'expérience ordonné maintenant depuis la les suites du Grenelle donc ordonné par le ministre de la justice, donc, qui demande au Parquet de faire remonter des retours. Fayence après chaque féminicides et puis je précise aussi que nous avons des observatoires territoriaux qui sont mis en place donc dans différents territoires et que j'attacherai d'ailleurs une importance particulière au développement de ces observatoires territoriaux qui permettent de voir au mieux justement la réalité. Des violences faites aux femmes et en particulier des féminicides, donc je serai aussi comme je l'ai indiqué à cet amendement, voilà madame la présidente. Merci. Hé ben, Madame la Ministre, je pense que vous faites tous les autres, aller. Dis donc, il s'agit donc des des amendements 509 et 541 qui concerne les ESAT et le fond de transformation des ESAT alors vous le savez, tout et tout se font de transformation a été mis en oeuvre l'an

sont en cours, même pas d'attribution, les projets sont en cours de repérage et d'arbitrage au niveau des ARS qui feront des contractualisation avec les projets retenus, de façon progressive entre cette fin d'année et le 1er semestre de l'année 2023 ces fonds ne sont pas utilisés aujourd'hui les fonds de 2022, donc ils sont à disposition pour l'année 2023, ce que nous vous proposons cette d'évaluer ce que ces fonds auront la façon dont ils auront été consommé et de prévoir pour 2024 une avancée sur ces fonds de transformation des ESAT parce que ces fonds sont importants néanmoins puisque ils vont participer à la transformation de ces établissements et surtout à la aux investissements dans l'outil de production qui permettra d'évoluer dans les les modes de formation et de de d'emploi des personnes en situation d'handicap, donc je vous propose ou de retirer ces amendements ou ben je me je me j'ai un avis défavorable. donc moi j'ai un peu trop mais bon peut être que c'est bien bon de toute façon vous êtes défavorable à tous voilà donc on va mettre aux voix à Madame la ministre, vous avez demandé non. Bon, donc je vais mettre aux voix, donc ces amendements. Pour le gouvernement, donc tous les avis sont défavorables à moins que vous retiriez un amendement donc je commence par le 422 donc avis de la commission défavorable. Gouvernement aussi qui est pour, qui est contre.

533 même avis même vote le 535 même avis même votre 538 plein ma vie même vote le 539 même avis même vote.

donc les amendements identiques 385 416 658 donc avis défavorable de la commission du gouvernement Monsieur Mounier. Madame la présidente, moi j'interviens aurait été pour l'ensemble de ces amendements, qui concerne le même sujet, qui soient des crédits supplémentaires, moi ce que je vous propose, j'ai entendu il avait de la commission, je ressens que bien entendu l'avis du gouvernement, de sang, vous auriez pu devenir qu'un seul ministre on aurait eu une vision globale de la ville négatif du gouvernement sur l'ensemble, mais pour revenir sur ces amendements, ce que je propose c'est peut être de soutenir mon amendement là le l'amendement de 60 qui a le même objet, et qui apporte des crédits, on va dire plus raisonnables à la contribution, donc ça donne le message des moyens supplémentaires pour l'accompagnement des jeunes majeurs sont pour s'aggraver de façon trop importante, les hotlines budgétaires, donc si vous en êtes d'accord,

Madame le Ministre, on connaît tous des difficultés justement moi aussi dans le département de la Marne j'ai eu l'occasion de rencontrer l'UDAF et des difficultés donc avec la protection des, des, des, des majeurs, c'est la raison pour laquelle il nous paraît important et visiblement, pour un un nombre de sénateurs sur tous ces bancs de faire en sorte de donner des, des, des, des moyens supplémentaires, c'est la raison pour laquelle moi je soutiendrai ces amendements, alors j'ai connu signé l'amendement de de Monsieur Lefebvre avec d'autres et je crois que pour tenir compte effectivement des des soucis budgétaires, il serait peut-être intéressant de se rallier, me semble-t-il et Docteur Chassaing et d'accord également de se rallier à la proposition de de Philippe mouiller ça donnera quand même un signe positif dans cette demande-là tout en respectant l'épure budgétaire. ça varie, vous retirez la, l'amendement donc de Monsieur Lefebvre Merci madame la présidente, donc moi effectivement que là, dans mon département, j'ai beaucoup de problèmes effectivement que la protection des des jeunes majeurs mais je comprends qu'il faut aussi faire des efforts et je veux bien me rallier à l'amendement de Philippe mouiller. Merci sur le rapporteur. Merci madame la présidente, mesdames les ministres, monsieur le ministre, il me semble, sous votre contrôle vous avoir entendu dire que dans ce dans le cadre de ce budget, il y avait une progression de 12 millions d'euros sur cet item protection des majeurs. un non, et la demande est de 40 millions dans l'amendement j'avais demandé l'avis du gouvernement, pour avoir une idée de du Delta. Le l'avis de la commission des finances, évidemment, est empreint de sagesse budgétaire donc dans la mesure où il y a 7 millions déjà de progression et des difficultés de recrutement des difficultés aussi pour former les personnels, on en restera donc un avis défavorable, mais avec une vigilance particulière, l'année prochaine, puisque manifestement nous dit qu'il y a des problèmes sur le terrain un peu partout,

amendement 537 donc avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient. Pas adopté amendements identiques 549594 même avis. Même votre l'amendement 710 même. si vous voulez, même la président Billon, donc nous mettons la, l'amendement 594 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour.

Amendement 554 avis favorable de la commission avis défavorable du gouvernement même Leblanc. Oui, oui, merci, madame la présidente,

une ligne de 10 millions d'euros dans le PLFSS je suis allée voir hein, mais cette ligne, elle est, elle, est certes à la main des ARS, mais elle est entièrement consommé et on ne peut absolument pas aujourd'hui penser qu'une ARS pourra dégager un 1000000 d'euros, pour un un projet dans un département, donc même si vous m'avez parlé d'une d'une d'une d'une enquête de l'IGAS, enfin d'une étude de l'IGAS, je trouve un petit peu dommage que vous ne que vous ne puissiez pas dégagé 10 millions 12 millions d'euros sur ce budget ce qui quand même n'est n'est pas extraordinaire je je je ne comprends pas, pour pouvoir commencer à régler ce problème qui pourtant vous tient à coeur. Merci Monsieur Oui, madame le président, je serai également cet cet amendement parce qu'au-delà de de l'état du vous avez fait, monsieur le Ministre, d'abord un concrètement aujourd'hui il y a pas de moyens dédiés au développement de ce type d'opération de maisons de répit d'ailleurs pouvoir consulter la CNSA, ils sont Hog allemand se favorable, enfin pas favorable à l'amendement, mais en tous les cas, ont besoin d'un fléchage complémentaires sur ce type de financement à hauteur de 10 millions d'euros et concernant le la mission mis en place par l'IGAS, le débat, c'est le délai puisqu'on a en face de renvoyer à une réflexion plus globale sur la branche donc voilà donc dans l'attente, je pense qu'il serait extrêmement intéressant de soutenir cette initiative, les projets sont prêts sur les territoires, le 1er d'ailleurs demain devrait démarrer dans les Landes, on a aujourd'hui des phases opérationnelles, les ARS, ils sont plutôt favorables, ce problématique aujourd'hui, c'est les premiers crédits envoyé voilà ah difficile 10 millions parce qu'il y a 10 projets je pense réellement aujourd'hui, c'est un besoin extrêmement important et qu'il faut être acteur de ce développement. Merci, monsieur le Ministre. Juste vous préciser que ça fait bien partie des mesures nouvelles de loger des dans le PLFSS PA PH, il y a bien dix millions d'euros pour les aidants dans le PLFSS et d'ailleurs c'est des crédits CNSA donc ça doit être dans le PLFSS. Merci à l'heure, je mets aux voix l'amendement 554 qui a reçu un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement. Et pour qui est contre qui s'abstient. Il est donc adopté l'amendement 599 et même à présent Billon. Oui, madame la présidente, merci de redonner la parole, moi je voudrais juste rappeler que le j'ai entendu le le rapporteur qui nous disait qu'il voyait plutôt ça dans le budget de la justice, je voudrais juste rappeler que j'ai parlé de cette. à 10000 jeunes mineurs qui se prostituent l'année dernière il y avait des budgets parce que c'était un reliquat lorsqu'on fait des politiques publiques, on s'engage pas pour une année, on s'engage dans la continuité il y a pas de budget fléchés pour la prostitution des mineurs, alors ça sert à rien demander des études ou des missions à la procureure Renault qui a fait un travail formidable, avec des propositions, si on donne pas les moyens derrière d'appliquer ce programme et ses propositions qui qui qu'elle a porté, nous l'avions auditionnées avec la délégation aux droits des femmes 7 à 10000 1000 mineurs, je le répète, donc nous vous avons besoin d'argent pour aider ces ces jeunes mineurs, donc je vous demande chers collègues de voter cet amendement parce que si on renvoie la balle à la justice, le budget de la justice, il est passé donc c'est terminé, on ne protégera pas les mineurs qui se prostituent en 2023. moi j'espère surtout que tout ceux qui. Sont présents, qui demande la parole là aujourd'hui seront là samedi également merci beaucoup. Donc je mets aux voix l'amendement 599 via à Madame la Ministre. comme le rapporteur l'a dit, le plan de lutte contre la prostitution a été sorti très tard dans l'année 2022, les appels à projets viennent juste d'être attribuées et donc on commence à dépenser l'argent qui a été attribué en 2022

Voilà un président de pardonnez-moi mais là depuis tout à l'heure, on ne peut pas écouter les avis à la fois des des rapporteurs des ministres de certains collègues qui ont déposé, qui ont pris du temps à déposer des amendements, je sais qu'on est dans un temps contraint mais on est aussi là pour débattre

le règlement intérieur est prévu ça, ça c'est la c'est la règle maintenant moi il y a pas de souci, moi c'est simplement qu'il va pas falloir venir me dire que j'aurais dû accélérer pour que justement cette mission ne soit pas examinée en partie samedi il y a l'ensemble des ministres aussi à l'ensemble des collègues, monsieur Iacovelli je osais pas donné la parole, c'est bon. Alors maintenant je mets aux voix l'amendement 599 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour.

C'est contre.

la vie même votre 712 même avis même votre amendement 329 avis favorable de la commission. Et le gouvernement. Je sais pas qui, qui a donné défavorable également. Donc, il est pour, qui est contre qui s'abstient parce qu'il est adopté, amendement 543 qui a reçu un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contraint qui s'abstient, il est adopté et fait tomber le suivant: le 714 668 avis défavorable de la commission du gouvernement qui est. Pour qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, amendement 542 même avis même votre amendement 500 même avis même votre amendement 573 même avis même votre amendement 574 même avis même votre amendement 667 même avis même vote. Les merci alors, nous passons à l'amendement 575 madame Poncet mon. Merci madame la présidente, alors un large pan des professionnels de la filière sociaux et éducatifs tels que les personnels logistique technique administratif reste encore écarté de la revalorisation salariale de 183 euros Net contenues dans le Ségur de la santé par exemple, si la médiation firme familiale s'inscrit dans au niveau politique que budgétaire sur la ligne de soutien à la parentalité, les médiateurs et médiatrice familiaux sont exclus désaccord du Ségur aussi les professionnels des sacs d'Etihad espace de la convention bad ne pouvant cumuler le bénéfice du Ségur et de l'avenant 43 qui était, je le rappelle, un accord de branche antérieur à la crise sanitaire se trouve à nouveau défavorisés par rapport aux autres établissements sanitaires et sociaux, médico-sociaux notamment les Epad et voilà leur crise d'attractivité perdurer et s'aggraver le Ségur, de l'aveu même du 1er ministre à une urgence et à une injustice nous proposons donc de corriger une fois pour toute cette injustice et d'allouer la prime de 183 euros ou aux oubliées du Ségur à savoir toute personne travaillant dans un établissement de la filière socio-éducatif au médiateur et médiatrice familiaux ainsi que les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les centres de soins infirmiers de la branche branche ceux d'aide à domicile, 2 ans après, il est quand même grand temps de mettre fin aux oubliées du Ségur et aux distorsion entre secteurs comme en infra-secteur établissements par cet établissement d'appel nous proposons donc la création d'un nouveau programme, élargissement du Ségur sociale à tous les personnels des établissements que j'ai cité précédemment, je vous remercie. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui merci Alain présidente le présent amendement propose une ouverture de crédits à hauteur de 500 millions d'euros pour financer la revalorisation salariale des services à complet d'accompagnement et d'aide à domicile, l'extension de la mesure choc du Ségur aux travailleurs sociaux s'élève dans ce PLF à près de 50 millions d'euros en outre 20 millions d'euros sont prévus pour la revalorisation des travailleurs dans les services de protection maternelle et infantile, il s'agit, à notre sens, d'un amendement d'appel destiné au gouvernement, c'est donc une demande de retrait pour nous.

qui est contre qui s'abstient n'est donc pas adoptée. 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune 2 amendements identiques, monsieur le Président, Ruquier. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs et mesdames les ministres, chers collègues, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé est une avancée très importante pour les personnes handicapées, elle va enfin mettre un terme au lieu de ne dépendance financière pour les bénéficiaires de la hache et son conjoint et ainsi assurer plus d'autonomie aux personnes concernées, cette réforme 100000 Hanovre au 1er octobre 2023, le temps que les différents outils sont mis en place, toutefois, lors du débat du projet de loi, pouvoir d'achat, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, j'ai dit favorable à une entrée en vigueur, plus rapide et, si cela s'avérait possible techniquement aussi cet amendement qui est porté par Maryse Carrère vise à octroyer davantage de crédits au programme 157 Handicap et dépendance pour permettre le financement de la déconjugalisation avant octobre 2023 afin que les bénéficiaires de la hache puissent bénéficier au plus vite cette réforme.

vingt-trois et interroger le gouvernement sur une potentielle rétroactivité de la mesure, à compter du premier avril 23, rappelons que la bande danse financière vis-à-vis de son partenaire qui entraîne se de Quaku à l'actuel pénalise tout particulièrement les femmes en situation de handicap, vivant en couple plus susceptibles d'être victimes de violences conjugales, on estime que 34 % dans telle d'entre elles subissent des violences commises par leurs partenaires, contre 19 % de femmes dans handicapés. Merci le 540 madame le héros. Alors il s'agit d'un amendement qui vise à étendre au-delà de 60 ans, le droit de toucher la hache pour les personnes qui en sont titulaires avec un taux d'incapacité permanente située entre 50 et 79 % il y a un trou de couverture entre la fin de la âge à 60 ans et le potentiel et le potentiel bénéfice de l'Aspa, donc l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui, elle, ne peut démarrer que à partir de 62 ans, donc il y a vraiment un trou de couverture, qu'il s'agit ici de combler. Merci l'avis de la commission, cela rapporte. nous avons interrogé lors de nos auditions, l'administration, la Dgccrs sur le sujet, il nous a été effectivement dit que elle se heurter à des obstacles techniques importants, il nous a été indiqué que l'ensemble des systèmes d'information relatifs aux prestations sociales était à ce jour, fondé sur une logique familialisé et que la mesure impliqué à cet égard, d'importants travaux d'adaptation, nous sommes restés un peu perplexe, je voudrais que le gouvernement nous confirme qu'il s'agit effectivement de problèmes techniques de mise en oeuvre de de cette déconjugalisation au premier avril sur le 540 l'amendement visant à étendre au-delà de 60 ans, le droit de toucher l'âge pour mémoire, l'âge de est versée aux personnes dont le taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % contre 80 % au moins pour la H hein et subissant des restrictions substantielle et durable d'accès à l'emploi, il s'agit donc d'une prestation destinée par nature aux actifs passé l'âge de 60 ans, les personnes concernées relève donc de l'assurance vieillesse ou de l'Aspa, en tout état de cause, la règle selon laquelle le bénéfice, l'âge de prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail est prévue par l'article L. du code de la sécurité sociale, cet amendement de crédit doit être doivent donc être considéré comme un un amendement d'appel, on peut tout de même interrogé le gouvernement sur la fixation de cet âge à soixante ans soit avant l'âge de la retraite, bon pour ces trois amendements, c'est une demande de retrait mais avec demande de précisions du gouvernement sur l'aspect technique. Merci l'avis du gouvernement, madame la ministre. Merci madame la la présidente oui là je la déconjugalisation, la mise en oeuvre de la déconjugalisation, et beaucoup le plus technique, on ne peut l'imaginer, notamment pour la Caisse nationale d'allocations familiales et qui traite le système informatique qui construit le système informatique qui va permettre de pouvoir mettre en place pour les bénéficiaires, cet âge, donc nous nous sommes engagés à. Mettre en place des décrets qui sont en cours d'examen actuellement au niveau de la CNCPH qui seront signés vers mi-décembre et ensuite la Caisse nationale d'allocations familiales travaille sur ce système d'information qui est complexe, qui est très complexe, parce que cette caisse n'a pas l'habitude de travailler avec des revenus déconjugaliser au contraire, tout, tout le les quotients familiaux sont sont du système de construction du système d'information de la caisse, donc c'est pour le premier octobre et ce à quoi je me suis engagé, c'est que si les choses étaient prêtes techniquement avant ce serait mis en oeuvre dès qu'elle serait prête, techniquement, l'important est que les préparations soit fine afin qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de bug à la mise en oeuvre de de l'âge déconjugaliser pour les usagers pour la H hein et de vous l'avez dit, jusqu'à l'âge de 62 ans permet d'assurer son continuité avec l'âge d'ouverture des droits à une pension de retraite et à l'ASPA, il ne paraît pas souhaitable, en revanche, d'aller au-delà et permettre aux bénéficiaires de la hache de de percevoir, celle-ci sans limitation de durée, comme c'est le cas pour les bénéficiaires de l'AAH pour bénéficier de la hache de la personne doit avoir donc un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, mais celui-ci doit être assortie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, elle ne peut être attribuée pour une durée supérieure à 5 ans contrairement à l'âge, hein, qui peut être attribuée sans limitation de durée, donc la possibilité pour les filles, le bénéficiaire de l'âge, hein, de conserver la prestation au-delà de l'âge de la retraite se justifie au regard de la possibilité de se voir reconnaître un droit sans limitation de durée et les bénéficiaires de la hache de ont la possibilité de faire une demande d'ASPA, dont le montant est comparable à celui de l'âge

C'est contre. Qui s'abstient ne ne sont pas adopté l'amendement 540 avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour.

Merci madame la présidente, cet amendement vise à mettre fin à une injustice dans la fonction publique hospitalière pour quelques professionnels travaillant dans des établissements médico-sociaux, en particulier dans les secteurs du handicap et de la protection de l'enfance, ce sont les oubliées du Ségur, c'est 0 3 % des personnels de la fonction publique hospitalière qui ne bénéficient pas du complément de traitement indiciaire soit 183 euros mensuels les établissements médico-sociaux ne peuvent pas lutter contre le départ de leurs salariés vers des aides des établissements ou des postes équivalents sont valorisés par un gain de pouvoir d'achat, ces fortes disparités entre les personnels fragilisés désorganise ces établissements qui peine à conserver leurs personnels et à recruter cet amendement propose donc un élargissement des bénéficiaires du complètement de traitement. Merci Merci madame la présidente, la pertinence de cet amendement sur les crédits de la mission Solidarité peut être interrogé, alors il semble davantage relever de la loi de financement de la Sécurité sociale, en tout état de cause, c'est à l'évidence un un amendement d'appel parce que le montant demandé, soit 15 millions d'euros ne nous semble pas correspondre réellement au coût du dispositif envisagé, c'est donc une demande de retrait. Merci même avis du blanc, même avis merci

que ça désorganise vraiment les établissements et que finalement, c'est la situation de ces jeunes qui ont besoin d'un accompagnement et d'une protection qui est mi-temps qui est mise en cause, pardon. Merci l'amendement 545 madame Le Houerou. c'est un amendement qui vise à octroyer 2 millions d'euros supplémentaires à la plateforme téléphonique 39 19 donc, la plateforme d'écoute et d'information et d'orientation à destination des femmes victimes de violences, il faut saluer tout d'abord, les efforts pour améliorer l'accueil téléphonique de 16 usagère en détresse, notamment l'évolution du fonctionnement de la plateforme en juin 2021 vers le vingt-quatre pour autant, selon le dernier bleu budgétaire cette plateforme à un taux d'appels traités en 2021 2 62 %, ce qui laisse 38 pour des usagères sans réponse, le gouvernement s'était fixé pour objectif dans le budget 2022 à 85 % de réponse en 2023, l'objectif est à la baisse à 75 %, donc c'est assez incompréhensible cette hausse donc du budget que nous demandons est nécessaire au regard de la pauvreté des moyens octroyés aux 39 19 et nous proposons donc voilà d'augmenter ce budget parce que le coût de ces non réponses et de la non prise en charge de de ces personnes, les coûts indirects sont plus important, une étude de plusieurs structures de recherches dont le Centre d'études européennes de Sciences Po, montre que le coup je dirais des violences sexuelles et sexistes est évalué à 3 6 milliards d'euros, donc ce coût pour la société est largement supérieur aux 2 millions d'euros supplémentaires qu'il vous est proposé d'allouer à cette plateforme. Merci, non, l'avis de la commission mamie, c'est d'abord l'avis de la commission sur le reportage. Merci madame la présidente, pardon, Madame la Ministre, ce sera très rapide, il nous paraît évident qu'il est nécessaire d'accompagner la montée en puissance du dispositif, passer de 24 heures 5 24h/24 et 7 jours sur 7 depuis le 2021, néanmoins le PLF prévoit déjà dans sa version initiale, une dotation dédié de de 9 millions d'euros, qui a été doublée en première lecture à l'Assemblée nationale l'amendement paraît donc satisfait, ce sera donc de la part de la commission des finances, une demande de retrait. Merci madame la ministre, de l'avis du gouvernement. Pardon, madame la présidente, comme l'a dit la Commission, effectivement, je suggère le retrait de cet amendement, puisque le PLF adopté en première lecture à l'Assemblée nationale a attribué 2 9 millions d'euros pour accompagner justement la structuration du trente-neuf 19 par la FNSF je précise d'ailleurs que le 2 fois plus d'appels sont pris en charge depuis 2017 on a à peu près 90000 appels et plus 114 % d'augmentation du budget du trente-neuf 19 depuis 2017 donc je propose de retirer cet amendement ou à défaut je je suis défavorable. Merci

Merci madame la présidente, cet amendement propose d'injecter 2 millions d'euros supplémentaires à l'action, dédié à l'égalité professionnelle afin tout d'abord, de mesurer les inégalités entre secteurs professionnels, puis l'impact qu'aurait des actions de revalorisation à leur juste valeur des métiers des secteurs à prédominance féminine l'index de l'égalité professionnelle, a permis depuis 2018 la publication annuelle des résultats des entreprises en matière d'égalité femmes-hommes sur les salaires en 2022 la note moyenne qui attribue de 80 6 sur 100 8 entreprises sur 10 serait donc parfaitement égalitaire et pourtant, comme chaque année, ce 4 novembre les femmes en France ont commencé à travailler gratuitement, selon le calcul des glorieuses du fait des inégalités persistantes de salaire entre femmes et hommes, alors quel est le problème, les critères de l'index de l'égalité ignorent un élément majeur, les inégalités entre secteurs professionnels, certains secteurs majoritairement féminin sont mal, voire très mal rémunérés comme les secteurs du prendre soin des aides-soignant les infirmières, les aides à domicile, les caissières et les caissières aussi ces métiers dont on a reconnu le caractère essentiel pendant la crise du Covid alors que faire le Québec en 1995 a décidé d'appliquer le principe de l'équité salariale tous les salariés ont reçu un questionnaire pour évaluer les spécificités de leur emploi et une étude a été conduite dans tout le pays pour prendre en compte ces données dans les salaires moyens et rééquilibrer les salaires par secteur,

nous gagnerons donc plusieurs décennies dans la lutte pour l'égalité, à faire de même et c'est pour cela que je que le le groupe vous propose cet amendement. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, cet amendement vise à renforcer de 2 millions d'euros, les moyens déployés au titre de l'index de l'égalité professionnelle, ce dispositif relève cependant du programme amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail de la mission Travail et emploi et en pratique de la direction générale du travail, il nous semble donc ça ne relève pas de de cette mission, et donc ce n'est pas le support approprié : demande de retrait. Merci l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, je m'associe à à la à l'avis de la commission s'agissant de cette demande de retrait ou sinon je j'ai bu un avis défavorable, précisant : tu également que c'est une somme totale de 143 millions d'euros, qui est affecté à l'égalité professionnelle, à travers la politique transversale adhère à travers la, le document de politique transversale menée donc sur ce sujet. Si, alors je mets aux voix donc cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement. Qui est pour, qui est contre qui s'abstient ne pas adopté l'amendement 597 la présidente Guillon. Merci madame la présidente, mes chers collègues, les Centre d'information sur les droits des femmes et des familles appelé CIDF sont des organismes de droit privé constituée sous forme d'associations, ils font l'objet d'un agrément par l'État afin de mettre à disposition des femmes et des familles, toutes les informations utiles tentant à promouvoir les droits des femmes, je connais leurs difficultés, je connais leur engagement pour tout toujours mieux accompagner ses victimes, alors je ne se félicite évidemment des un virgule 5 6 millions d'euros qui sont prévus au projet de loi de finances pour renforcer les CIDF et leur coeur de métier, cependant ces crédits ne prennent pas en compte la nécessaire revalorisation des salaires du personnel des CIDF qui n'a pas baisse des fichiers d'des revalorisations récentes, donc c'est l'objet de cet amendement revaloriser la subvention allouée allouée aussi des fêves, afin de garantir un juste niveau de rémunération des personnels de ces associations, je vous remercie. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente, comme l'a souligné, notre collègue et les auteurs de l'amendement un effort budgétaire a déjà été accompli par le PLF avec un relèvement de moyen de 1 virgule 6 millions d'euros pour le financement de l'État qui a au total à 6,3 millions d'euros, je voudrais qu'il y a des financements locaux aussi complémentaires, très important, c'est donc une demande de retrait. Merci la vie de du gouvernement, Madame la Ministre.

du CIDF pourront aussi bénéficier de la rivalisent de la revalorisation des salaires au titre justement de la prime Sigur puisqu'elles font partie, elles et ils feront partie justement de ce Champ visé par par la généralisation de cette prime, donc je, je propose que cet amendement soit retiré ou à défaut je j'ai pas d'avis défavorable. Merci donc je mets aux voix l'amendement 597 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. qui est contre Il n'est pas adopté, contre la précarité menstruelle en octobre 2019 rendez en effet un rapport intitulé précarité menstruelle changeons les règles ce rapport mettait en lumière la détresse dans laquelle se trouvaient et se trouve encore aujourd'hui près de 2 millions de femmes en France au moment de leur règle pour ces femmes, souvent en situation de précarité, avoir accès à des protections périodiques revient souvent à devoir choisir entre des besoins aussi essentiels que l'hygiène ou l'alimentation, je parle de choix, même s'il ne peut choisir que l'un d'un choix contraint car l'on ne décide pas d'avoir ou non, ces règles avec ce rapport, il s'agissait donc de lever le voile sur le tabou que représente les règles et d'insister sur la nécessité d'y consacrer un Verit une véritable politique publique les règles s'avère encore pour trop de femmes un facteur d'exclusion et d'aggravation des discriminations qu'elles peuvent connaître dans le prolongement de ce rapport, j'avais appuyé avec mes collègues et des pays, l'expérimentation de la mise à disposition gratuite des protections en direction des publics les plus fragiles, ce sont ainsi un million d'euros qui a, qui a, il y avait été consacré effort porté ensuite à 5 millions d'euros en 2000, est reconduit pour le même montant, dans le cadre du projet de loi de finances 2023 si je salue la prise de conscience du gouvernement sur ce sujet et l'engagement du président de la République en la matière, il faut reconnaître qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir aussi l'amendement défendu propose d'accroître de 20 % les moyens financiers consacrés à ce sujet, il s'agit d'un effort non négligeable mais qui reste raisonnable et qui est surtout légitime au moment où l'accès à des protections périodiques et les rondies encore plus difficile du fait de la hausse généralisée des prix je conclurai en remerciant notamment les sénateurs de mon groupe mais aussi ceux du groupe écologiste qui s'engage et soutiennent avec moi ce combat et j'espère que le gouvernement, qui n'est pas en reste, de ce de ce sujet ça, être attentif à cette proposition.

Il faut comprendre quand même que cet amendement est complémentaire des mesures dont vient de parler, hein, de cette fameuse ligne à 5 millions d'euros, qui a été reconduite et dont ce dont se félicite mais c'est et ça, il s'agit un petit peu de de mesures complémentaires afin d'accroître les actions de sensibilisation sur les menstruations et le bon usage des protections périodiques en milieu scolaire et auprès des femmes précaires et aussi de permettre la formation d'intervenants sociaux sur ces sujets, donc c'est c'est un petit peu, hein, une mesure d'accompagnement pour rendent tout à fait efficient les, les, la ligne de 5 millions d'euros, qui a été reconduite. Voilà, merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, c'est un sujet dont nous avons débattu à plusieurs reprises ici même, donc il est proposé d'ajouter un million un budget de 5 millions d'euros, je note toutefois qu'un effort budgétaire a déjà été menée dans dans un sens favorable puisque ces produits sont maintenant soumis à un taux de TVA deux réduit de 5,5 % je crois qu'il sera d'ailleurs intéressant de regarder l'évolution des prix ces dernières années pour voir si ce genre de mesure est efficace ou pas, parce que c'est un sujet qu'on a régulièrement en commission des finances, et ici même en séance publique, mais au-delà de de cette remarque : nous avons rendu un avis de sagesse.

un sujet qui est essentiel pour l'inclusion des des personnes qui sont en situation de de précarité et en particulier des des femmes, vous l'avez dit, on a fait un effort important en reconduisant le budget de 5 millions d'euros vous dire aussi que, il y a d'autres crédits qui sont consacrés à l'accès à l'hygiène dans le soutien qu'on apporte aux associations de lutte contre les exclusions et ce sujet fera l'objet à la fois d'une évaluation d'une réévaluation, dans le cadre de la mise en place du pacte des solidarités à partir de, de 2024 donc si vous voulez bien, je vous propose de retirer votre amendement pour qu'on continue sur cette lignée en 2023 et on continuera à investir sur cette question pour les années suivantes.

Merci madame la présidente, avec cet amendement, je vous propose de rehausser les crédits alloués au financement des centres de prise en charge des auteurs de violences, élément essentiel dans l'arsenal de lutte contre les violences faites aux femmes, ces centres ont été développées après le Grenelle des violences conjugales et on on décompte une trentaine aujourd'hui sur tout le territoire se sentent présente de nombreux avantages que je vais pas développer ce soir pour gagner du temps, donc la mise en en place de ces centrales nécessite des moyens, c'est l'objet de cet amendement, la prise en charge des auteurs de violence doit faire partie de l'arsenal encore plus de lutte contre les violences faites aux femmes, je vous remercie. explique déjà la majeure partie de la hausse des dépenses relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes dans le budget qui ne proposer cette année, il nous semble qu'il faut maintenant laisser le temps au dispositif de monter en puissance alors que les centres sont à peine créé, d'ailleurs, les auditions que nous avons conduite ne nous ont pas permis d'identifier une problématique particulière de sous-financement en la matière, en revanche, Madame la Ministre, en revanche, les associations, avec qui nous avons échangé considère que le financement de ces centres devraient relever du budget de la justice et non du programme 137 dont l'objet devrait être centré sur le soutien aux victimes demande de retraite. Merci la eu du gouvernement, Madame la Ministre. Oui effectivement madame la à la présidente : pas de protection des victimes sans prévention de la récidive, nous sommes bien d'accord, les 30 centres de prise en charge aurait été ouvert, on a accueilli plus de 12000 personnes déjà

prévoyait des cofinancements et que justement les CP-CE1 sont en train de développer leur partenariat, donc il est un peu tôt effectivement pour abonder les Budgets qui leur sont octroyés donc je propose que cet amendement soit retiré ou à défaut je j'émets un avis défavorable. Merci donc je mets aux voix l'amendement 624 qui a reçu, donc un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour.

Merci madame la présidente, alors par cet amendement d'appel, nous demandons la mise en place d'un revenu minimum garanti, afin de permettre à chacune et chacun de vivre dignement le récent rapport du Secours catholique, état de la pauvreté en France, 2022 souligne que 2 ans après le début de la crise 48 % des des ménages rencontrés par l'association en 2021, se retrouvent dans l'incapacité de couvrir leurs dépenses alimentaires quotidiennes ces dernières années, l'écart entre le taux de pauvreté avant redistribution et le taux de pauvreté après redistribution ne cesse de grandir, soulignant le rôle majeur des prestations et aide face à l'appauvrissement et la précarisation d'une partie de la population, toutefois, hé bien que participant largement à la réduction de 7 virgule demi du taux de pauvreté par les prestations sociales, les minima sociaux ne garantissent pas un niveau de vie suffisant et descend la stigmatisation des allocataires et les montants de prestations trop faible maintiennent une partie de nos concitoyens dans des situations de détresse qui les éloigne de l'emploi et du logement, des sphères essentielle à l'intégration sociale, le revenu minimum garanti, consiste en un minimum social pour chaque adulte sans emploi ou ayant de faibles revenus, sans contrepartie, et ce dès 18 ans, son montant à hauteur de 60 % du revenu médian permet de garantir à chaque individu, des conditions d'existence non inférieure au seuil de pauvreté, la mise en place d'un revenu minimum garanti est non seulement une réponse à l'urgence sociale, mais aussi une mesure de justice, il s'agit enfin de privilégier l'action structurelle aux mesures ponctuelles. Merci beaucoup à leur juste, je vais me permettre, en tant que président de la séance de vous dire que nous allons être dans je sais pas trois minutes je pense à 19 donc je veux bien prolonger de cinq minutes mais je peux pas aller au-delà, donc chacun effectivement peut défendre son amendement en se moquant de ceux qui sont derrière et qui devront revenir samedi donc l'avis de la commission monsieur. Monsieur le rapporteur, merci l'avis du gouvernement, même avis je mets aux voix donc l'amendement 576 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est. Pour qu'il est contraint qui s'abstient mais pas adopté l'amendement 670 même pensé mange.

il s'agit donc bon ben je je passe, je passe les raisons. Bon, il est défendu mais je trouve ça quand même, mais enfin là je tiens quand même à utiliser les secondes pour dire que les violences faites aux femmes, on a manifesté, c'est toujours un problème en France et donc il est temps de donner les crédits à la hauteur de ce qu'on demande à savoir. Comme bien d'adoption, le sujet, mais la vie, la commission demande de retrait, l'avis du gouvernement, même avis. Même avis je mets aux voix donc l'amendement 170 défavorable de la commission du gouvernement qui. Pour qui est contre qui s'abstient donc pas adoptée. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission Solidarité, insertion, égalité des chances, figurant l'étape taper, je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite je vous rappelle que la commission des finances, est favorable à l'adoption des crédits de cette mission j'donc le mettre aux voix qui est. Pour qui est contre, s'abstient. Donc adopté l'article 46 quater et les amendements tendant à insérer des articles additionnels sont attachés, pour leur examen aux crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, je vais mettre l'article 46 quater

Merci madame Méliès l'amendement que nous vous proposons vise à permettre la mise en oeuvre dans mon département, d'une avancée majeure que nous avons voté ici, l'été dernier, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, je vous demande chers collègues de voter cet amendement merci. L'avis de la commission l'avis du gouvernement qui est identique favorable oui ben vont travailler oui et votre amendement est défendu l'amendement du gouvernement, là il est défendu,

merci madame. Il est défendu pour vous remercier d'avoir mis deux minutes supplémentaires, je voudrais me ramènera un petit maroilles a fini de 3 mois. Monsieur Corbizet je vous remercie beaucoup pour le maroilles, vous savez que on en produit aussi dans mon département, avis de la commission, merci l'avis du gouvernement : avis favorable pour la raison que j'évoquais tout à l'heure : avis favorable oui merci, donc je mets aux voix donc l'amendement 418 avis défavorable de la commission avis favorable du gouvernement qui est pour.

Nous allons passer à la mission suivante, voilà, et le temps que je que les ministres s'en aille, ça ça, chacun s'installe. Faire une petite annonce donc par courrier en date du 28 novembre Madame Éliane Assassi, présidente du groupe CRCE demandent l'inscription second point de l'ordre du jour de l'espace réservé à son groupe du mercredi 7 décembre de la proposition de résolution, présenté en application de l'article 34 1 de la Constitution pour le développement du transport ferroviaire acte et donner de cette demande et à la demande du groupe CRCE nous pourrions prévoir une discussion générale de 45 minutes de plus comme il est d'usage lors de l'examen des propositions de résolution les interventions des orateurs des groupes vaudront, explications de vote sur le texte. Y a-t-il des observations, je n'en vois pas, elle en est ainsi décidé. Voilà. Alors, l'ordre du jour appelle l'examen des crédits de la mission Santé et l'article 46 bis du projet de loi de finances pour 2023 et la parole est à monsieur Christian Klinger, rapporteur spécial de la commission des finances pour cinq minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, année après année, notre assemblée a émis des doutes sur la pertinence de cette mission santé déséquilibré entre l'aide médicale d'État, dont la maîtrise budgétaire n'est toujours pas assurée et un programme, prévention, sécurité sanitaire, peu à peu vidé de toute substance se résumant à des actions hétérogène et résiduelle de santé publique, un élément nouveau intervient cette année avec la création du programme recevant les crédits européens de soutien à l'investissement en santé, soit 6 milliards d'euros d'ici 2000 le suivi budgétaire de ces fonds s'en trouvera améliorée, mais cela ne redonne pour autant pour autant d'impact à la mission en termes de politique publique, beaucoup d'actions financées par la mission ont été transférés à l'assurance maladie au fil des années toutefois pour les besoins de la gestion de la crise sanitaire l'état il y a rapatrié depuis 3 ans dans un fonds de concours, près d'un milliard de crédits venant de santé publique France ces sommes n'ont jamais fait l'objet d'approbation parlementaire, que ce soit en loi de finances initiale ou en collectif budgétaire, il est souhaitable de mettre ces fonds de concours en extinction et de clarifier et stabiliser la répartition des missions entre l'État et santé publique France en matière de veille sanitaire et de préparation aux crises, cent quatre connaît peu d'évolution, je relève toutefois une diminution de la dotation versée à l'Oniam tenant compte de la sous-consommation des crédits d'indemnisation des victimes de la j'ai souligné dans le contrôle budgétaire effectué sur ce sujet un non recours significatif à ce jour, il pourrait néanmoins s'atténuer en dotant l'Oniam des moyens nécessaires pour diminuer les délais et résorber les retards dans le traitement des dossiers, la mission intègre les premiers effets budgétaires du transfert à la ne cesse de compétences aujourd'hui dévolu à l'agence de de sécurité du médicament en matière de cosmétiques et de produits de tatouage, cette réforme repose sur des constats d'étayer de longue date, il est donc discutable qu'elle intervienne sous forme d'amendements déposés tardivement dans le PLF. L'aide médicale d'État demeure l'élément principal de la mission Santé : le gouvernement propose pour 2023, une majoration de 133 millions pour l'AME de droit commun. Les crédits atteindraient 1 milliard 145 millions, soit une hausse de 13,2 % par rapport à la loi de finances initiale 2022, la commission des finances, a jugé cette augmentation étonnante et contestable à plus d'un titre, d'abord, elle se fonde sur une prolongation pure et simple de l'évolution tendancielle, observée avant la crise sanitaire, c'est-à-dire que le gouvernement table sur une poursuite de la progression du nombre d'étrangers en situation irrégulière, au moment même où il prépare son projet de loi précisément destinée à le réduire, c'est une contradiction difficilement justifiables, deuxièmement, le gouvernement nous a présenté il y a 3 ans, des mesures de contrôle et de lutte contre la fraude, il n'en résulte aucune inflexion du rythme d'évolution des dépenses doit-on en déduire que ces mesures sont inefficaces, dans ce cas, c'est qu'elles sont insuffisantes et qu'il faut les renforcer, mais rien n'est proposé dans ce sens, troisièmement le PLFR adopté il y a quelques jours, établi la prévision de dépenses d'AME de droit commun à 944 millions en 2022, c'est donc en réalité une augmentation de près de 200 millions et de plus de 20 pour 100 qui est proposé, alors même que l'État dispose désormais d'une créance sur l'assurance maladie qui pourrait atteindre 45 millions fin 2022 face à ce pilotage déficient et cette charge budgétaire non maîtrisée, la commission des finances propose de nouveau de revoir l'étendue des soins pris en charge par la haine et de réduire les crédits pour 2023 par l'éventail des soins couverts là mieux constitue par rapport aux pays voisins, une exception difficile à justifier dans la plupart d'entre eux seuls les soins urgents les soins liés à la maternité, les soins aux mineurs et les dispositifs de soins préventifs dans les programmes sanitaires publics sont prises en charge gratuitement pour les étrangers en situation irrégulière. C'est ce que le Sénat avait adopté il y a 2 ans, sur notre proposition et celle de la commission des affaires sociales, la commission des des finances propose donc l'adoption des crédits de la mission assortie de ces amendements. Merci beaucoup, cher collègue, la parole est à madame Annie Delmont Koropoulis, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales pour 3 minutes. Madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues, voilà au moins 3 ans que la commission des affaires sociales, déplore le caractère à la fois hétéroclite chétif, sur le plan financier, et en définitive il aux enjeux sanitaires de la mission santé du PLF. En 2023, les crédits de la mission progresseront de 100 59 %, mais cette hausse ne s'explique que par la création d'un nouveau programme, doté de 1,93 milliards d'euros et Servent de simple Canal budgétaire ad-hoc pour faire transiter jusqu'en 2000 26 le soutien européen aux dépenses d'investissement Ségur la politique sanitaire n'gagne a pris, a priori pas grand-chose car pour le reste, les changements sont minces, les crédits de prévention sanitaire du programme 204 augmentent peu et le programme contribue de manière toujours aussi résiduel et hétérogène au financement des agences de santé et de la politique de prévention difficile dans ces conditions d'évaluer la sa contribution aux objectifs qu'il se fixe et au moyen d'indicateurs aussi disparates que ce qu'il retient quant aux crédits consacrés aux actions contentieuses il diminue de 11 millions d'euros, ce qu'il dit simplement l'ampleur du non-recours au mécanisme d'indemnisation des victimes de la dépakine ou l'incapacité à chiffrer l'impact financier de l'indemnisation des victimes de la campagne de vaccination contre le Covid 19. Appuyons-nous pour mieux anticiper sur les rapports rendus sur ce chapitre par nos collègues de la commission des finances et de l'OPEX, l'essentiel de la hausse des crédits de la mission à périmètre constant, s'explique par celle des dépenses de l'aide médicale de l'État qui atteindront 1,14 milliards d'euros en 2023 par le retour à la dynamique de dépenses antérieures à la crise sanitaire, c'est pourquoi nos collègues de la mission des finances ont adopté cette année encore l'amendement du rapporteur spécial Christophe qui recentre l'AME rebaptisé aide médicale de santé publique sur un noyau des dépenses d'urgence et aligne ainsi son périmètre sur celui du dispositif équivalent en Allemagne, la commission des affaires sociales, il y a vu elle aussi un bon moyen de recentrer le dispositif sur son objectif humanitaire et sanitaire, elle propose seulement de le compléter par la création d'un programme de soutien aux personnes en situation irrégulière, afin de leur proposer des examens de prévention et de dépistage, je le vois en Seine-Saint-Denis, en tant que parlementaire, mais aussi depuis des décennies en tant que médecin, et les élus d'Aubervilliers qui sont en tribune en témoignerait également les bénéficiaires potentiels de l'AME sont par hypothèse en situation précaire, leur état de santé est fragile, ils sont en outre la proie des dealers, il faut les protéger activement de ce fléau dans l'intérêt de tous, Merci, cher collègue. la parole est à Monsieur Daniel Chassain pour le groupe, les indépendants pour quatre minutes. Madame la présidente, madame la ministre, madame le rapporteur monsieur le rapporteur de la commission des finances, mes chers collègues, la crise sanitaire que nous tu as heure traversons un mis sous une lumière crue toute l'importance du secteur sanitaire, nous manquons d'infirmières, d'aides-soignantes, qu'il faut former massivement avec des IPA la suppression du numerus clausus la quatrième année, ne vont pas permettre d'augmenter le nombre de médecins avant plusieurs années, la mission de santé examiné aujourd'hui concerne 3 programmes le 379 avec 1 virgule 9 milliards d'euros concerne simplement un canal budgétaire pour la compensation de la sécurité sociale par des crédits européens pour des investissements en santé, le but, en fait, la mission c'est de programme le 204 avec 313 millions d'euros augmente de 1,6 % pour la prévention sanitaire maladies chroniques environnementale nutrition l'indemnisation amiable, lutte contre le tabac, indemnisation. Des. Modernisation des hommes de soins évaluation sur le dépistage colorectal et mais c'est surtout le programme 183 consacrée à l'aide médicale de l'État, ce dispositif est destiné à financer les loin des immigrés, des soins des immigrés en situation irrégulière, ils nous honore en 2023 les crédits qui sont alloués pro-progresse de 13 % c'est 1,14 milliards d'euros que nous concitoyens mon consacré à soigner les personnes en situation irrégulière sur le territoire français, le périmètre des soins remboursés plus large actuellement doit revenir sur ce qui se fait dans les pays voisins pendant les 3 premiers mois, nous devons recentrer les admissions sur les traitements et il m'a dit grave des soins d'urgence et prophylaxie des maladies graves, les grossesses c'est le dispositif humanitaire pratique en Allemagne et dans les pays voisins, d'autre part, certains patients proviennent parfois des pays du G20 n'habite pas en France depuis 3 mois, non pas de pathologie d'une extrême d'une exceptionnelle gravité et, souvent, hé bien le traitement pourrait être réalisé dans leur pays, c'est pris en charge se font dans le cadre d'une procédure d'admission au titre de séjour pour soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et se dix pousse dispositif est largement, largement, nous devons aussi contrôler les fraudes à l'identité aux ressources à la résidence, je soutiens l'amendement de Madame le rapporteur concernant l'attribution de crédits dans des actions mobile de prévention pour les personnes qui en ont besoin dans le cadre de maraudes notamment l'augmentation du nombre de bénéficiaires de 350 60 35000 en 2020, ils sont de 400000 environ en 2022, les mesures de 2019 comparution physique pour la demande en CA PAM Dédé d'ancienneté ont été supprimé pendant le Covid, il faudra y associer à mon avis, les maisons de France service car les CPAM sont parfois éloignées des populations, l'investissement de long terme en matière de sensé de santé doit rester notre priorité en ce qui concerne l'humanisme, nous devons rester comme l'indique Madame le rapporteur a des notions d'urgence pendant les 3 premiers mois, le groupe des indépendants, on votera donc en faveur de son adoption, merci. Merci beaucoup, la parole est à Madame Raymonde Poncet mon pour le groupe écologiste solidarité territoire pour quatre minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues, l'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité les mesures contenues dans ce projet de loi de finances dans la continuité du PLFSS monte que nous n'empruntons pas totalement le chemin de cet objectif sur le bien-être physique en France à l'heure du risque d'effondrement de l'hôpital et des zones sous-dotées en offre médicale, une part importante de Français renoncent à des soins médicaux, les maladies chroniques progresse, les indicateurs de périnatalité reste préoccupant : la santé mentale est en berne, et dans ce contexte, les crédits de la mission santé augmentent de seulement 4,2 je renvoie à l'inflation, en effet, l'augmentation de 100 59 % des crédits et liée à l'intégration du programme 379 qui reverse des crédits européens à mesure que les délais d'attente pour obtenir des rendez vous s'allonge avec ses pertes de chance, les délais pour que vous preniez les réelles mesures structurelles pour s'attaquer aux déterminants sociaux et géographiques des inégalités de santé s'avère tout aussi long, en effet, s'agissant du bien-être social, les fractures sociales et territoriales sont criantes fracture reflétée dans les finances, le budget de l'Action santé des populations dont l'objet est de corriger les inégalités de garantir pour tous les meilleures chances face à la maladie taille représentant 0 6 % du programme programme prévention sécurité sanitaire et offre de soins, lui-même sous-dotées, selon l'adresse pourtant de la naissance au grand âge, les problèmes de santé évoluent mais les inégalités demeurent à titre d'exemple, la part de personnes souffrant d'obésité diminue lorsque le niveau de vie ou de diplôme augmente et les femmes résidant dans les Drom présente un risque de mortalité maternelle multiplié par 4 par rapport à celles vivant en hexagone quant au bien-être mental je renvoie aux aux manifestations d'aujourd'hui: la santé mentale est au PLF ce que la psychiatrie est à la médecine, c'est-à-dire le parent pauvre des crédits de la mission santé. Tandis que le coût annuel Direct et indirect des troubles psychiques est estimé à 109 milliards d'euros, le PLF réserve à la santé mentale, une sous-action doté d'un 1000000 d'euros environ, soit une part infime des crédits de la mission, nous demandons au gouvernement de lancer enfin un plan d'urgence pour la psychiatrie enfin quant au budget de l'AME. Vient, il peut être de rappeler qu'ils ne représentent que 0,5 des dépenses de la maladie, et je vous demande cette fois cette focalisation de quoi est-elle le nom nous défendons, nous, à l'inverse, dans une logique de solidarité et aussi de santé publique, le retour aux conditions d'attribution de 2020, soit la fin du délai de résidence de 3 mois, les moyens dévolus à la mission santé reste insuffisamment ambitieux et notamment ceux dévolus à la santé globale à la prévention et surtout à la réduction des déterminants sociaux et territoriaux et territoriaux des inégalités de santé, c'est pourquoi le groupe écologiste solidarité et territoires, votera contre, je veux, c'est le budget de cette mission, je vous remercie. Merci, la parole est à monsieur Xavier Iacovelli pour le groupe Rassemblement des démocrates. Progressistes et indépendants pour quatre minutes. madame la présidente, madame amis chers collègues, la mission Santé traduit les engagements de l'État à développer la politique de prévention, assurer la sécurité sanitaire et organiser une offre de soins de qualité à toutes et à tous sur les territoires ou de la de la ligne budgétaire au-delà des chiffres, et par la mission comporte en son coeur une politique de solidarité qui nous est propre, l'aide médicale d'État, pour rappel, près de 300000 personnes bénéficiaient de l'AME de droit commun. En offrant également à ses bénéficiaires un accès aux soins de ville là elle me permet la prise en charge en amont des pathologies et évite ainsi les surcoûts liés à des soins retardés et pratiqués dans l'urgence, je souhaite souligner, mes chers collègues, quand, de 2000 19 et 2020, parallèlement aux actions menées en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, le gouvernement a mis en place des mesures pour réguler les dépenses et renforcer les contrôles dans le cadre du programme ciblé, si toutefois le périmètre de cette mission est assez limitée, elle comprend 3 programmes qui acte la solidarité de l'État et sa politique en matière de prévention, les exercices 2020, 2021 et 2022 ont été fortement marquée par la gestion de la crise de la Covid 19 mai 2023 devrait constituer une année charnière, notamment au regard des événements sportifs attendus fin 2023 qui justifie des réflexions pour anticiper des mesures de prévention à mettre en oeuvre les crédits de cette mission devrait donc continuer à être mobilisés au moins jusqu'au 1er semestre 2023 sur la gestion de la crise sanitaire et de ses impacts les crédits de la mission s'élève donc à 3,36 milliards, soit une hausse de 2 milliards par rapport à 2022, une hausse due à l'ajout des crédits dans le cadre du plan national de relance de résilience, il permettra à l'État de reverser à la sécurité sociale, les crédits européens perçu dans le cadre du plan de au titre au titre du financement des dépenses d'investissement dans les établissements de santé et médico-sociaux. Une hausse, conséquence des crédits est également visible concernant la sécurité sanitaire, plus 124 % par rapport à 2022 ces crédits permettront de poursuivent des objectifs en matière de veille de prévention des risques ou encore de gestion des crises cette mission santé tire donc en quelque sorte les leçons de la crise sanitaire et nous donnera donc les moyens adéquate pour préparer l'avenir, d'autre part, cette mission met également en avant la santé de la mère et de l'enfant via le financement du au profit d'associations jouant un rôle dans le domaine périnatale ces crédits viseront également à la à améliorer la prévention des troubles sensoriels et après et des apprentissages, mais aussi d'améliorer et de promouvoir la qualité de l'accueil des enfants malades en milieu intra et extra hospitaliers en France, plus d'1 virgule 1 1000000 de personnes sont atteintes de maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, selon les dernières estimations de l'Agence nationale de la santé publique et il existe plus de 2 millions d'aidants, soit au total plus de 3 millions de personnes concernées dans ce contexte, la prévention des maladies chroniques et la qualité de vie des malades représentent 24 % des crédits alloués et vise notamment au financement de l'Institut national du cancer pour quarante-cinq millions de la prévention des addictions des maladies neuro-dégénératives et des maladies liées au vieillissement, c'est un axe majeur pour prévenir le plus tôt possible, les complications de santé tout au long de la vie cette action comprend également des crédits dédiés à la santé mentale, un 1000000 d'euros afin de soutenir les acteurs associatifs, celle-ci doit être intensifiée, compte tenu de l'altération de la santé mentale de la population, suite à la crise de la Covid, et notamment chez les jeunes, il en va de l'avenir de de notre jeunesse dans la continuité du PLFSS cette mission donc suit la ligne de la prévention de la solidarité et du soutien des politiques publiques aux associations qui oeuvrent chaque jour aux côtés de ceux qui sont en difficulté et pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera cette mission. merci beaucoup, la parole est à monsieur. Bernard Jomier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour six minutes. Madame la présidente, madame la ministre avait rapporteur, mes chers collègues, nous étudions maintenant la mission santé du PLF, hein, qui est une mission au périmètre limité, nous allons dire et nous sommes pour notre part, convaincus qu'elle doit être conservé que le périmètre de l'action de l'État en la matière de doit d'ailleurs être repensée dans ses missions dans ses moyens, tant dans le domaine financier quand derme de gouvernance et de prévention s'il n'y a plus grand chose dans cette mission, c'est parce que l'État, délègue toujours davantage la politique de santé à l'assurance maladie, c'est le cas notamment des transferts financiers, c'est le cas de la dette Covid par exemple qui est pour son intégralité maintenant par les crédits de l'assurance maladie. Ne nous égarons donc pas ce budget qui est en augmentation de 2 fois et demie du montant de l'année précédente, est dû à à l'intégration du programme 379 qui permet à l'État de reverser à la sécurité sociale et crédits européens perçu dans le cadre du plan de relance, cela n'a donc aucune influence sur les politiques publiques portées dans le cadre de la mission, la mission de 4 elle prévention sécurité sanitaire et de soins est en augmentation par rapport à 2022 depuis le début de la crise sanitaire, elle sert de support indirect à la gestion de crise, avec par exemple l'achat de matériels ou de systèmes d'information, la commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques du Sénat a par ailleurs relevé que cette mission consacré des montants importants au paiement des cabinets de conseil, cette augmentation budgétaire n'apporte donc en ce début de quinquennat pas de nouvelles dispositions importantes, par ailleurs, nous sommes particulièrement déçu de l'absence totale de politique de prévention dans ce budget de l'État, le texte ne comporte que peu de programmes spécifiques et pas de hausse que de crédit significatives en faveur d'un programme de prévention et nous en sommes d'autant plus déçu qu'avant la publication du texte sur le PLFSS nous avions quelques espoirs en la matière, les propos du ministre de la santé, de porter un virage de la prévention avait recueillir recueille toujours notre soutien et nous aurions accueilli avec bienveillance, toutes les mesures fortes en la matière, mais c'était sans compter sur l'arbitrage politique du et du ministre des Comptes publics qui s'inscrit dans la lignée habituelle et non exceptionnel, des ministres portant une politique de contraintes sur le système de soins. Alors que la crise Covid est passé par là, nous pourrions dressé une longue liste des sujets manquants en matière de prévention mais nous nous limiterons à la santé environnementale qui depuis 2016 a inscrit dans la loi, a fait l'objet de nombreux travaux. Et nous ne voyons toujours aucune disposition du gouvernement en la matière, comme il n'y a d'ailleurs quasiment rien sur la psychiatrie et la santé mentale. mentale. Concernant les agences sanitaires nous regrettons toujours que l'Agence nationale de santé publique soit financé par la Sécurité sociale depuis tout son transfert au suspects opéraient dans la loi de finance de la Sécurité sociale en 2020 les missions de sécurité sanitaire et de gestion de crise dévolu à cette agence nous le rappelons sont des missions régaliennes qui exigent un retour dans le budget de l'État, par ailleurs, fallait-il créer fin octobre une énième agence une nouvelle agence, celle de l'innovation en santé pour accélérer la mise sur le marché des innovations françaises. Il existait une mission ministérielle avec deux. Personne 2 équivalents temps plein, mais ces personnes en d'âge il alors pas été transférés à l'agence, allons nous maintenir et accroître le mille-feuilles en la matière, cette agence, un pur produit d'un système de gouvernement qui n'est pas efficient parce qu'il multiplie les agences en organisant la confusion des rôles et des missions, j'en viens au programme 183 à l'aide médicale d'État, tous les ans et nous le regrettons, c'est un sujet qui est l'objet de posture et nous en débattrons lors de l'examen des amendements cette année les portes, les crédits sont portés à 1,14 milliards d'euros, je vous invite mes chers collègues, à vous pencher sur les raisons de cette augmentation, qui réside pour une large part dans la hausse du recours à l'hôpital et par ailleurs, quand on regarde le nombre de délivrance de titres de séjour sa diminution drastique dans notre pays, de facto, et immédiatement entraîne un accroissement des donc ces personnes qui relève de l'AME et non pas des dispositifs de l'assurance-maladie les mesures restrictives en la matière sont à contre-courant, l'installation, l'instauration d'un délai de carence de trois mois pour la c'est à la Puma des demandeurs d'asile ne fait qu'accroître la gravité des soins pris en charge et par ailleurs l'accès aux soins des étrangers en situation régulière et de plus en plus compliqué l'AME, mes chers collègues, ce n'est pas un outil de la politique migratoire, c'est un outil de santé publique et du reste, les tentatives de contrôle des montants par cette approche de politique migratoire sont vouées à l'échec, comme l'a constaté : la commission des finances, il serait plus fructueux à tous égards, de confier le régime d'aide médicale d'État à l'assurance maladie pour le coup, pour ces raisons, si les crédits de l'AME était maintenu et que s'instaurer un dialogue foutu E sur ces amendements, nous pourrions voter les crédits de cette mission, la suite nous le dira ce qu'il en fera, je vous remercie. Merci, la parole est à madame Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour quatre minutes. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, les lien intrinsèque entre la mission Santé le budget de la Sécurité sociale se retrouvent au sein du nouveau programme 379 simple canal budgétaire qui prévoit le financement par l'Union européenne des dépenses d'investissement dans les établissements de santé, médicaux, sociaux, suite à la pandémie du Covid 19 et qui constitue l'essentiel des crédits de cette mission concernant le programme 204 consacré à la prévention, la sécurité, Sana sanitaire et l'offre de soins qui vise à améliorer l'état de santé général de la population dans un souci de réduction des inégalités sociales, des inégalités, nous regrettons que le budget ne progresse que de 1,6 pour 100, car comme le souligne Cyrille Delpierre, directeur de recherche à l'INSERM, je cite, en France, on considère qu'il y a 13 ans d'écart entre l'espérance de vie des 5 % les plus riches et celle des 5 % les plus pauvres le PLF 2023 prévoit une baisse de crédits pour le pilotage de la politique de santé publique de 3 0 5 % et aucune évolution des crédits pour la réduction des inégalités de santé comment prétendent y parvenir avec en réalité des moyens en diminution, compte tenu notamment de l'inflation, nous avions espéré que le changement d'intitulé du ministère de la Santé, désormais, ministère de la Santé et de la prévention s'accompagne d'une politique ambitieuse en matière de prévention mais ce ne sont pas les 216 millions d'euros en 2023 qui permettront d'agir véritablement pour réduire les inégalités sociales, territoriales environnementales, de santé concernant les crédits du programme 183 sur la protection maladie je veux rappeler ici, notre proposition de loi déposée au mois de juin 2022, qui vise à intégrer le budget de l'aide médicale d'État dans le budget de la Sécurité sociale plus exactement de réintégrer les personnes étrangères dans le régime général de la Sécurité sociale, comme cela a été le cas avant la loi Pasqua du 24 août 1993 qui a rompu avec la logique universaliste de la sécurité sociale en subordonnant le droit à l'assurance maladie des étrangers à la régularité de leur séjour, la fusion de l'AME dans le régime général de la Sécurité sociale est demandé par les associations de de l'Observatoire du droit à la santé des étrangers mais également par le Conseil économique et social, le conseil national du SIDA, le Conseil national de politique de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et même l'inspection générale des finances et des affaires sociales, nous regrettons que chaque année, la droite fasse la courte échelle à l'extrême droite à l'occasion du débat sur la M pour réduire les dépenses des étrangers qui ne représente pourtant que 0 5 % des dépenses de santé, les 2 amendements du rapporteur Klinger illustrent malheureusement cette volonté la santé est un bien commun mondial et aujourd'hui les associations subissent déjà les réformes de l'aime, qui ont réduit l'accès aux prestations et considérablement complexifier les procédures, enfin je souhaite dénoncer ici l'attitude du groupe Sanofi qui refuse de financer l'indemnisation des victimes de la dépakine en épuisant l'ensemble des voies de recours juridictionnel pour contester sa responsabilité Sanofi occasionne d'importants frais de justice qui endette l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, ce qui est parfaitement scandaleux, le gouvernement doit a minima suspendre le versement du crédit impôt recherche à titre préventif pour contraindre Sanofi d'assumer sa responsabilité auprès de l'ensemble des victimes en conclusion les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE voteront contre les crédits de la mission Santé qui demeure cette année encore largement insuffisant, je vous remercie. Madame la présidente, monsieur, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, quand nous sommes jeunes, nous dépensons notre santé, pour se faire une fortune et quand nous sommes vieux nous dépensons notre fortune pour se faire une santé, je tiens à remercier notre collègue rapporteur madame Annie Delmont Koropoulis pour la qualité de son avis, qui éclaire avec précision les crédits de la mission Santé dans le PLF pour 2023 je ne fais que confirmer les résultats de son analyse la trajectoire des crédits de la mission santé est en hausse sur 2023 2025 en 2023, les crédits de la mission passeront de 1 virgule 3 à 3,36 milliards d'euros, principalement en raison de la création d'un nouveau programme 379 doté de 1,93 milliards d'euros, ce programme permet de reverser à la sécurité sociale des crédits européens perçu dans le cadre du plan de résilience type de financement des dépenses d'investissement dans les établissements de santé et médico-sociaux, ces crédits sont destinés à couvrir les coûts des doses de vaccins aux pays étrangers à soutenir le volet investissement Ségur du plan de relance français ce programme spécifique améliorer la traçabilité du suivi des fonds européens Servent de simple canal de transmission à l'assurance maladie, il ne redonne toutefois aucune substance particulière à la mission en termes de mise en oeuvre d'une politique publique le programme 183 porte 1 virgule 22 milliards d'euros de dépenses d'aide médicale d'État, le nombre de bénéficiaires continuent d'augmenter le PLF 2023 garantit l'accès aux soins des étrangers en situation irrégulière il nécessaire de prévenir les risques de détournement du dispositif et de renforcer et développer les mesures de lutte contre la fraude, tout en favorisant l'accès aux soins des plus vulnérables, le régime de l'AME constitue une exception en Europe, la plupart des pays voisins, ne prenant en charge gratuitement pour les étrangers en situation irrégulière, qu'un éventail de soins comprenant les soins urgents les soins liés à la maternité des soins aux mineurs et des dispositifs de soins préventifs dans des programmes sanitaires publics nous soutenons l'amendement de la commission des finances Résizon le montant de l'aide médicale d'État, pour tenir compte de sa transformation en une aide médicale de santé publique, comparables à celles en vigueur dans les principaux pays voisins les sénateurs du groupe Union centriste sont favorables également à l'amendement de la commission des affaires sociales portant sur la création d'un nouveau programme consacré au financement d'actions conduites par l'État, l'assurance maladie et les associations, notamment dans le cadre de maraudes d'équipes mobiles de prévention ou encore de barnomes, de dépistage, ces dispositifs sont destinées à proposer aux personnes en situation irrégulière, des examens de dépistage et à les sensibiliser à la nécessité de solliciter le dispositif de l'aide médicale de santé publique, le programme de 104 consacrent 213 millions d'euros à la prévention à la sécurité sanitaire et à l'offre de soins mais ne contribue plus qu'au financement de 2 agences sanitaires, l'institut, l'institut national du cancer et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail des moyens supplémentaires sont prévus pour financer des systèmes d'information, notamment les outils numériques pérenne pour améliorer la veille et d'anticipation des situations de crise, il s'agit notamment de financer le lancement de certains chantiers tels l'entrepôt national de données de biologie médicale, la politique de santé bénéficie en 2023 d'une hausse des financements pour soutenir plusieurs actions de prévention dont le plan de chlordécone le plan national santé environnement la stratégie nationale de l'Alimentation, de la nutrition et du climat, la santé sexuelle, la prévention des addictions toutefois ces actions hétérogène et extrêmement présente un impact limité sur la réalisation des objectifs de santé publique poursuivi en matière de prévention je souhaiterais aborder 2 points détection précoce des cancers et dégradation de la santé des hospitaliers, d'abord, je souligne l'importance de l'information au sujet du cancer de la prostate qui entraîne des décès qui pourraient être évités avec plus de 50 mais nouveaux cas par an en France, ce cancer est de plus plus fréquent chez l'homme, le dépistage anticipée permet une diminution de 41 % du risque de cancer métastatique, évitant ainsi l'aggravation de la maladie et les chimiothérapies traumatisante, il est essentiel de renforcer des campagnes d'information et des mesures de sensibilisation en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein au cours de l'année 2021 2 7 millions de femmes ont effectué une mammographie de dépistage organisé, ce qui correspond à un taux national de participations de cinquante c'est-à-dire ensuite la réalité de la santé des hospitaliers nous inquiète vivement, chers collègues, l'hôpital a tenu est une phrase que l'on entend souvent si l'hôpital tiens c'est bien grâce aux hospitaliers, or ceux-ci apparaissent à bout de souffle, une étude menée par la MNH, en partenariat avec la chaire Santé de Sciences Po met en exergue un état de santé physique et mentale dégradé, notamment par rapport au reste de la population pour les hospitaliers d'exercice professionnel constitue une source de détérioration de leur état de santé, il devient urgent de prendre soin des femmes et des hommes qui prennent soin de nous puisque prendre soin de sa santé ne change pas l'issue, mais le trajet pour reprendre les mots de Niamey il nécessaire de déceler les axes prioritaires potentiellement efficace, l'amélioration des conditions de travail, la libération du temps consacré aux démarches administratives, le soulagement des professions en tension autant de leviers pour réduire la souffrance forte continue mais désormais profonde qui atteint les hospitaliers, la mission Santé vise en principe à développer la stratégie de prévention, assurer la sécurité sanitaire et organiser une offre de soins de qualité dans tous les territoires et sénateurs du groupe Union centriste regrette néanmoins le caractère inadapté de cette mission aux objectifs et aux enjeux sanitaires, ce qui rend difficile toute évaluation en conséquence, le gouvernement doit entamer une réflexion pour élaborer une vision stratégique à long terme, il est temps d'organiser l'action et de la financer, autour d'une politique sanitaire fondée sur la prévention, chers voilà, en dépit de ces remarques en espérant. Que même entendu oui, merci beaucoup, je vais passer la parole à Madame Catherine Bell Rithy que le groupe les Républicains pour cinq minutes. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. La dotation du PLF 2023 pour la mission Santé connaît une croissance de près de 100 59 % par rapport à 2022 qui s'explique par le coût de la gestion de la crise sanitaire et il faut le souligner un important investissement santé pour les 6 prochaines années, or de ce dernier programme, donc, qui n'est qu'un simple canal budgétaire, les crédits de paiement de la mission connaissent une hausse de 11 % par rapport à la loi de finances initiale de 2022, le programme de prévention et de sécurité sanitaire ne connaît pas d'évolution majeure et il faut souligner que le fonds de concours initialement créé pour prendre en charge les dépenses liées à la crise sanitaire devrait s'éteindre à la fin de cette année, la hausse de la mission Santé et donc particulièrement par celle des crédits de l'aide médicale de l'État qui est de 13 % par rapport à 2022, il faut aller au fond des choses, à ce sujet et les évoquer avec clarté, ces dépenses sont essentiellement liées à l'AME de droit commun, cette dernière bénéficie aux étrangers en situation irrégulière résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. L'AME de droit commun prévoit dès lors une prise en charge intégrale des soins médicaux et hospitaliers sans avance de frais dans les limites des tarifs de la Sécurité sociale, or les chiffres de l'me blesse, il baisse d'abord le budget de l'État puisque la ne représentait que 139 millions d'euros lors de sa création en 1999, elle est ensuite passée de 772 millions en 2016 à plus d'un milliard en 2023. Et pour cause, le système français d'accès aux soins des étrangers en situation irrégulière et l'un des plus généreux de l'Union européenne. Qu'en déduire sinon que cette dépense est devenue incontrôlable non maîtrisée, comme l'ont très justement dit. Comme l'a très justement dit pardon, ma collègue Annie Delmont Koropoulis ces chiffrent blesse plus encore l'acceptabilité sociale du budget de l'État, les débats de société directement corrélée à ce budget relatif à l'accueil, à la gestion des personnes étrangères en situation irrégulière se répète pourtant et, plus encore que les dispositifs législatifs, c'est l'efficacité exécutive qui interroge à cet égard, il ne s'agit pas ici de faire resurgir, d'autres sujets, mais simplement de les rappeler les chiffres, le nombre des bénéficiaires de l'AME de droit commun était de 150000 en 2002 il est désormais de 400000 près de 80 % d'entre eux sont présents sur le sol français depuis plus de 3 ans, une situation irrégulière peut-elle être à durée indéterminée. Et le rapport fait par notre collègue Christian Klinger de conclure avec une clarté Adam Antin que ce nombre ne fera qu'augmenter à un rythme quasi exponentielle, si aucune réforme n'est entreprise. Comment faire supporter à nos concitoyens les conséquences aveugle d'une articulation erratique entre politiques publiques et d'une réforme de l'AME jusqu'à présent repoussé ces constats force l'adoption de réformes urgentes car, comme les rapporteurs précitée, l'ont rappelé les effets des mesures adoptées jusqu'à présent n'ont été qu'un qu'un certain en matière de régulation des dépenses est insuffisant en matière de lutte contre la fraude. Les rapports des commissions préconisé, il est d'abord nécessaire de recentrer la AME sur les soins urgents comme le font les autres pays d'Europe, il apparaît ensuite nécessaire d'exclure du panier de soins, certains gestes médicaux et certains traitements de maladies non grave dans le prolongement des amendements déposés cette année l'amendement proposé par la commission des finances à ce sujet revêt une importance décisive dont il faut remercier nos collègues et qu'il faut soutenir l'aide médicale d'État se comptent désormais en milliards, l'État doit cesser de se comporter en payeur aveugle, je vous remercie. Merci. Alors je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 21 heures 35 pour la suite de l'examen de la mission Santé la séance est suspendue.